du projet de loi relatif à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen, élu en France aux élections de 2019. Acte et donner de cette demande, la commission des Lois se réunira pour examiner le rapport et le texte, le mercredi 15 mai matin le délai limite de dépôt des amendements de séance sur ce texte pourrait être fixée à l'ouverture de la discussion générale et la réunion de la commission pour l'examen des amendements soutient Brett, à l'issue de celle-ci, y a-t-il des observations. Il en est ainsi décidé j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française et du projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, ont été publiés ces candidatures seront ratifiées c'est la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement, l'ordre du jour appelle le débat sur la zone Euro, demandé par le groupe, les républicains, nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents, je vous rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de 8 minutes, puis le gouvernement répond pour une durée équivalente, la parole est tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat monsieur Jean-François Rapin pour le groupe, les républicains pour 8 minutes je vous en prie.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, portée sur les fonts baptismaux le 1er janvier 1999, la monnaie unique fête cette année le 20ème anniversaire d'une existence particulièrement mouvementée, en effet, nous ne pouvons oublier la crise mondiale de 2008 2009 et plus encore la crise des dettes souveraines, propre à la zone Euro en 2011, 2012, depuis lors, beaucoup a été fait pour renforcer ce pilier de la construction européenne, y compris grâce à l'action décisive de la BCE dans des moments critiques et régler certains problèmes structurels gras sur et à une réforme menée entre 2010 et 2012, les débats sur la légitimité, l'orientation, la cohérence ou la solidité de l'Union économique et monétaire n'ont toutefois jamais cessé. Les leçons de la dernière campagne présidentielle ont été retenus et leur à ce le rassemblement national avancent désormais masqués sur son projet de suppression de l'Euro, auquel les Français, vous le savez sont minces Mons massivement opposés, s'il y a 2 ans à peine, Marine Le Pen ne jurait que par le retour au franc et la dévaluation, l'objectif est aujourd'hui euphémiser est renvoyé à un calendrier plus lointain, nous savons tous que la fin de l'Euro se traduirait immanquablement par une nouvelle explosion de notre dette, un profond taper affaiblissement de notre économie et au final un appauvrissement général des Français. De l'autre côté du spectre, le président de la République, vous serez moins d'accord, Monsieur le Ministre propose quant Ali l'exact inverse l'exact inverse, soutenant que l'avenir de la monnaie unique sera fédérale ou ne sera pas sa proposition phare : créer un budget autonome de la zone Euro équivalent à plusieurs points de PIB, soit un montant se chiffrant en centaines de milliards d'euros comme on pouvait s'y attendre ces ambitions ont été rapidement douché et ont reçu une fin de non-recevoir cinglante de la part de plusieurs États-membres ainsi qu'un soutien aussi timide qu'ambigu de notre partenaire allemand, car si le principe d'un instrument budgétaire spécifique a bel et bien été actés par le Conseil européen, son volume sera sans doute dérisoire par rapport au souhait du président de la République surtout son rôle devrait se concentrer sur la convergence et la compétitivité, ce qui est essentiel, en excluant toutefois la fonction de stabilisation qui constituaient le coeur de la proposition présidentielle cet échec annoncé était largement prévisible, Emmanuel Macron, pouvait-il en effet ignorer que la crise de la zone Euro en grande partie, nourrie par les politiques irresponsables de certains États-membres avait laissé des marques profondes et que dans ce contexte, les solutions, appelant à une mutualisation des risques financiers sont vouées à l'échec sans ce préalable indispensable le retour de la confiance mutuelle entre partenaires, or la politique menée par le gouvernement depuis 2 ans on ne resteront pas la crédibilité économique de la France ne saurait permettre le rétablissement de cette confiance, les réformes structurelles nécessaires à la remise en ordre de notre économie, ont certes été promise mais n'ont pas été entreprise où étaient conduites à minima. De surcroît, notre trajectoire budgétaire comme celle d'ailleurs de l'Italie demeure le plus puissant des arguments contre toute union de transferts, le gouvernement a ainsi déjà fait une croix sur son objectif de retour à l'équilibre en 2022, à rebours de la quasi-totalité de nos partenaires de la zone Euro qui l'ont déjà atteint, on s'en rapproche très rapidement alors que le déficit moyen de la zone Euro devrait s'établir aux alentours de 06 pourcent du PIB pour 2018, celui de la France reste encalminé à 2,5 pourcent et devrait même atteindre 3,1 pourcent l'année prochaine, quant à notre déficit structurel et à notre dette il n'enregistre aucune baisse dans le même temps, la dépense publique continue de s'accroître inexorablement avec un immeuble avec un niveau de 56 pourcent du PIB, elle reste supérieure de 12 points à la moyenne des autres membres de la zone Euro. Cette voie n'est pas soutenable, elle ne fait qu'accroître au niveau national, les risques que le président de la République entend mutualiser au niveau européen et face à l'aléa moral qu'il représente le fédéralisme budgétaire prônée par Emmanuel Macron s'apparentera pour un temps sans doute encore long à une impasse politique. D'autres moyens plus pragmatiques doivent donc donc être mis en oeuvre pour renforcer la résilience de la zone Euro et la convergence en son sein la première des clés restent nationale l'Europe n'a pas vocation à se substituer aux États pour régler leurs problèmes économiques à leur place, et c'est à chacun d'entre eux qu'il appartient de prendre ses responsabilités, cette orientation générale dans le dans le maître mot n'est pas l'austérité, mais l'équilibres servi servirait en outre l'objectif d'une plus forte coordination économique d'ensemble et pourrait par exemple inciter davantage les États excédentaire à dépasser leurs réticences et à mobiliser leurs marges de manoeuvre pour soutenir leur propre croissance, et celle de la zone Euro, d'un point de vue institutionnel, le dire, il le directoire politique aujourd'hui organiser de manière temporaire ou à l'échelle des ministres et non des chefs d'État doit pouvoir être pérennisé, afin d'oeuvrer davantage au pilotage économique de la zone Euro dans cette optique, il est nécessaire d'impliquer les parlements nationaux dans le cadre de ces discussions, les conditions seront alors réunies pour que leur coordination économique de la zone Euro se penche également sur la nécessaire mise en place d'un mécanisme de convergence des règles relatives au marché du. Travail et aux systèmes sociaux ainsi qu'aux systèmes fiscaux appliqués aux entreprises les avancées dans ces domaines ne se feront sans doute pas d'emblée à 19, n'hésitons pas à leur amener ce travail avec un groupe peut-être plus restreint d'États membres le récit de le récent traité d'Aix-la-Chapelle, a affiché de hautes ambitions en la matière, nous attendons maintenant leur concrétisation gardons enfin à l'esprit que les mécanismes privés de partage des risques, qui passe par l'intégration des marchés bancaires et financiers nationaux sont aussi important et efficace que les mécanismes publics en cours de discussion. Qu'il s'agisse du budget de la zone Euro, ou des évolutions bienvenues du mécanisme européen de stabilité, en effet, la fragmentation persistante du secteur bancaire et financier pose des inconvénients majeurs qui sont au coeur des débats sur la zone Euro, elle a tenu la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle, elles alimentent le cercle vicieux de la contagion entre risque bancaire et risque souverain, elle renforce la polarisation des activités économiques, ce qui entrave le processus de convergence, elle freine enfin la mobilité des actes, des capitaux et le recyclage de l'excédent d'épargne des pays du Nord 340 milliards en 2018 en investissement pour ceux du Sud, enfin elle empêche la diversification des risques privé, qui joue pourtant un rôle essentiel dans l'absorption chocs asymétriques. On estime en effet qu'aux États-Unis ce type de choc est amorti aux 3 quarts par le crédit bancaire et les marchés de capitaux, ce qui diminue d'autant la nécessité des transferts budgétaires fédéraux finaliser l'architecture de l'union bancaire et de l'Union des marchés de capitaux et avancer plus vite sur leur contenu technique doit donc à l'évidence constituer une priorité malgré des difficultés comme par exemple sur le front unique de garantie des dépôts ce chantier a surtout l'Avantage de faire l'objet d'un consensus politique de principe exempt de graves clivages de doctrine, ce qui est loin d'être le cas du fédéralisme budgétaire pour finir affirmer le rôle international de l'Euro est devenu un objectif incontournable : l'Euro et la 2ème monnaie mondiale, mais il ne concurrence pas suffisamment le dollar qui reste la devise de référence et qui constitue un formidable instrument de la puissance américaine, notamment lorsqu'il s'agit pour les États-Unis d'imposer leurs lois extraterritoriales. Pour s'affirmer dans la mondialisation, l'Europe doit désormais penser sa monnaie comme un outil stratégique et plus simplement comme ennemi un instrument facilitant le fonctionnement de l'économie, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les nuages de tous types s'amoncellent sur la croissance mondiale et européenne à cet égard, après avoir mené une politique monétaire accommodante et décisive pour soutenir l'activité économique en Europe, la BCE revoit aujourd'hui ses capacités d'action fortement amoindri la mobilisation doit rester forte face au défi de l'Euro et si c'est avant tout les États dans les États membres, que se joue l'avenir de l'économie européenne. Et de la monnaie unique des voies d'action collective existent, mais elles ne pourront être empruntés à une seule condition celle d'être avant tout pragmatique, je vous remercie. Merci Monsieur de sénateur, monsieur le ministre, ce Bruno Lemaire minutes. Faute de l'économie et des finances pour 8 minutes. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, d'abord vous remercier d'être venus nombreux pour ce débat fondamental sur la zone Euro. Je voudrais dire tout de suite aux sénateurs Jean-François Rapin, que je partage son constat de départ. Et son ambition de fin un peu moins certains propos du milieu mais c'est de bonne guerre, je le reconnais bien volontiers je partage d'abord son constat de départ oui, la zone Euro. Et inachevé. Et donc aujourd'hui fragile face au risque de nouvelle crise économique ou de nouvelles crises financières, nous sommes au milieu du gué et il n'y a pas situation plus défavorable qu'être au milieu du gué, soit on est sur une rive, soit on est sur l'autre, mais rester au milieu des courants les plus puissants, ceux d'une zone Euro qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la crise financière de 2008, qui ne s'est pas doté de tous les instruments pour résister face à une nouvelle crise financière qui ne s'est pas dotée d'un budget indispensable pour renforcer la convergence des États-membres, ça ce serait une erreur profonde, il n'y a pas de statu quo possible pour la zone Euro. Soit on avance, soit nous y renonçons mais le statu quo ne peut pas être une solution et d'ailleurs, ni les marchés. Ni nos concurrents ne nous en laisseront le loisir, je partage également l'ambition parfaitement formulée à la fin de votre intervention sur l'Euro qui doit devenir une monnaie de référence. Bien entendu, contre la monnaie chinoise, d'un côté, qui s'affirme de plus en plus et le dollar qui est une monnaie de référence sur les marchés internationaux : l'Euro doit devenir une monnaie de référence internationale. Parce qu'elle nous donnera une puissance politique considérable pour peser sur le cours des affaires du monde et notamment sur les questions commerciales ensuite, comment peut-on y arriver, c'est là que nos avis vont évidemment légèrement diverge. D'abord il faut retrouver sa crédibilité nationale. Et je partage là aussi cette nécessité absolue qu'il y a, pour la France. être crédible auprès de ses partenaires européens, monsieur Raffarin, vous reconnaissez tout de même que nous avons réussi à sortir la France la procédure pour déficit public excessif dans laquelle était englué depuis disons que pour la première fois depuis des années, nous respectons enfin les 3 pourcent de déficit public, nous sommes en dessous et que nous allons tenir cet engagement sur la durée du quinquennat il y a une seule exception, c'était en 2019 parce que nous transformons le CICE en allégement de charges définitif, mais si nous retirons cet événement exceptionnel sur la durée du quinquennat pour la première fois depuis 10 ans, la France sera sous les 3 pourcent le déficit public et elle sera sorti la procédure pour déficit public excessif, j'entends des sénateurs dire c'est faux mais les faits sont têtus, la 2ème chose qui garantit la crédibilité nationale c'est la poursuite des réformes de structures qui sont d'ailleurs saluées par nos partenaires européens, nous avons déjà engagé une réforme de la fiscalité du capital qui allège la fiscalité sur le capital, suppression de l'ISF. Prélèvement forfaitaire unique. Réduction du taux d'impôt, ces sociétés qui va être ramené de 33 véhicules 3 à 25 pourcent d'ici 2022, je rappelle que le président de la République a confirmé avec courage toutes ces orientations fiscales pour la durée du quinquennat nous avons réformé le marché du travail, nous avons réformé le statut de la SNCF nous allons désarmer engager le chantier de l'indemnisation du chômage pour plus de justice et permettre à tous ceux qui cherchent un emploi de le retrouver plus facilement, nous allons engager la réforme de la fonction publique, nous allons engager une réforme sans précédent du régime de retraite pour avoir un système qui soit plus juste, plus équitable, qui soit par point qui soit transparent et et plus les différences que nous regrettons tous entre les agents du service public et les agents du secteur privé, donc vous voyez que les réformes structurelles qui garantissent la crédibilité de la France, elles sont bien au rendez-vous 3ème, chose sur laquelle je voulais insister une fois que nous sommes d'accord sur l'objectif final et nous le sommes. Une fois que nous sommes d'accord sur le constat de risques qui pèsent sur la zone Euro, et nous le sommes, que la France a retrouvé sa crédibilité nationale pourquoi doit-elle plaidé, elle doit plaider en aucun cas pour un fédéralisme budgétaire et relisez attentivement les déclarations et discours du président de la République, jamais le président de la République d'employer le mot de scélérate Prism ce n'est pas notre projet. Notre projet et je vous invite à lire toutes mes déclarations sur le sujet, c'est celui d'États nation qui travaillent plus étroitement ensemble pour rassembler leurs forces et garantir l'efficacité de la zone le 1er objectif c'est l'union bancaire je développe pas trop longtemps, ou l'avez parfaitement fait je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'à force de reculer les décisions sur le Lyon bancaire pour toutes sortes de prétextes qui ne tiennent absolument pas la route, qu'est ce qui se passe, nous ouvrons tout grand le marché unique à nos concurrents américains et les grandes banques américaines qui sont des banques solides à succès sont passés de 43 pourcent du marché unique européen en l'espace de quelques années pour continuer comme ça et faire du marché unique européen, le terrain de jeu des banques américaines, je préférerais que ce soit le terrain de jeu des banques européennes, et pour cela il nous faut l'union bancaire, l'Union des marchés de capitaux est aussi une nécessité absolue et vous avez raison de le rappeler sans Union des marchés de capitaux, il n'y a pas d'investissement sans investissement n'avait pas de champions mondiaux, n'allez pas chercher ailleurs notre incapacité à faire émerger des géants du numérique, quand vous regardez le nombre de Start-Up, quel est aujourd'hui le premier États en Europe en terme de Start-Up de créativité technologique. La France. Et nous pouvons en être siècle. Mais qu'est-ce qui pêche ensuite. C'est la taille de ces entreprises, notre capacité à grandir, nous n'arrivons pas à faire émerger au niveau européen, les champions du numérique, la même taille que Google, Facebook, Amazon ou d'autres, parce que nous n'avons pas un marché unique de capitaux efficace et que les montants de capital-risque investi chaque année en 2018 c'est 100 milliards de dollars aux États-Unis, ces 80 milliards de dollars en Chine et ces 20 milliards en Europe. Pensez petit n'est pas à la hauteur, ni les circonstances ni du projet politique européen que nous portons, enfin le 3ème instrument, c'est le budget. Avec 2 objectifs, là aussi, je ne reviens pas sur les propos de monsieur Rapin la convergence et la stabilisation. Nous avons, et là j'ai un point de divergence avec vous en revanche obtenu un accord historique à Meseberg entre la chancelière Angela Merkel et le président de la République française, nous irons travailler pendant des mois avec mon homologue le vice-chancelier et ministre des Finances, Olaf Scholz diront passer des nuits blanches, pourquoi, parce qu'il y a 2 ans quand j'ai été nommé ministre des Finances, je ne pouvais même pas prononcer le mot, le budget de la zone Euro, quand je me rendais en Allemagne, on parlait d'instruments monétaires d'instruments de convergence, mais surtout pas de budget et, 2 ans après année je Berg le choc, la chancelière allemande et le président de la République française signe un accord dans lequel il était dit et écrit, nous allons mettre en place un budget de la zone Euro pour favoriser la convergence entre les États-membres de la zone Euro et en juin prochain dans un mois nous aurons tous les éléments qui permettront de mettre en place ce budget de la zone Euro en 2 ans, nous avons accompli ce que le président de la République avait promis aux Français et à la nation française, en revanche c'est vrai. Choix stabilisation je regrette que nous n'ayons pas davantage progressé. Mais le problème n'est pas franco-allemand, j'entends beaucoup dire ici qu'il y aurait des difficultés entre la France et l'Allemagne, moi je regardais réalisations depuis 2 ans, et elles sont importantes, la stabilisation, ce n'est pas l'Allemagne qui s'y opposer. Car Aulas Shaul ce lui-même avait proposé un instrument de stabilisation que je trouve tout à fait pertinent, qui était un instrument d'assurance chômage qui disait voilà, si jamais un État membre de la zone Euro qui est en difficulté. Et qui voit son taux de chômage exploser mais qui en même temps respecter ses engagements budgétaires, il a fait tous les efforts de compétitivité nécessaire. Nous paierons à sa place. Les montants d'indemnisation du chômage supplémentaire parce que nous préférons qu'ils continuent à investir, innover à financer ces entreprises plutôt qui retire cet argent-là pour financer l'indemnisation du chômage, c'était un mécanisme vertueux et je continue à penser qu'au-delà de l'indispensable convergence, il faut aussi un instrument de stabilisation, voilà les quelques remarques que je voulais faire, j'aurai d'autres occasions d'intervenir, mais je me féliciter de la qualité des débats que Jean-François Rapin a ouvert avec son intervention et vous remercie également une fois encore sur un sujet qui quête ardue et qui ne suscite pas toujours l'enthousiasme des foules, alors qu'il est décisif pour l'avenir de nos compatriotes d'être venus aussi nombreux. Dans la suite du débat chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassés. La parole est à Monsieur André Gattolin. Oui, merci, merci, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, les prochains mois seront sans doute déterminants pour l'état de santé de l'Union européenne et de la zone Euro en particulier, ainsi le niveau global d'endettement public qui avait légèrement décru en 2018 semblent reprendre sa course en avant notamment en Grèce et en Italie Italie où ce taux atteint plus de 132 pourcent du PIB pour 2018 dans son dernier bulletin économique, la BCE, soulignent les risques pesant sur les perspectives de croissance en zone là encore la situation italienne a de quoi préoccuper puisque le gouvernement vient de ré-abaisser récemment ses prévisions de croissance pour pour 2019 à 0 1 pourcent du PIB, bien loin des espoirs qu'il nourrissait initialement dans un climat déjà des plus atone en raison du Brexit et de la guerre commerciale sino-américaine cette faiblesse de l'Italie menace aujourd'hui la stabilité de la zone Euro, d'autant que l'Allemagne déjà peu enclines à la mansuétude à l'endroit de l'Italie voit sa croissance en Net ralentissement, cette D et s'inquiète de l'important déséquilibre des soldes respectif de leur banque centrale et de celle de l'Italie auprès de la BCE aussi dans ce contexte et dans la perspective de la future réforme de la zone Euro, quelles sont, monsieur le ministre, les mesures préconisées par le gouvernement pour éviter que cette situation inquiétante influe trop négativement sur la résilience tant attendue de la zone Euro je merci. Parole est à monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur, des tôles, hein, je veux d'abord dire que je partage votre préoccupation, enfin, il faut peut-être qu'on ouvre les yeux, un moment donné, on peut toujours dire : tout va très bien madame la marquise, moi ce que je constate, c'est qu'il y a des tensions commerciales fortes qui conduisent à un ralentissement très marqué de la croissance en zone Euro. Avec une situation de récession en Italie. Et un niveau de croissance estimée à 0,5 pourcent pour 2019 pour l'Allemagne qui est censé être la locomotive de la zone Euro. Quand la locomotive est jour régler 5 pourcent de croissance, les wagons derrière ont lieu de s'inquiéter, nous nous faisons je le rappelle, 0,3 point de croissance au 1er trimestres. 2019. Donc, c'est aussi le rôle de la France de faire des propositions pour que nous sortions de ce risque de marasme. Nous ne sommes pas encore. Mais nous pouvons est tombé. Et l'art de la politique, c'est pas de rester scotché à la vitre, c'est d'un d'anticiper ce qui pourrait se produire, j'ai donc proposé à nos partenaires européens, je profite de cette séance pour le rappeler : un contrat de croissance auquel je crois profondément, je ne suis pas le ministre des Finances français qui, comme d'habitude, va dire à nos amis allemands, investissez plus investissaient plus investissaient plus je leur propose. Un contrat dans lequel la France s'engage à poursuivre ces transformations économiques de fond pour gagner en compétitivité, c'est le 1er pilier, le 2ème pilier, c'est que nous accélérions tous ensembles, les décisions nécessaires quant tout est parfaitement rappelés par monsieur Rapin sur l'achèvement de la zone Euro, union bancaire union des marchés de capitaux, budget de la zone Euro en quelques mois, tout ça doit pouvoir être clos fin 2019, ce n'est qu'une question de volonté politique, tous les éléments techniques sont sur la table et nous les connaissons par coeur un peu de volonté politique et un peu de courage le 3ème élément de ce contrat de croissance et de profiter la politique accommodante de la BCE. Nous avons une politique accommodante de la BCE, elle ne durera pas éternellement. Donc utilisons cette fenêtre d'opportunité pour mettre en oeuvre ce contrat de croissance que je propose des réformes pour ceux qui doivent encore en faire, c'est le cas de la France et je le reconnais avec sincérité et honnêteté, plus d'investissement de la part de ceux qui peuvent se le permettre, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres États qui ont une situation budgétaire meilleure. L'achèvement des décisions nécessaires sur la zone Euro, union bancaire nous des marchés de capitaux et budget en profitant de la politique accommodante de la BCE, c'est la proposition que nous faisons nos partenaires européens. Monsieur Gattolin, vous disposez de 51 secondes pour une réplique souhaité voulait non. Quelle élégance, en effet, la parole est à monsieur Pierre Laurent pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, si rien ne change, la zone Euro s'approche d'une nouvelle crise économique et financière, les prévisions de croissance sont mauvaises, vous venez de le répéter et de le redire, en France, elles sont faibles, elles sont plus mauvais en Allemagne encore et en Italie encore davantage la production industrielle de la zone Euro recule, particulièrement en Allemagne, mais de surcroît il y a un grave problème de contenu, prix compétitivité-prix qui domine dégradent le contenu social et écologique de cette croissance on abîmant nos sociétés, les droits sociaux, le pouvoir d'achat, les services publics et en creusant les inégalités de revenus, comme le reconnaît l'OCDE les réponses apportées depuis la crise de 2008 sont en plus inefficace, le niveau de dette publique est aujourd'hui supérieur à celui d'avant-crise et les inégalités dans laquelle ces politiques enfonce l'Europe coûte en plus politiquement de plus en plus cher, comme le montre encore le score alarmant de Vox en Allemagne car la poussée des extrêmes droites en Europe et l'enfant de la faillite libérale européenne face à cette situation, les gouvernements de la zone Euro semble ne pas réagir en cherchant à achever la zone Euro, comme vous venez de le dire, mais sans repenser son contenu, la Banque centrale européenne vient d'ailleurs de confirmer son cap sur la politique déjà menées, il faut changer de trajectoire, Monsieur le Ministre et pour changer de trajectoire, les parlementaires communistes avancent notamment de propositions propres précise pour mobiliser autrement l'argent de la zone Euro, premières propositions changer les critères de la BCE pour cibler ses refinancements vers un autre type de développement économique riche en emplois relocalisent l'activité industrielle utile socialement, écologiquement et, deuxièmement, créer un fonds européen dédié au financement des services publics, le gouvernement est-il prêt à soutenir ces 2 propositions. La parole est à monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le, le sénateur Laurent moi je partage là encore la nécessité d'une réorientation. De la zone Euro et les politiques de la zone Euro pour tenir compte. Ce que nous voyons partout la montée des populismes les inquiétudes de la part de pop qui dise voilà cette zone Euro ne répond pas à nos attentes. La première attendent chacun aime à le dire : c'est la prospérité. Et la zone Euro doit être une garantie de prospérité pour tous les États-membres. Et puis de protection. De protection face à la Chine face aux États-Unis, face aux grands ensembles, ça, ça passe par les décisions dont j'ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus qui permettront de renforcer la zone Euro et de lui permettent d'être plus proche. Le contrat de croissance que je propose, il répond aussi à votre remarque qui est juste, personne ne peut se satisfaire de ce ralentissement de la croissance de la zone Euro en disant : ça ira mieux demain, dans ce cas-là, ne faisons plus de politique ne prenons plus de décisions et laissant les marchés décider à notre place, mais si c'est le marché qui décide entièrement à notre place, c'est toute notre ambition politique qui réduite à néant, moi je crois à la volonté politique, y compris en matière économique et si je propose ce contrat de croissance, c'est que je crois profondément que lorsqu'il y a-t-elle ralentissement qui peut avoir un untel impacts sur la vie quotidienne de nos compatriotes, notre responsabilité c'est de dire il faut faire Entremont. Enfin, sur le contenu, moi je suis prêt à regarder des propositions, y compris des propositions iconoclastes, président de la République a proposé un bouclier social. C'est une proposition qui est iconoclaste dans la zone Euro mais qui pourrait garantir un minimum à toutes les personnes qui travaillent toutes les personnes qui sont, eux, en situation de difficulté dans la zone Euro qui permettraient de montrer que le modèle de développement économique européen, c'est pas celui du dumping social toujours plus vers le bas, c'est celui de la dignité du travail et de la dignité de la rémunération. Sur la Banque centrale européenne, je suis prêt à ce que nous regardions un engagement de toutes les banques centrales. Bon centrale européenne mais aussi les autres banques centrales nationales sur la finance verte, je crois, nécessité d'un financement vers je suis presque nous étudions cette possibilité là. Monsieur Laurent, vous disposez de 30 secondes pour une réplique. Monsieur le ministre, en matière de propositions iconoclastes, vous pouvez compter sur nous, nous n'en manquons pas et j'en ai soumis une sur laquelle vous n'avez pas réagit, c'est la création d'un fonds de développement consacré au développement des services publics, c'est un grand problème dans notre pays, vous le savez, c'est un grand problème dans beaucoup de pays européens et si nous voulons combler les inégalités en Europe il y a de quoi faire pour utiliser la finance, de la Banque centrale européenne pour aider à Tropez à rattraper les retards existants, nous avons donc beaucoup de propositions iconoclastes comme vous les appelez qui sont utiles à être reprise par le gouvernement, merci. La parole est à monsieur Jean Michel Houlgate pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, l'objectif fondamental de l'Union européenne, mais aussi de l'Union économique et monétaire et de garantir le développement économique et la stabilité, ainsi que le progrès et la prospérité pour tous en 2016 Jacques Delors lançait un avertissement clair et qui plus que toujours demeure d'actualité, il disait si l'élaboration des politiques européennes compromet la cohésion et sacrifie des normes sociales : le projet européen n'a aucune chance de recueillir le soutien des citoyens européens, or la création de l'Union économique et monétaire cette accompagné de règles précises relatives aux dépenses publiques dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, il est d'ailleurs à noter que le célèbre économiste Jean Pisani-Ferry dans une communication très récente s'interroge sur la pertinence du maintien de ces règles, notamment celles des 3 pourcent de déficit, alors que les conditions ont sensiblement évolué depuis leur entrée en vigueur en 1997 sous l'effet de la crise, ces règles ont conduit les États à adopter des politiques d'austérité, réduction drastique des dépenses, donc des services publics, diminution des investissements, baisse des dépenses sociales, augmentation de la flexibilité du marché du travail et gel des salaires pour améliorer la compétitivité des entreprises, contribuant ainsi à renforcer le camps des eurosceptiques alors Monsieur M. le Ministre, ma question est double : d'une part, quel rôle entend jouer la France pour réformer le pacte de stabilité, afin de permettre aux États de profiter des taux bas pour financer des uns Davis des investissements productifs, tels que ceux liés à la transition vers une économie bas carbone, d'autre part, en vue de la préparation du prochain sommet pour l'avenir de l'Europe qui se déroulera le 9 mai prochain quelles initiatives la France souhaite-t-elle prendre pour traduire dans des lois européennes au moins au niveau de la zone Euro, hé bien les du socle européen des droits sociaux et notamment les annonces que vous avez mentionné faite par le président de la République pour un salaire minimum européen et pour l'alignement du paiement des cotisations sociales des travailleurs détachés sur des niveaux des pays d'accueil, je vous en remercie. La parole est à monsieur le ministre, pour 2 minutes. On s'écarte à un tout petit peu de la zone Euro mais je veux simplement vous redire notre détermination, celle de tout le gouvernement à mettre en place ce socle des droits sociaux. Notamment, le salaire minimum et pour la rémunération des travailleurs détachés les mêmes exigences que celle que vous avez mentionné, donc ce sera à la ministre des Affaires sociales, le ministre du Travail de porter ses ambitions là le fait déjà avec beaucoup de détermination, mais je veux vous redire que je partage votre analyse, il ne peut pas y avoir d'Europe sans une dimension de solidarité, l'Europe ne peut pas être la compétition sans fin des États européens les uns contre les autres, il faut que nous ayons cette garantie de solidarité, en revanche, les règles, je vais être très clair avec vous, je trouve que. C'est toujours les cancres qui contestent le système de notation. Donc, lorsque vous avez de très bons résultats scolaires pouvaient dire voilà, toutes ces notations c'est absurde, c'est stupide, lorsque vous avez de moins bons résultats scolaires, vous êtes un tout petit peu moins fondé à contester le système de notation donc moi mon exigence comme ministre des Finances et de faire en sorte que la France apporte la preuve à ses partenaires quelle est enfin capable de respecter ses engagements, dont nous sommes touchés dépositaires les 3 pourcent de déficit public en 1er lieu parce qu'on peut contester la pertinence du chiffre pourquoi 3 pourquoi pas de, pourquoi pas 4, bien entendu, mais il faut bien une règle et je pense que la France sera plus crédible pour contester les règles le jour où elle les respectera, elle nous aura respecté pendant plusieurs années d'affilée. La parole est à monsieur Yvon Collin pour 2 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela a déjà été rappelé dans quelques mois l'Euro fêtera les 20 ans de sa création, mais ce sera sans doute Monsieur le Ministre, l'occasion de dresser un bilan de cette monnaie commune à 19 pays de l'Union européenne, nous savons déjà que la progression du PIB par habitant a été de 89 pourcent sur la zone Euro depuis 2000 tandis qu'elle n'a été que de 58 pourcent pour nos amis britanniques à la livre, l'Euro a permis une stabilité des prix et des charges des taux de crédit relativement bas, à la fois pour les ménages et les entreprises, un cas bénéfique à la croissance de la zone Euro, même si on aurait monsieur le ministre, sans doute souhaité mieux actuellement, comme d'autres monnaies, l'Euro est en repli par rapport au dollar en passant sous l'et 1,12 dollars, soit une perte de 2,8 pourcent depuis le mois de janvier dernier, souvent qualifiés de monnaie de confiance : l'Euro doit conforter son assise et ainsi mieux affirmer sa souveraineté en particulier par rapport au dollar mais tout cela suppose évidemment une consolidation des instruments économiques que porte la zone Euro, ainsi que la stimulation de la croissance qui est quelque peu léthargique, malgré un léger rebond finalement observé pour ce trimestre aussi parmi les recommandations du Conseil Ecofine je retiendrai celles qui consiste à demander aux pays de la zone Euro soutenir l'investissement public et privé d'alléger le coût du travail est d'assainir les finances publiques en réponse au mouvement des Gilets jaunes, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces sur le plan économique et fiscale qui à certains égards pourraient envoyer des signaux contradictoires, je pense notamment à la baisse des impôts, bien que perçu par les marchés de change tant qu'elle ne creuse pas notre déficit public, monsieur le Ministre, dans ces conditions, comment la France va-t-elle articuler les exigences qui nous lie à Zone Euro et les dites promesses à nos concitoyens, voilà la question que vous souhaitez vous posez, je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre, pour 2 minutes. Oui, monsieur le sénateur Yvon Collin, je vois beaucoup de contestations aujourd'hui de la zone Euro. Contestation parfois artificielle et je voudrais rappeler que beaucoup de simplicité, quels sont les avantages. Considérable. Que la zone Euro, apporte à nos compatriotes à nos entreprises et à nos concitoyens. D'abord il y a plus d'inflation. On peut le regretter, se dire, faudrait peut-être un tout petit peu plus d'inflation. Mais il n'y a plus cette inflation massive qu'il pouvait y avoir, il y a encore quelques décennies, qui est, je le rappelle, un impôt sur les pour. Car ceux qui perdent le plus, parce qu'il y a une inflation forte, ce sont les ménages les plus modestes ne pas avoir d'inflation, c'est une protection pour les plus fragiles de nos compatriotes. 2ème élément décisif, c'est que vous avez une liberté de circulation des entreprises et du commerce, à l'intérieur d'une zone où il n'y a pas de frais de change, on a la même monnaie et ça facilite le commerce et quand vous avez un commerce intra-européen, qui représente 60 pourcent des échanges commerciaux français, c'est un Avantage considérable pour le développement de nos entreprises, quand elles vont exporter vers Rome vers Berlin ou vers Madrid, elles n'ont pas à payer de frais de change, c'est un Avantage compétitif enfin 3ème Avantage c'est la solidité de cette monnaie qui nous garantit des capacités d'exportation parce que vous avez une monnaie qui est solide, une monnaie qui est forte et que ça facilite les échanges commerciaux extérieurs donc ces 3 avantages décisifs de la zone Euro doivent être mis en avant sans relâche et il y a une faiblesse, mais vous l'avez parfaitement souligné, c'est qu'il n'y a pas assez de convergences au sein de la zone Euro, et que malheureusement certains États objectivement ont davantage bénéficié de cette zone, d'autres en ont moins bénéficié, c'est pour cela que nous avons proposé que le président de la République, le budget de la zone Euro, c'est pour mettre plus de convergence, là où il y a eu au cours des dernières années : trop de divergences.

Oui, monsieur le ministre, quand on a créé la zone Euro, on nous a expliqué que c'était une zone qui ferait contrepoids et qui serait en balance avec le dollar et que la monnaie, l'Euro était en une force pour pour pour les pays adhérents à cette monnaie et pour l'Europe en général et donc pour la France dans dans tout son commerce international, or moi je suis absolument scandalisé de voir la nullité de la zone Euro pour résister aux pressions de Monsieur Trump qui essayent de nous empêcher, par exemple, de commercer avec l'Iran, de faire un certain nombre d'actes de commerce je crois que vraiment s'il y a bien un domaine où l'Euro aura été utile c'est pour résister à la mainmise et à la domination du dollar, or actuellement notre politique étrangère est asservie, je dis bien servi disons : nous sommes à genoux devant le dollar de Monsieur Trump qui nous impose les pays avec lesquels nous pouvons commercer et ceux avec lesquels nous n'avons pas le droit de commercer, moi je lui dis : Monsieur le ministe et scandaleux, c'est de la nullité intégrale des gouvernements qui s'occupe de l'Euro. La parole est à monsieur le Ministre. Heureusement, Monsieur, sénateur, vous avez dit les gouvernements et pas à la France parce que sinon je vous invite à participer à mes entretiens à Washington avec l'administration américaine et vous verrez qu'ils sont musclés, car on nous reproche justement. Quelque chose, qu'en bon gaulliste je soutiens fortement l'indépendance et la souveraineté française, quand le président de la République refuse. De s'engager dans une négociation avec les États-Unis, négociations commerciales, parce que les États-Unis sont sortis des accords de Paris, la réponse est musclée quand nous taxons les géants du numérique parce que nous estimons qu'une question de justice fiscale, la réponse est musclé également, en revanche, je vous rejoins totalement sur la nécessité de résister aux sanctions extraterritoriales américaines, enfin, les États-Unis n'ont pas à être le gendarme de la planète. Et le dollar n'a pas à être l'étalon de l'ensemble du commerce mondial, donc lorsque les États-Unis ont décidé de mettre en place des sanctions extraterritoriales contre l'Iran, alors même que l'Iran est toujours membre de l'accord d'ici et que nous avons signé ensemble, nous avons mis en place avec la Grande-Bretagne avec l'Allemagne un instrument spécifique pour pouvoir continuer à faire du commerce avec l'Iran contre les sanctions extraterritoriales américaines s'il n'y avait pas eu. Cette capacité européenne, je vous aurais dit d'accord, on n'a pas été à la hauteur de l'année des circonstances là je constate que les Européens ont eu le courage de mettre en place cet instrument maintenant je connais suffisamment. Le manque de détermination de certains face aux États-Unis pour savoir que c'est au pied du mur qu'on verra le maçon. Et donc cette au pied de cette institution financière que nous verrons la détermination des États européens à résister aux États-Unis d'Amérique.

à la limite vous me donner raison, mais si on regarde, on constate quand même que nos échanges internationaux avec l'Iran ont baissé de plus que moitié bon alors on ne peut pas être satisfait, non mais franchement, on ne peut pas être satisfait et les dirigeants de l'Euro en général les les pays qui font partie de l'Euro sont totalement, totalement nul et on baisse les bras face aux États-Unis, moi je crois que c'est scandaleux, et si on continue à se laisser faire comme ça, c'est toute notre politique étrangère, tous nos échanges internationaux qui vont être aux ordres des États-Unis, et j'insiste, Monsieur le Ministre, ah, il serait temps de mettre un vrai blocage au sein de l'Euro tant que cette affaire-là il pas réglé. La parole est à monsieur Jean-François longs jours pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, un petit bout d'Europe entre nos mains, c'est ainsi que l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, qualifier l'Euro en 2002, car la zone Euro est au coeur de l'Europe et représente une étape essentielle de l'achèvement du marché intérieur et de l'intégration économique et financière du continent utilisé par près de 340 millions de citoyens travailleurs à travers 19 États-membres faisant de l'Euro, la réalisation la plus concrète de l'intégration européenne, celui-ci souffre toutefois d'un manque d'un cas d'incarnation politique et peinent à avancer en raison de l'obstruction de pays davantage eurosceptique, or le renforcement de l'union économique et monétaire doit être la première priorité, alors que 19 États ont choisi de partager une monnaie commune, de mettre en commun leur souveraineté, il fallait, il faut aller plus loin et accepté une Europe en cercles concentriques dans le dans le coeur sera la zone Euro, avec un marché du travail beaucoup plus intégré une convergence sociale assumée, une meilleure coordination des politiques économiques et budgétaires permettra de consolider ce coeur de l'Europe, toutefois, il est primordial qu'un instrument budgétaire commun puisse s'articuler avec une politique monétaire par définition communautariser les règles de coordination et de convergence des politiques économiques nationales ne son masquer le manque criant d'un outil budgétaire commun qui permettra de facto de limiter les divergences économiques enfin malgré sa technicité l'union bancaire lancée en pleine crise des dettes souveraines européennes doit être achevée, les 2 premiers piliers, à savoir la supervision commune des banques et le mécanisme des résolutions de crises et de gestion des faillites bancaires doivent être accomplis approfondi, tandis que le 3ème pilier, à savoir un système de garantie commune des dépôts reste à construire, monsieur le ministre, pour ces 3 points, quelles sont les priorités françaises en vue de la prochaine réunion de l'Eurogroupe, du 16 mai prochain, quelles sont les priorités du gouvernement pour relancer l'Union européenne en son coeur, tandis que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, mais en en garde contre tout attentisme au sein de la zone Euro, je vous remercie. Oui, il y avait beaucoup de questions dans les interrogations du sénateur sur la supervision bancaire il y a une supervision de la zone Euro, il faut une supervision plus solide des banques européennes. Et ce qui vient de se passer avec une banque danoise attendent ce que Bank montre très clairement qu'il est indispensable de renforcer la supervision bancaire de l'Union européenne et c'est souvent les mêmes qui nous font des leçons de morale en nous disant vous respectez pas ceci vous respectez pas cela va Les règles bancaires européennes et qui soient conformes aux règles anti-blanchiment. Faut pas demander de renforcer les règles pour les uns et pas pour soi-même, donc je souhaite qu'on ait une supervision bancaire européenne plus solide sur l'incarnation, je vous rejoins là-aussi totalement. Une fois que toujours mis en place tous ses instruments et pour moi le calendrier c'est fin 2019, si ce n'est pas le cas, c'est que les États européens, membres de la zone Euro n'auront pas été à la hauteur de leur responsabilité historique, union bancaire une des marchés de capitaux, budget de la zone Euro, budget de convergence et je l'espère, dans un second temps plus tard j'espère arriver à convaincre partenaire qu'un instrument stabilisation est absolument indispensable, mais aujourd'hui le point, chacun le sait, est bloqué, mais il faudra, dans une perspective de long terme, une incarnation, bien sûr. Et l'incarnation, ce sera le ministre des Finances de la zone Euro qui sera un prix s'une perd paraissent et ont rejoint la construction politique que nous vous proposons celle d'États-Nations et pas d'une fédération qui travaillent davantage ensemble, prenez l'exemple de la Banque centrale européenne qui marche remarquablement bien, il y a un prix mouche terre paraissent Mario Draghi, président de la BCE, qui prend ses responsabilités quand c'est nécessaire, mais autour de la table, vous avez tous les présidents de banques centrales, membre de la zone Euro qui donnent leur avis, apportent leur regard sur la situation, c'est à mon avis le bon modèle demain pour la zone Euro. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, la création de l'Euro incarne la réussite la plus palpable de l'Union européenne après avec près de 75 pourcent du PIB de l'Union européenne, la zone Euro finalement constitue la 3ème puissance économique mondiale, elle représente le noyau dur de l'Union européenne, l'Euro a délivré de promesse fondatrice et vous l'avez rappelé la stabilité des prix, avec une inflation moyenne de 1,7 pourcent par an en Europe depuis sa création, c'est-à-dire en fait 3 fois moins qu'au cours des 20 dernières années, fin des années précédentes, les récentes crises ont démontré sa solidité et sa capacité à protéger les économies des États-membres, pourtant, il faut encore progresser, relever les défis qui se présentent à nous, l'achèvement de l'union bancaire la convergence des réformes économiques nationales le renforcement et la souveraineté, l'union économique, la défense du rôle international de l'Euro, les États les plus performants, contribue à la croissance de la zone Euro mais chaque État doit faire preuve de sérieux budgétaire l'idée d'un contrat de croissance et de bon aloi, ces avancées sont d'autant plus nécessaire dans un contexte de concurrence accrue de tensions commerciales et internationales et d'incertitudes liées au Brexit, il est indispensable d'engager des réformes et vous l'avez dit, évitant toute divergence entre les politiques menées par les États-membres et surtout pour peser face à de grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine, la zone Euro renforce nos positions sur les marchés mondiaux, alors que la dette européenne baisse globalement et que la croissance semble se maintenir dans la zone Euro, l'Italie, qui mène une politique expansionniste voit sa dette augmenter sans reprise de sa croissance, les décisions budgétaires de que ce pays prend peuvent avoir des répercussions très négatives sur ses voisins qui font des efforts budgétaires demandés fort pas toujours populaires d'ailleurs auprès de nos concitoyens, monsieur le Ministre, alors même que la commission doit refaire un point de situation budgétaire en juin : comment éviter que des États comme l'Italie mène des politiques économiques allant à l'encontre des autres États-membres : que compte faire la France pourra faire avancer concrètement ces réformes indispensables de la zone Euro pour convaincre nos partenaires, et notamment pour développer le soft power de la zone Euro, merci de votre réponse. La parole est à monsieur le ministre. Je ne suis pas satisfait du niveau de croissance dans la zone Euro. Et ça a été dit par d'autres sénateurs, je pense que si on se satisfait de ce niveau de croissance. Il faudra pas s'étonner de la montée des populismes partout en Europe, qui auront mais écoutez votre Euro c'est bien sympathique, mais si c'est pour avoir 0 0 2 0 5 point de croissance, être à la traîne, là où d'autres grandes nations comme les États-Unis ont de meilleurs résultats que nous, c'est que votre Euro ne marche pas. Donc il est temps que nous prenions nos responsabilités, c'est le contrat de croissance que j'ai proposé des réformes, d'un côté pour ceux qui en ont besoin, dont la France, plus d'investissements, pour ceux qui en ont la capacité budgétaire dont l'Allemagne. L'Allemagne dépense plus qu'elle ne le faisait auparavant, mais elle peut dépenser encore davantage pour financer des investissements qui bénéficieront à l'ensemble de la zone Euro, c'est le contrat que je propose, vous parlez ensuite de la situation italienne. Moi ce que je dis à chaque fois, nos partenaires italiens, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons abandonné notre souveraineté monétaire, j'entends certains dire la campagne européenne, il n'y a pas de souveraineté européenne, parce que là, ce qu'ils ont abandonné l'Euro car l'Euro, c'est un instrument de souveraineté européenne, s'il n'y a pas Chevrette européenne il n'y a pas d'euros donc tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de souveraineté européenne ont des facto renoncer à l'Euro et à la zone Euro. Mais à partir du moment où nous avons partagé cette souveraineté que nous avons une monnaie commune, il faut que chacun respecte les règles, c'est trop facile d'aller voir chacun sa propre population nous en ont fait ce qu'on veut, on est complètement libre, on est complètement indépendant et on se moque de ce que dira l'Allemagne, la France, l'Espagne ou autre, alors même que c'est notre cohésion qui fait notre force, que c'est des règles que nous respectons tous qui font la force de notre zone commune, personne ne peut s'abstraire de règles qui a librement et souverainement choisi parce qu'elle le protège et elle protège la zone Euro dans son ensemble. La parole est à monsieur René Danizy pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur les ministres, mes chers collègues, le dollar est la monnaie la plus utilisée pour les échanges internationaux de biens et de services, mais aussi pour les réserves de change dans le monde cette supériorité du dollar permet aux États-Unis de pratiquer une politique extérieure agressive et cela au point de faire condamner à de lourdes amendes les entreprises non américaines, qui ont utilisé le dollar pour des transactions avec des pays que les États-Unis boycottent avec son internationalisation le Yukon chinois est intégrée aux réserves de change de plusieurs États, dont la Russie, certes, le FMI estime à moins de 2 pourcent la part du Yuan chinois dans le total des réserves de change des 149 pays suivis par cet organisme, mais la part du One ou chinois a quasiment doublé dans ce pays entre 2017, 2018, la valeur du Yuan chinois, c'est la volonté de la Chine d'en faire progressivement une bonne le concurrent du dollar devienne le sujet central dans les vif débat entre la Chine et les États-Unis, il n'en est pas de même pour l'Euro, dont la position, pourtant, est bien plus forte maintenant inquiète guère les États-Unis et pour cause, en effet, l'Euro remplit gentiment un rôle d'intermédiaire des échanges internationaux à hauteur de 36 pourcent contre 46 pourcent pour le dollar, mais d'une part, plus de 80 pourcent des importations d'hydrocarbures des pays de l'Union européenne sont payées en dollars, d'autre part, seulement 22 pourcent des réserves mondiales de change sont détenus en euros contre 60 pourcent en dollars dans ce rapport annuel de 2018, la Banque centrale européenne juge que la place de l'Euro dans le monde n'a jamais été aussi réduite selon la BCE, l'Euro a perdu 3, dans les réserves mondiales de change entre 2008 et 2017, certes la fiabilité économique de l'Euro et rassurante mais sa crédibilité géopolitique n'est pas à la hauteur de la puissance économique que l'Union européenne pourrait être si elle en avait la volonté politique, l'alignement des principaux pays de l'Union européenne sur la politique étrangère agressive des États-Unis comme ça le cas vis-à-vis de la Russie, on leur incapacité à s'y soustraire efficacement comme ça le cas vis-à-vis de l'Iran permettra pas à l'Euro de trouver cette crédibilité GO pour. Chers collègues Je termine, madame la présidente, la France qui affiche ses ambitions pour une Europe qui protège à-t-elle, consciente qu'un Euro réellement indépendant du dollar serait le meilleur bouclier de l'Europe et citait le cas quelles sont les propositions concrètes que la France prête à faire à ses partenaires pour forger ce bouclier. La parole est à monsieur le ministre. Monsieur le sénateur. Il n'y a pas de puissance. Et le projet politique sans monnaie. Et l'Euro doit être l'instrument de la puissance politique européenne. Sinon, là encore. L'Euro n'a pas d'avenir et toutes les discussions que nous avons aujourd'hui montre bien le chemin qu'il y a à suivre, il faut une incarnation, le ministre des Finances de la zone Euro. Il faut des instruments complémentaires, union bancaire union des marchés de capitaux, budget de la zone Euro. Et il faut une ambition. Elle y ont pas peur d'employer ce mot, il faut que l'Europe politique est une ambition et son ambition doit être que l'Euro soit demain une monnaie de réserve équivalente au dollar. Et c'est possible. Nous avons le marché de consommateurs, le plus riche de la planète, on a un peu tendance à l'oublier, mais je rappelle que les 500 millions de consommateurs européens font le marché le plus attractif et le plus riche de la planète. Nous avons une monnaie qui est solide, stable, l'Euro. Il y a un certain nombre de décisions maintenant à prendre, ça peut être des décisions très concrètes : premières propositions que les facturations se fasse désormais en euros et pas en dollars pour les entreprises européennes qui exportent. C'est un moyen de faire de l'Euro, une monnaie de référence sur la scène internationale. 2ème proposition on en a rappelé les contours tout à l'heure avec Monsieur c'est d'avoir un instrument financier, avec des réserves en euros qui nous permettent de financer les échanges commerciaux, y compris avec des États placés sous sanctions extraterritoriales américaines. L'Euro, outil d'autonomie outil d'indépendance politique, mais pour ça il faut cette institution financière totalement indépendante, enfin 3ème volet, être capable de développer le commerce en euros en ayant conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers la planète. Quand vous regardez le montant total des investissements de l'Exim Bank chinoise en Afrique. Ils sont supérieurs aux investissements de la Banque mondiale. Depuis 2 ans. c'est ça, dit le renversement de puissance qui est en train de s'observer aujourd'hui bien face à cela, notre intérêt et faire de l'Euro, une monnaie de référence internationale, la Commission européenne a fait des propositions en ce sens-là, nous les soutenons et j'y ajoute celle que je viens de faire la facturation en Euro, l'outil financier indépendant et le développement des échanges commerciaux, sur la base de notre monnaie commune. La parole est à monsieur Yannick Botrel pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, lors du Conseil européen de décembre dernier, les 27 États membres se sont accordés sur le principe d'un budget de la zone Euro toutefois éloigné du projet porté ces dernières années, tout comme d'ailleurs de l'ambition initiale défendue par le président de la République en début de son mandat, la France, nous semble-t-il, a reculé sur plusieurs points essentiels à nos yeux, et ce dès la déclaration commune avec l'Allemagne en décembre 2018, loin des déclarations du mois du mois de juin précédents, à l'occasion du sommet de Meseberg le 1er point concerne l'investissement, l'intérêt d'un budget à la disposition des États-membres de la zone Euro, aurait été de favoriser leurs convergences afin de réduire les risques de dysfonctionnement économique nous en sommes éloignés, le 2ème point porte sur l'abandon de la fonction de stabilisation économique que nous n'avons cessé de demander et qui donnerait tout son sens à la dimension budgétaire afin d'en faire un véritable outil de protection en cas de nouvelle crise financière, or l'idée d'un fonds permettant de résister aux chocs asymétriques et de disposer notamment d'un système d'assurance chômage européen qu'un État membre de la zone Euro pourrait activer a littéralement disparu de la position commune franco-allemande, le 3ème aspect concerne le financement de ce budget, celui-ci est réduit, le fait à une simple ligne budgétaire du budget général de l'Union. Ce budget court le risque de se résumer à un simple fonds européen très éloigné de ce qu'on aurait pu attendre et c'est ce qui serait nécessaire, vous l'aurez compris monsieur le ministre, de sommes préoccupés du tour que prennent aujourd'hui les négociations, il ne suffit pas en effet d'annoncer un projet mais il faut faire en sorte qu'il puisse, une fois adoptée, porter des ambitions, monsieur le ministre, ma question est la suivante, elle est double : reste-t-il encore une marge de manoeuvre afin de retrouver un budget de la zone Euro qui intégrerait plus étroitement les pays partageant la monnaie unique. à ce stade, la France peut-elle encore défendre le principe d'une fonction de stabilisation pour ce budget. Oui, Monsieur le Sénateur Botrel. Moi, je ne suis pas très savant. Donc j'écoute. Ceux qui savent plus que moi. Le FMI, l'OCDE. Le président de la Banque centrale européenne. Tous disent : il faut que le budget de la zone Euro est une fonction de stabilisation. Moi, je l'ai dit, je l'ai répété il y a aujourd'hui une opposition farouche un certain nombres d'États à toute fonction de stabilisation de la zone Euro. Je pense en particulier aux Pays-Bas qui se sont fortement opposés à toute idée d'une fonction de stabilisation pour le budget de la zone Euro. L'Union européenne, elle se bâtit pas à pas, Dieu sait que j'aimerais parfois qu'elle chausse les bottes de 7 lieues mais il se trouve qu'on est obligé pour avancer et de faire de temps en temps, des compromis. Les compromis ne doivent jamais être des renoncements. Aujourd'hui, nous avons le principe d'un budget de la zone Euro, c'est déjà un progrès considérable par rapport à il y a 2. Nous avons acté la fonction de convergence, c'est-à-dire des investissements supplémentaires pour que les économies convergent alors qu'aujourd'hui elles sont en train de diverger et ça menace l'avenir de la zone Euro, je ne renonce pas à la fonction de stabilisation de la zone Euro, je veux le dire avec beaucoup de simplicité parce que j'y crois et parce que je considère que lorsqu'on aura une prochaine crise économique, on sera bien content d'avoir des instruments stabilisation pour éviter que lié un état 2 états 3 États qui coule et qui soit entraînés vers le fond, faute de solidarité et ce mot solidarité entre les États membres de la zone Euro, on ne doit pas en avoir peur, la compétition oui mais à condition qu'il est aussi de la solidarité. Enfin, sur le financement, il faut qu'il y ait des ressources propres, je pense, par exemple la Taxe transactions financières, on peut imaginer aussi d'affecter une partie des ressources issues de la taxation des géants du numérique, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. La gouvernance de la zone Euro, elle doit se faire à 19. 19. Il faut qu'il y ait un instrument de gouvernance à 19 de la zone Euro. Et si les États non membres de la zone Euro veulent participer à la décision, hé bien ma recommandation, c'est qu'ils adhère à la zone Euro. La parole est à Madame Sylvie Vermeil et pour 2 minutes je vous en prie. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi a déclaré il y a quelques semaines que les risques liés aux perspectives de croissance de la zone Euro sont toujours orientés à la baisse en raison de la persistance d'incertitudes liées aux facteurs géopolitiques à la menace du protectionnisme et aux vulnérabilité des marchés émergents, cette baisse de la croissance qui affecte au-delà de la zone Euro, l'ensemble des économies industrialisées, a conduit la BCE à poursuivre sa politique monétaire dites à Cottbus accommodante, avec notamment des taux d'intérêt très bas. Cette politique a 2 objectifs principaux : d'une part, la relance de l'activité économique, force est de constater que les résultats ne sont pas ici, à la hauteur des attentes, d'autre part, éviter une augmentation brusque des déficits publics qui entraînerait une hausse de la dette publique concernant ce 2ème aspect, il convient de rappeler que la crise des dettes souveraines européennes entre 2010 et 2012 a failli tourner à la faillite de l'État grec et à l'éclatement de la zone Euro, c'est donc une priorité que d'éviter que ce scénario ne se reproduise et les pays membres de la zone Euro ont d'ores et déjà mis en place des mécanismes de stabilité ces réformes bienvenue nous semble cependant par trop partielle voire incomplètes au regard des enjeux et des risques que la situation économique actuelle fait peser sur la stabilité de la zone Euro et de l'Union européenne dans son ensemble, nous pouvons, par ailleurs nous demander si c'est bien le rôle de la Banque centrale que de veiller à ce que les États ne se retrouvent pas en faillite, qui plus est, sa politique monétaire accommodante ne pourra se poursuivre éternellement, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, nous devons sortir de cette situation inconfortable où en sont donc les propositions de la France, monsieur le Ministre, en faveur d'une intégration politique plus poussée des pays membres de la zone Euro, je vous remercie. La parole est à monsieur le Ministre. Madame la sénatrice, les divergences actuelles. De situation économique entre les États membres de la zone Euro ne sont pas tenable. Je le redis avec beaucoup de gravité. Vous ne pouvez pas avoir une union monétaire et des divergences croissantes entre les États membres de cette zone monétaire, ce n'est pas tenable. La croissance aujourd'hui et la faiblesse de la croissance de la zone Euro n'est pas tenable non plus sur le long terme. Donc, je partage l'appréciation du président de la Banque centrale européenne, il est urgent de réagir, alors il y a des responsabilités nationales, c'est ce que j'ai dit ce que je martèle c'est la poursuite des transformations pour gagner en compétitivité et réussir davantage économiquement. Mais il faut également que l'Union européenne, la zone Euro sera capable, je le disais tout à l'heure à monsieur Botrel, de faire preuve de plus de solidarité. Vous ne pouvez pas d'un côté exiger des réformes structurelles, exiger le rétablissement des finances publiques et de l'eau, vous direz voudrait contrepartie rien. ça, c'est pas possible. La contrepartie, c'est de la solidarité, la garantie des dépôts bancaires et un instrument budgétaire qui permettent aussi de faire de la stabilisation, enfin, puisque vous avez beaucoup cité la BCE, je voudrais en profiter pour rendre hommage au président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Qui, en pleine crise des dettes souveraines, à un moment où les spread entre l'Italie, la Grèce et l'Allemagne pouvaient atteindre 300 400 600 points de base. Et où la zone Euro était menacée d'éclater. A eu le courage de venir devant la presse, devant l'opinion publique européenne et dire : nous prendrons toutes les décisions nécessaires. Pour rétablir la situation, souvenez-vous de sa fameuse phrase : Whatever It Tex. Eh bien moi, j'aime l'Europe quand il y a à la tête d'une de ses institutions, un homme qui a le courage et la lucidité pour prendre les décisions qui s'imposent et je veux dire à tous mes homologues européens que nous sommes aujourd'hui dans une situation analogue. analogue. C'est à Madame Christine L'avare de pour 2 minutes. Monsieur le ministre, le 15 décembre 2018 le sommet de la zone Euro, a demandé à l'Eurogroupe d'élaborer d'ici la fin du mois de juin une proposition détaillée pour un instrument budgétaire spécifique à la zone Euro selon le mandat donné au ministre des Finances, par les chefs d'État et de gouvernement cet instrument se concentrera uniquement sur le soutien à la convergence et à la compétitivité, la Commission avait proposé en mai dernier un outil de stabilisation reposant sur un système de pré-propositions déjà en retrait par rapport à celle formulée par le président de la République toutefois aucun consensus n'a pu émerger pour soutenir cette idée qui a donc été exclu du monde a adopté en décembre, malgré cette première clarification les divergences d'appréciation semble toujours très forte entre les États-membres et de nombreuses questions demeurent en suspens sur les principaux aspects de cette capacité budgétaire notamment sur la nature et à la finalité de ces dépenses sur sa base juridique sa gouvernance son lien avec le semestre européen et surtout l'origine de ces recettes et son temps, la France et l'Allemagne ont notamment proposé qu'il soit alimenté par des ressources propres ici de nouvelles taxes par des contributions nationales et par des financements européens, à ce titre, la Commission avait proposé dans son projet de cadre financier pluriannuel de mieux 21 2027 un programme doté de 25 milliards de retour sur 7 ans pour financer un outil d'aide à la mise en place de réformes structurelles, ainsi qu'un mécanisme de convergence, monsieur le Ministre, même si les négociations sur ce point sont toujours en cours, pouvez-vous nous indiquer sur quelle base travaille la Commission et les États membres en ce qui concerne le volume financier de l'instrument budgétaire pour la zone Euro par ailleurs les difficultés rencontrées par la taxe sur les services numériques ou la taxe sur les transactions financières sont indiqué que celui-ci ne sera pas financée dans un horizon prévisible par de nouvelles ressources propres, mais essentiellement par des contributions budgétaires nationales, pouvez-vous dès lors nous préciser le montant attendu de la participation française et son impact sur le aux finances publiques, je vous remercie. Nous avons accepté, madame la sénatrice pour que il y ait un accord sur le budget de la zone Euro, un accord d'abord avec l'Allemagne, puis un accord à 19. Nous avons accepté des compromis. Je vous accepter d'abord qu'il y a un lien entre le budget, la zone Euro et les perspectives financières pour l'Union européenne pour les années à venir alors qu'on aurait pu très bien imaginer une indépendance totale, nous avons accepté, qui un lien. Nous avons accepté également, ça a été souligné par beaucoup d'entre vous que ce soit un budget de convergence et pas un budget de stabilisation qui privilégie l'investissement mais qui ne permettent pas de réagir en cas de crise économique. Nous n'iront pas plus loin sur les concessions. Nous n'irons pas plus loin. Nous devons avoir désormais en juin prochain. Un certain nombre de décisions et ces décisions doivent être prises. La gouvernance, je le redis, doit se faire à 19. Et la France n'acceptera pas que la gouvernance de la zone Euro se fasse par des États qui ne sont pas membres de la zone Euro, je ne vois pas pourquoi ceux qui ont abandonné leur souveraineté monétaire, pour avoir une monnaie commune se verraient dicter l'avenir de cette zone Euro par ceux qui n'ont pas renoncé à leur souveraineté monétaire. Et là-dessus, que les choses soient bien claires, nous voulons une gouvernance à 19. La 2ème chose c'est qu'il faut des ressources propres. La Taxe transactions financières, nous ne sommes pas loin d'un accord, ça peut être une ressource propre pour la zone au. Enfin, le 3ème, point sur lequel je veux insister, en réponse à votre question, c'est que c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée, je continue à considérer qu'il faudra à un moment ou un autre et je préfère qu'on le fasse en dehors de la crise plutôt que de faire comme à chaque fois on dit non non non non, puis il y a une crise, et on dit : oui, il serait plus raisonnable de dire oui tout de suite et de comprendre qu'il faut une fonction de stabilisation au budget de la zone au. Madame la présidente, ce Ministre, mes chers collègues, l'Europe ne produit plus d'Européens, ce constat est terrible, certes, mais bien réels dans cette aire géopolitique, elle nous européenne et qui, pour la première fois dans d'ailleurs beaucoup d'autres ensembles européens pour ce qui s'est bâti, pardon, sur la base du choix des États et non pas sous le joug de telle ou telle armée mais d'ailleurs, et je l'évoque ce que de Gabon collecte à l'heure, une des plus grandes réussites de l'Union européenne, c'est effectivement de sa maîtresse, sait l'Euro, mais l'Euro, qui était pensé au départ comme un outil au service de l'Union, un instrument de protection, développement des économies. Tant en interne qu'en externe, aujourd'hui il y a aussi un constat pour beaucoup d'échecs quant à son rôle dans ce qu'est l'Union européenne, car au-delà de cette monnaie que nous partageons, qu'il a ce qu'est ce qui la composent une gouvernance démocratique, pas vraiment une convergence fiscale pas davantage une convergence sociale, encore moins, en effet, dans cet ensemble plusieurs États censés coopérer se livrent en fait une véritable concurrence parfois fiscale et la France, récemment encore apporter sa Pierre à signifie fils avec la flaque taxe et l'exit tax et 12 euros c'était qu'effectivement le budget de la zone Euro soit orienté, encore une fois bien sûr vers le développement économique mais également vers une politique sociale digne de ce nom, digne d'une puissance économique qu'est l'Europe. Je pense même en au mécanisme européen d'assurance chômage à la sociale européenne en passant par le roi de la formation, mais aussi un salaire minimum européen et je crois que dans le débat européen des européennes, certains ont tenté, mais en se prenant les pieds dans le tapis et aussi d'intégrer des indicateurs sociaux dans le processus semestre européen. J'en veux dire que l'échec de la directive des travailleurs détachés en tout cas votre vision est un contre-exemple aussi Monsieur le Ministre, comment comptez-vous dorénavant un peu peser dans les discussions et surtout au niveau européen, pas d'actions concrètes pour faire en sorte que ce budget, la zone Euro soit réellement un service un outil au service de la croissance, mes jambes dire surtout de la convergence sociale dans l'Union européenne, qui est quand même aujourd'hui, je crois, beaucoup d'extrémistes et faire en sorte qu'il y est effectivement une véritable direction une véritable gouvernance politique à 19 de la zone Euro. La parole est à monsieur lui 10. Monsieur le sénateur Thema, l'une des conditions de la convergence sociale, c'est la convergence fiscale. Parce que la convergence fiscale et vite. Ce qui à mon avis peut profondément déstabilisé la zone Euro, le dumping fiscal. Le dumping fiscal est une plaie dont il ne sortira rien de bon. Ni croissance ni emploi ni capacité de résistance face aux États-Unis où face à la Chine. La convergence fiscale est au coeur de l'accord de Meseberg je redis que cet accord de Meseberg entre la chancelière, président de la République est un accord historique, vous avez la convergence fiscale sur l'impôt sur les sociétés dans l'accord de Meseberg nous le construisons nous avançons notamment en rapprochant les droit des faillites français et droit des faillites allemand donc tout cela avance et je souhaite que les autres États-membres de la zone Euro nous suivent dans cette convergence de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, si nous voulons vraiment une convergence, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il faut qu'on passe de l'unanimité à la majorité qualifiée en matière fiscale. C'est la seule façon d'avancer, regardez ce qui s'est passé sur la taxation des géants du numérique, nous étions seuls au départ puis 5 ensuite 23 autres Européens totalement mobilisé là-dessus, la Commission européenne, qui propose un texte, un texte solide convaincant pas parfait, mais il était solide et l'été convaincant et puis 4 états qui se mettent en posture d'opposition systématique à la taxation du numérique, malheureusement, il savait que, quoi qu'il arrive, il fallait les limiter, donc si on n'arrivait pas à les convaincre, il bloquerait ils ont bloqué et c'est l'Union européenne tout entière qui est fragilisé, donc si nous voulons vraiment la convergence ayons du courage et passion l'unanimité à la majorité qualifiée en matière fiscale. la parole. ça monsieur Serge pas Bari pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, monsieur le ministre, vous venez de proposer à nos partenaires européens un nouveau contrat de croissance pour la zone Euro, ce nouveau contrat est justifié par le constat d'un ralentissement de la croissance mondiale, il repose sur 4 piliers, dont notamment l'accélération de la transformation de la zone Euro, avec un budget disponible pour juin prochain et l'union bancaire Alizé d'ici fin 2019, la zone Euro a déjà connu plusieurs réformes qui lui ont permis de surmonter les crises je pense ici aux prémices de cette union bancaire au renforcement de la gouvernance économique ou encore à la création d'un mécanisme de sauvetage permanent qui peut mobiliser jusqu'à 700 milliards d'euros, la zone Euro s'invente grâce aux crises ces réformes desquels les peuples ont été tenus à l'écart, ont cependant eu un prix démocratique, le Brexit, l'émergence d'eurosceptiques, voire d'europhobes en témoigne aussi, ce contrat est un 1er pas mais il ne remplacera pas la réforme d'envergure qui est attendu et qui conditionnera l'avenir de la zone Euro, s'il est indispensable de renforcer le pilotage exécutif de la zone, en se posant la question du contrôle démocratique de la place des partenaires et des parlements nationaux, l'enjeu démocratique n'est pas qu'institutionnel, la zone Euro, a été mis en place, mais les politiques budgétaires, économiques, fiscales et sociales sont restées indépendantes, c'est l'existence d'une Union européenne à 27 et d'une union monétaire, à 19 sans aucune convergence des législations qui pose aujourd'hui problème, l'Europe est perçu par les peuples de la zone Euro, comme celle qui entravent qui admet le déséquilibre si un État est exigeant, il s'impose des normes de qualité, il sera confronté au sein même de la zone Euro à la concurrence, de produits émanant d'autres États fabriquer à moindre coût et de moindre qualité, il est urgent de renforcer la confiance des peuples dans l'Europe, redonner confiance, c'est d'abord créer une Europe et une union monétaire intelligible, c'est aussi, à mon sens, créer les conditions de marché structuré, le choix est simple : est ce que lorsque on se contente d'administrer, de réfléchir à une gouvernance ou est-ce que l'on crée les conditions de marché structuré au sein de l'Union monétaire en renforçant l'équilibre, l'équité, la concurrence loyale entre États de l'Union, par une convergence économique, fiscale et sociale, je vous remercie. La parole est à monsieur le Ministre. Vous savez, Monsieur le Sénateur, Barry, qui aiment bien. Châtie bien. Et si je suis parfois sévères, avec une européenne, c'est parce que j'aime profondément européenne et que je crois profondément au destin français en Europe et au destin européen. Et quand je regarde ce qui est nécessaire, devant nous, il voulait parfaitement dit. L'Europe ne se réforme qu'en situation de crise. Mais on pouvait se permettent cela. Jusqu'au Brexit. Jusqu'à l'émergence des partis extrémistes partout en Europe, maintenant que nous voyons le danger tous ceux qui croient dans le Démocratie libérale. Tous ceux qui croient dans la nécessité de garder un système démocratique comme celui que nous avons devrait se dire, il y a urgence à décider, urgence à faire progresser la zone Euro, urgence à mettre en place les instruments dont nous avons parlé et je le dis très simplement je pense qu'aujourd'hui, l'organisation institutionnelle de la zone Euro n'est pas satisfaisante que tout est fait pour qu'on ne puisse pas décidé. C'est très concret, la politique, vous êtes tous ici des élus, tous les responsables politiques chevronnés, vous savez que les formats sont décisifs, vous savez que les corps sont décisifs, quand on vous arrivez comme ministre des Finances. De la zone Euro, l'un des pays les plus importants de la zone Euro, que vous voyez autour de la table, qu'il y a évidemment les 19, ministre des Finances de la zone Euro mais il y a aussi la Commission européenne et puis il y a le vice-président qui a Banque Centrale européenne et puis il y a le vice-président la Banque centrale européenne et puis le représentant du mécanisme européen de stabilité et puis il a le représentant du service légal de la commission et puis il y a aussi des États non membres de la zone Euro, parce qu'il faut quand même qu'il participe à la discussion, on pourra aussi invité tous les États étrangers à venir assister à nos réunions pour savoir ce qui s'y passe, tout est fait, est organisé pour qu'on ne décide pas ça suffit. Je le dis avec beaucoup de gravité, il faut passer à autre chose. Il y a d'autres modèles de gouvernance qui serait 1000 fois plus efficace qu'il faut être capable d'anticiper et d'imaginer le jour où j'aurais autour de la table, les 19 ministres des Finances et imprime auch in their paraissent ministres des Finances de la zone Euro qui aura la petite voix décisive supplémentaire pour dire voilà où nous allons, il y en a qui sont pas d'accord, il raconte des réticences, c'est pas grave, on avance dans cette direction, parce que c'est comme ça que nous serons tous ensemble plus fort là nous aurons franchi le cap décisif que nous n'avons toujours pas franchi aujourd'hui et je préfère monsieur Bovary le faire en situation le calme qu'en période de crise. La parole est à madame Nicole Duranton pour 2 minutes chers collègues. Présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le temps a passé, depuis la signature de la déclaration de Meseberg en juin 2018 et la signature du traité d'Aix- la-Chapelle, en janvier dernier, le 1er texte nous engager à réaliser des progrès décisifs vers une union des marchés de capitaux et à créer un budget de la zone Euro, dont le but serait de promouvoir la compétitivité, la convergence et la stabilisation de la dite zone le second afficher plusieurs projets prioritaires dont le suivi serait assuré par le conseil des ministres franco-allemand, avec une volonté de coopération au sein de l'Union européenne dans le domaine des services et des marchés financiers, la chancelière en Nigel à Merkel puis les pays nordiques groupés derrière le chef du gouvernement néerlandais ont largement minoré l'ambition et les objectifs de ce projet de budget, ils refusent que ce budget joue un rôle de stabilisateur en cas de choc économique et à juste titre, compte tenu de la situation économique et financière de la France, on ne peut pas convaincre nos partenaires européens, sans leur apporter la preuve que nous pouvons restaurer nos comptes publics, au risque de donner l'image d'un projet déresponsabilisant les États qui, quelle que soit leur gestion seront de toute façon, par ce fonds, ce dernier n'aura que peu de réserve en raison de la mauvaise santé économique de ses contributeurs, plus récemment, la tribune intitulée pour une renaissance européenne que le président de la République a publié en mars dernier, n'évoque pas une seule fois la zone Euro, cela est très significatif d'un renoncement à réformer en profondeur l'union économique et monétaire au profit d'un repositionnement sur les questions de liberté et de sécurité, l'accord est fragile entre la France et l'Allemagne, car il ne semble pas vouloir aller pour l'instant, au-delà des bonnes intentions, monsieur le ministre, vous avez répondu en partie à mes questions en ce qui concerne de ce que la France compte faire pour maintenir ses finances publiques pour rassurer nos partenaires européens, mais la trajectoire d'ici 2000 22 et loin de celle de ses partenaires de la zone Euro, pouvez-vous me préciser qu'en matière de convergence, il y aura une concrétisation de ses ambitions et quelles sont les pistes et les discussions qui porteront en juin, nos concitoyens et nos partenaires européens ont besoin d'être rassurés sur l'engagement de la France, je vous remercie. La parole est à monsieur le Ministre. La France a pris et Madame Duranton. 2 engagements vis-à-vis de ses partenaires européens et surtout 2 engagements vis-à-vis de nos compatriotes. Le 1er engagement c'est le rétablissement des finances publiques, le 2ème, c'est la poursuite de la transformation économique de notre pays, nous tiendrons ces 2 engagements. Ces transformations économiques, j'ai eu l'occasion de le dire, l'indemnisation du chômage, les retraites, la fonction publique. Feront l'objet de réformes structurelles dès 2019, le président de la République et le 1er ministre l'ont indiqué. S'agissant des finances publiques, nous resterons sous les 3 pourcent de déficit public et nous devons continuer non seulement à stabiliser mais abaissé la dette publique qui est, je le reconnais bien volontiers le point noir de la situation des finances publiques françaises, ça veut dire tout simplement que si nous ne voulons pas aggraver la charge de la dette, à chaque fois qu'il y a une nouvelle dépense, il faut trouver des recettes équivalentes. Sur les 5 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu, il faut qu'il y ait un financement et le financement, le président la République a été très clair sur ce sujet, il doit reposer sur. Les organismes publics, dont un certain nombre doivent être transformée en profondeur. Quelques niches fiscales portant sur les entreprises, mais je le redis, cette une partie du financement seulement moi pas financer l'intégralité des 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu par la remise en cause. De niche fiscale sur les entreprises, ce serait totalement incohérent et le 3ème volet qu'a signalé le président de la République, c'est sur la durée du travail, voilà les modalités de financement sur lesquels, à la demande du 1er ministre nous travaillons dès aujourd'hui avec Gérald Darmanin prenez l'exemple des organismes publics, nous allons avec Gérald Darmanin dès cette semaine en vue d'une prochaine réunion autour du 1er ministre lundi faire la revue de l'ensemble de ces organismes publics pour lesquels sont efficaces les le sont moins et où nous pouvons faire des économies, nous avons ici au Sénat, une longue discussion sur les chambres de commerce et d'industrie, moi je voulais citer en exemple car les chambres de commerce et d'industrie, bénéficier d'une taxe affectée de plus d'un milliard d'euros, elles ont accepté une transformation en profondeur la réforme de leur statut, un financement par prestation et non plus uniquement par taxe affectée ça se solde par un demi-milliard d'euros d'économies donc les économies sur la dépense publique, c'est une affaire de volonté et avec Gérald Darmanin nous avons cette volonté à la demande de prêt Ministre du président de la République de regarder soigneusement attentivement en profondeur tous les organismes publics pour voir où nous pouvons faire des économies. La parole est à monsieur Yves Boulou pour 2 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, chaque collègue c'est sur la question de la stabilité financière que je souhaiterais vous interroger Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, vous déclariez dans une interview accordée à Reuters qu'il vous nous faut mettre en place l'union bancaire, je cite, dans les prochains mois et pas dans les prochaines années, difficile de ne pas me rejoint dans cet objectif, mais aujourd'hui, le contexte politique actuel est telle que cette affirmation présente une valeur relative dans le débat public d'autant plus que vous parlez de mesures techniques, sans préciser les mesures visées, or la plupart sont des facto des mesures politiques aujourd'hui, avant même l'achèvement d'union bancaire nous avons une forme d'union au sein de la zone Euro notamment, nous avons un fonds de résolution unique qui doit être doté de 55 milliards d'euros à l'horizon 2023 et qui était l'été dernier, doté de 24,9 milliards d'euros, nous avons un système européen d'ASUS d'assurance des dépôts qui prendra la forme d'un mécanisme commun de co-assurance en 2020, 2000 24 à hauteur de 45 milliards d'euros, face à cette union bancaire on peut relever 2 types de risques va plus structurelle concerne les prêts non performants, d'après une étude de l'OFCE, publiée l'an dernier le solde de prêts non performants qui n'a pas été provisionnés était de 395 milliards d'euros fin 2017, l'autre, celui d'une crise économique et financière dans les mois ou les années à venir, sur laquelle plusieurs économistes et responsables d'organisations internationales nous alerte déjà pour avoir une idée de l'ampleur potentielle d'une cuisse, d'un point de vue financier, on peut regarder les montants des aides d'État accordées aux banques après la crise entre 2018 et 2017, au cours de cette période, l'Union européenne avait déboursé 665 milliards d'euros en capital et 1296 milliards d'euros d'aide en trésorerie, ce chiffre ne saurait suffire à évaluer la robustesse de notre système européen mais ils donnent une idée des gens de grandeur hier au Sénat dans le cadre du débat qui s'est tenue sans vote malheureusement sur le programme de stabilité, vous avez déclaré que la zone Euro n'est pas armée pour faire face à ce une ce une nouvelle crise économique et financière et que les instruments mis en place après la crise de 2008 sont insuffisants, par conséquent, je vous pose cette question quel péril et de quelle ampleur nos finances publiques, si une crise financière se déclenche demain, personne ne peut l'exclure et quels instruments complet concret pardon pour y remédier, je vous remercie. La parole est à monsieur le Ministre. nous nous avançons monsieur le sénateur, mais nous avançons trop lentement et je ne veux pas que nous soyons pris de court par les événements Kariane pire en pilotis que d'être pris de court par les événements, nous avons mis en place mais, interrogé sur les instrument concrets, le backstop du fonds de résolution unique, le backstop, c'est le filet de sécurité qui permet de doubler le montant du fonds de résolution unique, donc il est de l'ordre de 55 milliards d'euros, nous aurons désormais avec ce filet de sécurité, le fameux backstop, environ 100 milliards d'euros de disponible en cas de crise financière, ce backstop, il sera disponible à partir de 2024 si nous pouvons avancer l'entrée en vigueur, nous le ferons et nous essayons d'y travailler, un des éléments absolument clé des décisions prises à Meseberg par le président de la République et par la chancelière allemande, nous avons aujourd'hui un fonds de réserve qui a été doublée par ce filet de sécurité qui porte le montant des réserves à 100 milliards d'euros, un peu plus que 100 milliards 2ème chose c'est l'assainissement des banques, vous avez parfaitement raison, il faut nous débarrasser le plus vite possible de ces fameux prêts non performants Les MPL qui sont dans le bilan des banques et qu'ils font encourir une menace la stabilité financière de la zone Euro, nous avons engagé là aussi le processus et nous avons fixé toujours dans le cas de Meseberg car les références se font à partir de l'accord de Meseberg franco-allemand, un niveau de prêts non performants un niveau cibles que nous sommes en train d'atteindre un rythme qui est tout à fait régulier, enfin 3ème élément que j'ai indiqué tout-à-l'heure il faut renforcer la supervision bancaire l'ensemble des banques européennes pour éviter les défaillances que nous avons vu aujourd'hui, notamment dans une grande banque danoise, enfin le dernier point sur lequel je veux insister, c'est qu'il faut de la consolidation bancaire en Europe. Bon sont trop petites. Et lorsque vous banques sont trop petites, ça empêche le développement économique et ça ou votre marché à vos concurrents américains, donc je crois à la nécessité d'une consolidation bancaire en Europe. La parole est à monsieur Cyrill Penn va pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme cela a été préalablement indiqué afin de soutenir les réformes et les investissements nationaux, la France et l'Allemagne ont émis une proposition commune pour la création d'un nouvel instrument budgétaire pour la zone Euro. Ce nouvel instrument fiscal qui ne sera pas mis en place avant 2021 aura pour objectif d'améliorer la compétitivité à la convergence parmi les pays de la zone Euro et les États candidats à la monnaie unique, la revendication du président Emmanuel Macron concernant la fonction stabilisatrice de ce budget en cas de crise n'a en revanche pas été retenu cet instrument ne permettra pas de soutenir un État en cas de crise la France et l'Allemagne estime néanmoins qu'avec plus de compétitivité de convergence à la stabilité de la zone Euro s'améliorent, ce nouvel instrument budgétaire pour la zone Euro peut sembler être utile en tant qu'instrument de convergence au niveau de la zone Euro, étant donné que la divergence est plus forte au niveau de la zone Euro, que de l'Union européenne, mais sans la fonction stabilisatrice, considérez-vous qu'il s'agisse d'une occasion manquée. Pour atteindre ses objectifs de compétitivité de convergence, ce nouveau fonds servira à financer les coûts occasionnés par les réformes et les dépenses d'investissements dans des domaines stratégiques liés aux réformes et aux priorités d'investissement identifiés au cours du semestre européen, il s'agirait surtout d'investissement dans l'innovation et le capital humain qui remplacerait des dépenses aujourd'hui purement nationale alors que le montant du budget de la zone Euro n'est pas encore fixé, puisqu'il sera déterminé lors des négociations du prochain budget européen pluriannuel en 2021 2027 je m'interroge sur la finalité peu précises et le fonctionnement de ce budget, monsieur le Ministre, pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce pour que, sur ce, ce que le budget est censée financer sa règle de fonctionnement sera-t-il utilisé sous forme de subventions ou de près, pourra-t-il servir à financer des investissements publics ou non, je vous remercie pour les réponses que pourrait nous apporter. La parole est à monsieur le ministre. La réponse est oui, monsieur le sénateur, le 20, c'est-à-dire que ces fonds d'investissement, le budget d'investissement de la zone Euro pourront servir au financement d'investissements publics. Ensuite, sur le fonds de stabilisation, j'ai pas revenir sur le sujet en 2 déjà longuement étudié mais je ne renonce absolument pas à ce que dans les années qui viennent, il y a une dimension de stabilisation dans le budget européen. R : je vais vous dire parfois on me dit mais c'est absolument de portée il y a des oppositions farouches très bien. Mais prenez des exemples très récents. L'opposition totale à des projets, la France. Le budget de la zone Euro. Beaucoup de gens, nous y sommes arrivés, prenez un 2ème exemple encore plus frappant les aides d'État il y a 5 ans, mais vous ne pouvez même pas prononcer le mot d'aides d'État des publics à des investissements dans l'innovation dans la recherche était impensable, on a apporté la preuve que c'était quand même compliqué de ne pas avoir des aides publiques à des projets d'investissement, là où les Chinois et les Américains se privait pas de le faire parce que SpaceX, n'est pas né comme ça tout seul du génie de monsieur SpaceX à profiter des installations, des infrastructures et des commandes de l'État fédéral américain et des installations de la Nasa. Et c'est comme ça qu'ils ont lance renouvelables aujourd'hui et que nous, hélas, nous n'en avons pas. La Chine subventionne massivement ces véhicules électriques et ses batteries électriques que leur noms serait là comme le dindon de la farce au milieu avec un libéralisme absolu, une croyance aveugle dans les forces du marché et à dire jamais d'intervention publique. Ce que je constate c'est que grâce à la persévérance française aujourd'hui, il est possible d'apporter des aides publiques des aides d'État à des projets d'innovation structurants et si dans 2 jours, je vais pouvoir annoncer avec Peter Altmayer, la création d'une filière pour les batteries électriques européennes qui nous permettent d'être souverain et indépendant par rapport aux batteries chinoise ou par rapport aux batteries sud-coréenne, c'est qu'on a accepté qu'au-delà des financements allemand des financements français d'entreprises privées, il y a aussi des aides d'État il y a aussi des aides publiques, c'est comme ça que l'Europe réussira ce n'est pas en répétant sans cesse un mantra idéologiques dépassés c'est en étant capable d'inventer l'économie du XXIe siècle. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues,

fut un acte économique fort autant qu'un acte politique politique fondamentale, il a procuré aux pays qui l'ont adopté des avantages économiques que nous avons tendance à oublier et nous donnerions tort de sous-estimer l'ampleur, il est surtout devenu le bien commun des 340 millions d'Européens qui l'utilisent aujourd'hui quotidiennement au cours de ces 2 décennies d'existence, la monnaie unique a dû surmonter bien des épreuves et nombreux sont ceux qui, à sa création, lors de la crise financière ou lors de la crise des dettes souveraines lui ont prédit avec certitude une fin aussi imminente que retentissante pourtant malgré les vicissitudes, les polémiques, l'Euro est toujours là et à ceux qui prônent sa disparition, les Européens répondent massivement par une volonté croissante au fil des ans de le préserver ne serait toutefois en déduire que le bilan de l'Union économique et monétaire est pleinement satisfaisant dans tous les domaines, certes le roi parfaitement joué son rôle de bouclier anti-crise monétaire et de stabilisateur des prix et d'échanges, et grâce aux réformes impulsées entre 2010 et 2012, conjugué à l'action de la Banque centrale européenne dans les moments décisifs, la zone Euro est aujourd'hui bien plus solide qu'à l'origine, mais la création de la monnaie unique porte en elle une promesse de prospérité qui n'a pas été suffisamment tenu dans tous les pays, après la crise devait engendrer une convergence naturelle ascendante des économies européennes, c'est au contraire et vous l'avez souligné à plusieurs reprises monsieur le Ministre alors évolution divergente que nous avons insisté pour remédier à cette situation, certains préconisent d'en finir avec ce qu'ils appellent le dogme de l'austérité, refusant de voir que les dérives budgétaires individuel dans les États-membres sont le 1er des risques pesant sur l'ensemble de l'édifice commun la responsabilité première de tout pays ayant fait le choix d'appartenir à la zone Euro reste donc de mener des politiques budgétaires non pas rigoriste mais équilibré ainsi que et surtout des réformes structurelles visant à relever son potentiel de croissance économique et là, Monsieur le Ministre, je voudrais vous avouer que nos analyses en ce qui concerne les réformes structurelles mises en place dans ce pays particulièrement divergent, d'autres comme le président de la République prône quant à eux une mutualisation de ces risques budgétaires par la création d'un budget de la zone Euro suffisamment conséquent pour mette sur pied une union de transferts permanents ou tout au moins pour assurer une fonction de stabilisation macroéconomique puissante, l'idée ne manque pas de fondements théoriques, j'avoue que ça peut paraître séduisant mais elle est aujourd'hui politiquement irréaliste tant les crises qui ont marqué cette décennie ont miné la confiance entre États membres et la force est de constater que la France au vu de son incapacité à redresser ses comptes publics et à transformer son économie n'est sans doute pas l'avocat indiqué pour défendre une telle évolution de la zone Euro, chacun a souvenir que c'est en 1974 que la France avait, pour la dernière fois équilibrer son budget, c'est donc avant tout en nous appuyant sur des réformes, les vrais que nous pourrons poursuivre le renforcement de l'union économique et monétaire et améliorer la situation économique structurelle de la sonore

à la majorité qualifiée, oui, 3 fois oui mais les résultats je dirais semble je dirais à tendre et en ce qui concerne la convergence l'union bancaire et l'Union des marchés de capitaux sont essentielles, leur achèvement permettrait d'une part de mieux absorber les chocs économiques en diversifiant les risques spécifiques aux différents pays de la zone Euro, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un budget commun de stabilisation. vous avez chacun a pu concevoir si vous voulez qu'il y a une différence tant dans l'analyse que dans la prospective entre l'approche allemande et l'approche française pour reprendre les mots de François Villeroy de Galhau, une union de financement contribuant à rétablir la circulation des capitaux dans les pays de la zone Euro serait essentiel l'épargne excédentaire dans un pays viendrait ainsi plus fils financer les investissements efficace dans un autre et soutenir la croissance, ce qui est l'un des objectifs d'une union monétaire pour améliorer la qualité de ses investissements, notons au passage qu'outre la poursuite des réformes structurelles nationales, l'émergence d'une politique industrielle européenne dans le secteur stratégique apporterait une contribution essentielle le temps me manque pour élaborer

il y a d'énormes progrès à faire, enfin, c'est une question qui a été porté abordé par beaucoup de nos collègues, la dimension de la zone Euro nécessite bien évidemment, si je puis dire que cette monnaie soit davantage utilisé dans les accords commerciaux internationaux, elle était au lendemain de la crise de Lehman Brothers, à hauteur de 40 pourcent dans les 2 ans qui ont suivi la crise de Lehman Brothers et les retombées aujourd'hui à moins de 30 pourcent et c'est la seule et véritable réponse à l'extraterritorialité des lois américaines sur fond de fragilité de l'Organisation mondiale du commerce, il y a pas d'autre tout solution que celle-ci, je vous remercie. Je Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16 heures 45 pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est suspendue.

La séance s'est reprise. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous remercie d'excuser le président Gérard Larché, en déplacement à l'étranger, je vous rappelle que la séance est retransmise en Direct sur Public Sénat sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, observé au cours de nos échanges, l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps, La parole est à Madame Sylvie Vermeil et pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le 1er ministre, mes chers collègues, jeudi dernier, le président de la République a annoncé les mesures qu'il souhaitait mettre en oeuvre, à l'issue du grand débat national ajouté à la suppression intégrale de la taxe d'habitation et aux mesures prises en décembre dernier la baisse prévue de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et la réindexation des plus petites retraites porte la facture à plus de 25 milliards d'euros, le chef de l'État a esquissé quelques pistes de financement, évoquant pêle-mêle l'abrogation de certaines niches fiscales aux entreprises un allongement de la durée de cotisation ou encore du bout des lèvres, la réduction des dépenses publiques, mais nul ne sait très bien aujourd'hui selon quelle méthode et quels ventilation quelles niches fiscales allez-vous rabotez ou supprimer le taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation sera-t-il concerné, quid de l'exonération d'impôt sur les sociétés des organismes d'HLM et des dérogations en faveur du mécénat au titre des économies budgétaires qui ne sont jusque là supporter que par les seuls colite le président de la République semble surtout miser sur les taux artificiellement bas de la Banque centrale européenne, par pur optimisme budgétaire merci dégradent ainsi ses prévisions monétaires pour se ménager plusieurs milliards de réserves budgétaires monsieur le 1er ministre la situation préoccupante de nos finances publiques exige beaucoup plus et beaucoup mieux, pouvez-vous nous indiquer quelle sera l'effort budgétaire de l'État, à quelle hauteur et dans quel ministère, je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des Comptes publics. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, merci merci pour votre question qui me permet d'aborder, effectivement, vous l'avez noté le financement et la manière dont nous allons mettre en oeuvre les mesures annoncées par le président de la République, ces mesures, vous l'avez souligné ce sont des mesures importantes, elles viennent s'ajouter aux mesures annoncées le 10 décembre dernier avec l'augmentation de la prime d'activité avec la diminution du taux de CSG payée par un grand nombre de retraités, ou encore avec l'exonération des heures supplémentaires, nous avons comme objectif, d'ici le 1er janvier 2020 la mise en oeuvre d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros la réindexation des pensions de retraite de moins de 1000 euros sur l'inflation et au 1er janvier 2021 la réindexation de toutes les pensions de retraite, nous avons fait la démonstration au cours des années précédentes, de notre capacité à la fois à tenir les engagements européens, je pense notamment au fait que pour la 2ème année consécutive, 2018 c'est terminé avec un déficit public inférieur à 3 pourcent est égal à 2,5 pour 100, soit 0,2 point de moins que les prévisions du PLF pour 2018 je pense aussi au fait que 2018 s'est caractérisé et c'est une première dans notre histoire contemporaine, par une diminution en volume de la défense de la dépense publique à hauteur de 0,3 à la fois par un pilotage extrêmement strict des dépenses de l'État par la maîtrise de l'augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à hauteur de 0,7 pourcent et par une amélioration des comptes sociaux de 4 milliards d'euros par rapport à 2017, le 1er ministre et le président de la République, ont indiqué que pour financer les nouvelles mesures nous précède oriente de manière la première piste consiste à dégager des économies budgétaires sur la dépense publique, nous l'avons fait en 2018 et nous pouvons à nouveau le fer en 2000 19 et en 2020 la seconde vise à réexaminer, un un certain nombre de niches fiscales dont bénéficient les entreprises avec une première précaution qui est de ne pas qu'on s'de ne pas toucher aux niches fiscales qui garantisse la compétitivité des entreprises et l'emploi, nous aurons à à débatte de cela d'ici au mois de juin, en juillet, à l'occasion du débat d'orientation sur les finances publiques et nous serons particulièrement à l'écoute, madame la sénatrice des propositions des parlementaires en la matière. Madame vermeil et vous disposez de 15 secondes pour une réplique. Je crois que redonner du pouvoir d'achat était un préalable indispensable mais il s'agit maintenant de redonner la confiance pour que ce pouvoir d'achat dope l'économie française et ne se dissimule pas en épargne pour redonner la confiance, il faut que l'État montre l'exemple qui prouve qu'il a la volonté de faire des économies et qu'ils les fassent je crois que c'est à vous d'ouvrir la marche parce que sinon nous allons tous cela raté. La parole est à monsieur Didier Rambaud pour le groupe, la République en marche. Madame la présidente, chers collègues, ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, lundi 4 individus étaient mises en garde à vue dans le cadre d'une d'une enquête pour association de malfaiteurs terroriste criminelle ils préparaient une attaque prochaine extrêmement violente son aux forces de l'ordre à brève échéance, 3 d'entre eux seraient connu pour des faits de droit commun, le dernier un mineur aurait déjà été condamné à de la prison pour avoir cherché à se rendre en Syrie, je sais que vous ne pourrez pas nous donner plus de détails sur cette affaire, confiée à la direction générale de la sécurité intérieure, mais je veux ici saluer le travail de nos forces de l'ordre et de nos services de renseignements qui ont permis de déjouer avec brio ce projet d'attentat contrôler leur c'est le 58ème attentats déjoué depuis 2015 à travers la police française, c'était une fois encore, toute une nation qu'le visait, dans un contexte de forte sollicitation, nos services de renseignement l'ensemble de nos forces de sécurité demeure fortement mobilisés pour prévenir de nouveaux drames humains, ils le sont depuis les terribles attentats de 2015, qui ont suscité un renforcement de notre dispositif de sécurité intérieure, si son utilité était encore approuver le projet d'attentat déjoué vendredi dernier démontre une nouvelle fois son efficacité c'était épisode vient surtout nous rappeler que la menace terroriste reste toujours présente et que nous concerne toutes et tous, pas seulement en France mais également à l'étranger, et nous pensons aux attaques perpétrées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, mais également à Colombo, au Sri Lanka, le terrorisme n'a pas de frontières, et nous sommes tous concernés, face à cette menace terroriste toujours bien réel, et même si le risque 0 n'existe pas, pouvez vous ne pouvez-vous nous dire si nous sommes dans cette lutte mieux armé qu'hier et nous préciser les moyens mis en oeuvre pour renforcer la lutte contre ce fléau, Parole est à monsieur Laurent Munier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez raison de de rappeler que, donc, il y a, vendredi, pour être précis, ont été Tintin interpellé 4 individus un mineurs et 3 majeurs qui s'apprêtait à commettre une action violente l'arme automatique et nous avions de bonnes raisons de penser que le passage à l'acte pouvait se faire à brève échéance, et donc sur autorisation bien évidemment instruction du parquet de Paris, ces individus ont été interpellés, vous comprenez que je ne peux pas vous en dire plus, mais répondent précisément à votre question, d'abord sur la nature de la menace, oui, la menace existe toujours à la une forme endogène avec des individus qui peuvent être présents sur le territoire et passer à l'acte en répondant à la propagande de Daech on a vu encore que Al-Baghdadi a diffusé ces jours derniers, hier, une une vidéo, et donc il faut être extrêmement attentif, le dispositif qui est mis en place qui a été mis en place sous le quinquennat précédent et puis renforcée par le président de la République par le 1er ministre vise à faire en sorte que l'ensemble des services de renseignements travaillent ensemble, sous la coordination de la direction générale de la sécurité intérieure, l'ensemble des individus, connu pour radicalisation sont suivis en renseignements je tiens salue également le travail qui est effectué dans l'administration pénitentiaire, avec le service du renseignement pénitentiaire et l'ensemble des services, échangent des informations sur les objectifs, pour s'assurer que tous sont bien pris en compte et suivi, je tiens à préciser naturellement que les moyens mis à disposition des services ont été renforcés, ils le seront encore cette année ou la DGS, il voit son budget augmenter de 20 millions pour des dispositifs techniques techniques de renseignement dispositif humain qui est renforcé avec des recrutements de plus de 1900 personnes au total sur le quinquennat dans les services de renseignement et le dispositif juridique, vous l'avez souligné avec la loi s'il te bien évidemment vous rassurer également ce dispositif fonctionne puisque ces individus n'était pas connue que pour des faits de droit commun, il était aussi suivi au titre de l'arrêt de la radicalisation et c'est dans le cadre de ce dispositif dont je viens de parler qu'ils ont été détectés, puis judiciariser, donc c'est à dire que les services de renseignement ont décidé de les poursuivre pour association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste, voilà ce que je pouvais voir apporter comme éléments de réponse en remercions et félicitons à mon tour, ceux qui ont été mes anciens collaborateurs, je veux saluer, donc l'ensemble des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure qui, sous l'autorité d'abord du du directeur général, puis ensuite du parquet de Paris on fait un travail remarquable qui a permis de jouer le 58ème attentat merci. La parole est à madame Mireille joue pour le groupe Rassemblement démocratique et social européen. Madame la présidente, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre, dans le cas de la restitution du grand débat, le président de la République a fait part de sa volonté de mener 2 réformes visant à favoriser l'apprentissage des fondamentaux à l'école la première consiste au sein du réseau d'éducation prioritaire dans l'extension aux grandes sections de maternelle du dispositif de dédoublement des classes actuellement mis en oeuvre pour les CP et CE1, la seconde, or des REP tend à plafonner à 24 élèves des effectifs des classes au sein de ces 3 mêmes niveaux d'enseignement, ces mesures ont vocation à être déployés sur l'ensemble du territoire d'ici la rentrée 2022, monsieur le ministre, nous nous en félicitons les efforts consentis sont tout à fait opportun, toutefois, à l'instar de l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, nous constatons que ces nouvelles évolutions engage ça peut certainement autant nos communes que l'État, d'après les chiffres communiqués par vos services le déploiement de la première mesure nécessitera la création de 6000 classes supplémentaires, quand la seconde requerra de 3000 à 5000 nouvelles classes une classe supplémentaire, c'est un enseignant supplémentaire mais pas uniquement, ce sont aussi des personnels municipaux et surtout des locaux municipaux supplémentaires, monsieur le Ministre notre Haute assemblée a débuté ce jour en commission, l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, il y sera notamment question du soutien financier de l'État aux communes dans le cadre de l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire et de l'évolution du forfait communal alloués aux établissements privés sous contrat, le dimensionnement de ce soutien fait largement débat auprès des maires, monsieur le ministre, l'annonce du 25 avril dernier a fait naître de nouvelles inquiétudes dans leurs rangs, pouvez-vous nous apporter des premiers éléments de réponse, y aura-t-il un accompagnement financier significatif des communes et ce, alors que 17 milliards d'euros de nouvelles mesures fiscales vont venir grever le budget de l'État. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs Madame la Serra sénatrice Mireille Jouve, les annonces du président de la République, concernant l'éducation, dans sa conférence de presse consacre une étape fondamentale dans l'histoire de l'éducation nationale, parce qu'elles consacrent le rôle de l'école comme vecteur de lutte contre les inégalités sociales, à ce titre, la mesure que vous avez rappelé de dédoublement des classes en grande session maternelle dans les territoires prioritaires et dans les quartiers prioritaires vient amplifier l'action qui est menée par Jean-Michel Blanquer depuis 2 ans et qui a conduit à dédoubler les classes en CP et en CE1 dans les rets et nous voyons des aujourd'hui les effets produits sur les élèves dans ces territoires, c'est des désapprentissage des fondamentaux plus rapide et c'est de la lutte contre les inégalités sociales, nous poursuivons avec les grandes sections de maternelle mais ces annonces, elle consacre aussi le rôle de l'école comme vecteur d'égalité des territoires et les mesures sont très importantes, vous en avez rappelé une qui est le plafonnement à 24 élèves par classe dans toutes les écoles pour les CP et CE1 c'est une mesure importante qui fait écho, je crois à beaucoup de débats que nous avons ici, que ce soit pendant les questions au gouvernement, ou d'autres textes, où un certain nombre d'entre vous sont intervenus pour donner des exemples d'écoles de leur territoire qui n'est pas en territoire en quartiers prioritaires avec un grand nombre d'élèves par classe, nous plafonnant à 24 élèves par classe, à l'avenir, c'est une mesure d'égalité des territoires, je veux aussi insister, puisque vous avez parlé des élus, vous n'avez pas rappeler, une mesure qui est très importante, qui est l'absence de fermeture d'école à l'avenir pendant ce quinquennat sans accord du maire, c'est aussi une mesure d'égalité des territoires, c'est aussi une manière de remettre l'élu le maire au centre du jeu, il y a eu ces 6 dernières années 2000, fermeture d'école, entre les ouvertures et les fermetures de 1000 Net, nous mettons fin à ce à ce ces fermetures, sans accord du maire, c'est une mesure qui est extrêmement importante pour le reste, je veux rappeler que sur l'abaissement de la scolarité à 3 ans des compensations sont intervenus ont été annoncées et seront déployés pour les communes, ça a déjà été annoncée par Jean-Michel Blanquer, ça fait un certain nombre de débats, d'ailleurs, dans les 2 sens et je suis sûr que ces débats continueront dans l'école, dans le projet de loi sur l'école de la confiance, je pense qu'il faut se réjouir, se réjouir de ces annonces, parce que je pense que ce qui peut nous rassembler toutes et tous, ici, c'est bien à cette question, l'apprentissage des fondamentaux, c'est bien que beaucoup se joue dès le plus jeune âge pour l'ensemble des enfants de notre pays pour la lutte contre l'équipe des inégalités et l'égalité des territoires, et je pense que ce sont de beaux débats qui continueront pendant le projet de loi sur l'école de la confiance, je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologistes. Merci madame la présidente, monsieur le 1er ministre, mes chers collègues dans la révision générale annoncée des niches fiscales accordées aux entreprises, vous annoncez maintenir en l'état, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, ainsi que le crédit d'impôt recherche afin, dites-vous, de créer des emplois, une politique qui n'a pas donné les résultats escomptés, alors que hier existent désormais depuis plus de 30 années, ce choix a un coût pour nos compatriotes 42 milliards d'euros pour le CICE et 6,2 milliards pour le hier, pour la seule année 2019, la France est championne d'Europe des aides publiques à la recherche et développement, aux entreprises, sans résultat probant vis-à-vis de nos voisins pour financer ces aides vont couper dans les dépenses publiques utiles à tous, selon l'OFCE, l'effort s'élève à plus de 20 milliards d'euros, la transformation en allégements de cotisations va mettre en péril le financement et le fonctionnement de notre système de protection sociale si ces dépenses créent de l'emploi aidés en priorité les petites et moyennes entreprises soutenaient les artisans de nos territoires, nous pourrions porter un regard bienveillant et pourtant cette ponction d'argent public n'a qu'un effet très limité sur l'emploi et profite d'abord aux plus grandes entreprises de même le crédit d'impôt recherche était de plus en plus utilisée comme un levier par les grandes multinationales pour faire financer la recherche par l'État français et transféré ensuite dans beaucoup trop de cas leur production dans des pays à bas coût, je vous sais féru de musique et Europe monsieur le 1er ministre, je vous laisse méditer ces paroles de Kurt Cobain, une idéologie est un système de pensée cohérent avec lui-même, mais non avec la réalité, fin de citation alors pourquoi monsieur le 1er ministre vous obstinez-vous à maintenir de telles mesures injustes et inefficaces. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des Comptes publics. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Bocquet seul sénateur, vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous ne partageons pas votre constat sur 2 points: le 1er point concerne le CICE, pour 2 raisons : d'abord parce qu'à compter de cette année 2009, le CICE n'est plus un crédit d'impôt, nous l'avons transformé en logement pérenne des cotisations payées par les entreprises et c'est la raison pour laquelle, en 2009, le coût pour les finances publiques s'élève à 40 milliards d'euros puisque ça vous savez aussi que nous soldons dans le crédit d'impôt dû au titre de l'année 2018, nous considérons que les crédits d'impôt créé en 2013 dont la pérennisation sous forme d'allégements de cotisations avait atteint, on sait dès 2016, mais dans la pérennisation est annoncé, a été finalement acquitté en 2019 est un outil utile pour préserver l'emploi et pour améliorer la compétitivité des entreprises concernant crédit d'impôt recherche nous considérons aussi que c'est un outil particulièrement efficace pour permettre le maintien de la compétitivité, le développement de programmes de recherche dans les entreprises, et ainsi permettre à l'industrie française et à l'économie française d'être plus forte sur la scène internationale, comme sur la scène européenne, y compris sur le territoire national, nous avons dit à l'occasion des différentes annonces d'abord par le président de la République, hier, par le 1er ministre que nous allions examiner un certain nombre de niches fiscales, celle dont bénéficient les entreprises, à l'exception de celle que j'ai, quelle que soit la nature du CICE et avec un souci majeur, qui est de préserver la compétitivité nous ne toucherons pas aux niches fiscales des ménages, celle qui donne du pouvoir d'achat, celle qui accompagne la rénovation thermique, c'est l'enfant qui permettent aussi l'emploi notamment de salariés à domicile, une grande partie des mesures ont déjà été a déjà été financés celle annoncée le 10 décembre à hauteur de 10 milliards d'euros, qui représentent environ 7 à 8 milliards d'euros seront financés à la fois par des économies sur la dépense publique et par la révision des niches que je viens d'évoquer nous referons en maintenant notre trajectoire budgétaire, nous le ferons maintenant et en respectant les engagements pris par le président de la République pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et nous le ferons avec le Parlement, et comme je disais Madame dernier nous attendons toutes les propositions, je termine, madame la présidente, en vous disant, Monsieur Bocquet, dans un clin d'oeil que j'ai cru comprendre

11 milliards 111 milliards d'euros accordés aux entreprises sous forme de créance fiscale entre 2013, 2018 pour 100 1000 emplois créés, selon France Stratégie mais nous apprenons il y a quelques minutes, que le géant la distribution Auchan dans ma région, annonce la suppression de 720 emplois sur 21 sites, ce groupe a touché 88 millions de ou d'Euro de CICE. La parole est à monsieur Rachid c'est mal pour le groupe socialiste et républicain. Merci a fait non plus chers collègues, mesdames, messieurs les ministres, ma question s'adresse au 1er ministre monsieur prémices à l'origine de la conférence de presse du président la République de la semaine dernière, 5 mois de crise sociale sans précédent, une crise dont vous n'êtes pas bien sûr intégralement responsable mais quand même crise déclenchée et amplifiée par une politique votre politique pour y pondre un président nous a dit qu'il découvrait les problèmes des Français du pays et qu'il restait convaincu que sa politique est dans le bon sens et c'est pour ça qu'il n'a pas convaincu les Français d'ailleurs, comme nous-mêmes, je prendrai 2 exemples d'abord la question du pouvoir d'achat, pas une fois le mot salaire dans les propos du président de la République, les retraites, il fera dorénavant travailler plus pour avoir une retraite à taux plein la réindexation des retraites, c'est pour plus tard et pas toutes les retraites pour autant pour l'ISF, il n'a pas vu autant de tergiversations et rapidement, vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de rétablissement de l'ISF alors que les Français le souhaitent sur les services publics et les territoires, alors qu'il faudrait entendre les locaux, vous leur demandez de faire plus, avait encore moins, alors tout à l'heure monsieur Attal nous a parlé de la non-fermeture des classes le mais ce qu'il oublie de rappeler c'est que dorénavant il y aura toujours la fermeture de classe dans les écoles et donc Monsieur Blank a l'a rappelé il y a quelques jours, donc encore une fois une promesse déjà non tenues,

à vos projets sur les retraites à vos projets sur la son chômage mais pourquoi pas commencer par un 1er vrai sujet : la question des salaires et faire en sorte que les engagements pris par les uns, les par les autres et qu'ils soient tenus et public. La parole est à madame qui pète Ndyaye, secrétaire d'État au. Près du 1er ministre porte-parole du gouvernement. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous le savez, vous l'avez dit vous-même dans votre intervention, la crise des gilets jaunes est une crise inédite qui a révélé bien des inquiétudes qui traversent notre pays au cours de cette crise, nos concitoyens ont exprimé une triple inquiétude à la fois une inquiétude vis-à-vis d'un sentiment d'injustice fiscale mais au également d'injustice sociale et enfin d'injustices territoriales dès le 10 décembre 2018 par un 1er train de mesures et, ensuite, lors de sa conférence de presse de la semaine dernière, le président de la République a apporté un certain nombre de mesures, à un certain nombre d'annonces à la fois des chantiers qui ont été ouverts pour l'avenir, mais également des mesures extrêmement concrètes et j'y reviendrai, ces annonces ont été complétés à la suite du séminaire de la majorité et du gouvernement par un calendrier que je qualifierais de calendrier d'efficacité qui a été présenté par le 1er ministre et qui permet de mettre sur les rails de manière opérationnelle et concrète l'ensemble des annonces qui ont été réalisées par le président de la République, au fond, que nous permettent de faire ses annonces, elles nous permettent de répondre à la fois au sujet de l'injustice fiscale, c'est l'annonce d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros dès le 1er janvier 2020 et ça c'est du concret, c'est également des réponses à l'injustice sociale, je crois que vous avez oublié un peu vite, monsieur le sénateur, en parlant de la question des salaires la l'augmentation de 100 euros de la prime d'activité dont bénéficie aujourd'hui dont bénéficie aujourd'hui, sauf qu'à la fin monsieur, c'est de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes dans la dans la poche des français et ça, c'est une réponse de justice sociale, vous avez également oublié de mentionner les pensions alimentaires qui désormais pourront être recouvrée directement par un tiers, en l'occurrence la Caisse d'allocations familiales et c'est une réponse importante à l'attention des femmes qui, aujourd'hui, vivent des situations désespérées lorsque leur conjoint ne versent pas la pension alimentaire, enfin sur la question de l'injustice territoriale, monsieur le sénateur vous zoom était de parler du lancement 2 d'une nouvelle étape de décentralisation Alain quand elle nous sommes attachés et qui vous permettra de résoudre ces inégalités merci. La parole est à monsieur Claude Malhuret pour le groupe, les indépendants républiques territoires. Monsieur le madame la présidente, monsieur le 1er ministre, mes chers collègues, l'actualité est marquée par l'effroyable attentat du 21 avril dernier au Sri Lanka, la vidéo menaçante du calife Abubaker El Baghdadi, la multiplication des attaques terroristes au Sahel et leur extension préoccupante dans plusieurs pays d'Asie, elle confirme que, comme l'avait annoncé, de nombreux spécialistes du renseignement, la défaite sur le terrain de l'État islamique en Syrie et en Irak ne signe pas la fin du terrorisme international, mais pourrait bien au contraire préluder à sa recrudescence et à une nouvelle stratégie de globalisation, la France, nous le savons tous car nous l'avons chèrement payée est une des cibles principales : d'abord parce qu'elle est une terre occidentale de liberté mais aussi en raison de son action contre le terrorisme dans le monde entier, notre pays est en première ligne dans la zone stratégique constitué par plusieurs pays sahéliens il a activement combattues les djihadistes au Moyen-Orient et la visite du président du Sénat et de sa délégation qui rencontreront aujourd'hui ou demain, les militaires de l'opération Chamal pour les remercier et les féliciter en est l'illustration en France même les forces de l'ordre, continue d'être l'une des cibles privilégiées du terrorisme, comme en témoigne l'attentat préparé contre elle, déjouée vendredi dernier et je voudrais à mon tour, salué le dévouement et l'efficacité de nos services de sécurité, mais elles ne sont bien sûr pas les seuls visés, compte tenu des signes convergents que semble indiquer l'ensemble de ses actualités, pouvez-vous, Monsieur le 1er ministre de faire le point sur la situation de la menace terroriste et nous dire si elle appelle de la part du gouvernement des mesures particulières mais pouvez-vous nous dire également si elle appelle à adapter notre intervention et notre soutien aux pays du Sahel, dont certains sont dans une situation critique, je vous remercie. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président malgré. Nous avons tous je crois et le monde entier, elle a été été choqués par la violence des attentats qui se sont déroulés au Sri Lanka, au moment de Pâques. Pour avoir vu dans notre pays et parfois connu directement. De tels attentats pour avoir vécu de telles scènes nous nous faisons une représentation très claire de l'horreur qui s'est déchaînée au Sri Lanka et nous adressons évidemment toute notre sympathie, notre amitié aux autorités plus largement au peuple srilankais, confronté à cette vague de violence terrible. Vous évoquez Monsieur le Président, la menace terroriste, la menace terroriste à l'étranger et la menace terroriste sur notre territoire. Cette menace terroriste, vous avez raison de le dire, Monsieur le Président allez-permanente. Et Et il y a quelque chose de singulier, a constaté que dans les périodes de calme, il y en a parfois. Rappeler que cette menace terroriste était imminente et permanente donne parfois le sentiment, à certains que l'on voudrait jouer sur les peurs. Et puis quand parfois malheureusement un attentat se produit ou Kant heureusement un attentat et déjoué, alors on se rend compte pendant un instant, qu'en effet, cette menace est puissante et permanente. à l'étranger, nous pouvons aider un certain nombre d'États à lutter contre la menace terroriste qui de manquerait pas d'avoir des répercussions sur nous-mêmes. Nous faisons par des politiques d'échange d'informations et de bonne Intelligence entre services de renseignement avec une très grand nombre d'États dans le monde et cet échange d'informations est cruciale, la capacité à travailler en confiance avec des services de renseignements sur ces aspects est absolument crucial et je sais que les services français pratique ces échanges d'informations avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux et que c'est à un élément très important de notre défense collective, nous nous sommes engagés militairement dans la lutte contre le terrorisme en Syrie, c'est vrai, ou Daech a été vaincu et il faut s'en réjouir mais vous avez raison, dire : Monsieur le Président Malhuret que la défaite militaire de Daech en Syrie ne fait pas disparaître la menace terroriste à l'étranger, comment la menace terroriste en France d'autres zones dans le monde sont ou deviennent des réservoirs et des lieux de non-droit où peuvent se développer telle ou telle groupes se reconstituer telles ou telles alliances se former telle ou telle cellule, c'est la raison pour laquelle, après l'intervention décidée par le précédent président de la République, François Hollande, au Mali, nous sommes restés sur place pour accompagner la lutte contre des mouvements terroristes et pour éviter la recomposition de cellules ou de routes qui viendraient nous impacter directement. Sur le plan national, la menace est endogène. Certes le califat a disparu, mais nous savons que, partout en France, il peut y avoir des basculements des passages à l'acte, nous l'avons constaté à Strasbourg en décembre et qu'il est très difficile de les prévenir, ou de les identifier, mais nous savons aussi que les services français se livre à un travail remarquable de concentration, de sérieux, de vigilance et que le chiffre a été donné tout à l'heure, depuis 2015 c'est près de 58 attentats qui ont été déjoués. Ce sont des victoires silencieuse, on les évoque, et nous nous en réjouissons, la vérité c'est que ce sont des victoires silencieuse mais ce sont des victoires, et nous devons féliciter et saluer le remarquable travail de ceux qui, souvent dans l'ombre, nous protège et nous protège efficacement au sans se faire d'illusions sur l'idée que le risque 0 pour être totalement assuré, il n'existe pas, mais en mettant le meilleur d'eux-mêmes dans une lutte de tous les jours, nous accompagnons ce travail à la fois juridiquement, financièrement et organisationnellement. Mesurons bien l'effort. Juridiquement, c'est la loi et c'est la sortie de l'état d'urgence pour faire en sorte que notre dispositif juridique soit en dehors d'un loi d'exception qui date de 1955. Financièrement, c'est en donnant plus de moyens, notamment la DGSE 1000 900 recrutements supplémentaires pour la DGSE sur la durée du quinquennat c'est plus d'hommes et de femmes plus de compétences plus de capacité à bloquer des évolutions vers la radicalisation ou vers le passage à l'acte et une plus grande efficacité opérationnelle avec la création du coordonnateur national du renseignement et la lutte contre le terrorisme, avec le rôle de coordination opérationnelle, confie à la DGA, si cela peut sembler ça peut sembler des mots mais la coordination opérationnelle par la DGS, il a effectivement donné des résultats dans la lutte contre le terrorisme, cette, enfin toute une série de mesures sur le renseignement pénitentiaire qui sentent absolument décisif et c'est la création récente du parc national antiterroriste qui permettra, du point de vue judiciaire une meilleure coordination des procédures, enfin, je voudrais dire qu'on ne combat pas monsieur le président, la menace terroriste, simplement par des mesures sécuritaires au judiciaire, nous en avons parfaitement conscience, cela passe à la fois s'agissant de la menace à l'extérieur par des politiques de coopération et d'aide au développement, elle semble, elle semble presque. La menace est tellement grande, la tâche est tellement immense, que dire que nous allons augmenter l'aide publique au développement, dire que nous allons aider des des politiques locales de développement économique de développement culturel ça ne semble pas la mesure de la tâche, mais la vérité c'est que c'est le seul moyen de lutter efficacement et dans la durée et puis nous voulons sur le territoire national nous livrer à une lutte sans merci contre l'ensemble des territoires et l'ensemble de ceux qui veulent remettre en cause le pacte républicain, un mot pour vous dire, Monsieur le Président, durée et j'en conclurai car je sais que je réponds très longuement mais on connaissait que le sujet s'y prête de 9 depuis depuis février 2018 nous avons fermé 4 écoles hors contrat où nous avions des raisons de penser que des thèses qui pouvait conduire à la radicalisation était développé, nous avons fermé 7 lieux de culte, nous avons fermé 8 établissements culturels ou associatifs, nous avons fermé 89 débits de boissons pour les raisons que j'évoque, parce que des thèses ou des mouvements étaient en train de scier organisé la loi d'avril 2018 prise à l'initiative d'une de vos collègues Madame Castel a permis 15 procédures d'opposition à des écoles, donc nous avions des raisons de penser qu'elle ne respecterait pas le pacte républicain et qu'elle pouvait être un lieu de radicalisation, autrement dit, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, oui, la menace est permanente et je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que si je ne vous disais pas ça je vous mentirais oui, la menace est permanente, mais la détermination des forces de sécurité et de l'ensemble de ceux qui concourent à la sécurité de ce pays est totale pour être à la hauteur des enjeux et pour offrir le plus grand niveau de sécurité possible à nos concitoyens, je vous remercie, monsieur le président. La parole est à monsieur Jean-Pierre Leleux pour le groupe, les républicains. Merci madame la présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la culture Monsieur Ministre le soir du dramatique incendie qui a ravagé, Notre-Dame de Paris, le chef de l'État s'est engagé à une restauration complète de la cathédrale, dans un délai de 5 ans, j'avais alors pensé qu'une émotion bien légitime d'ailleurs avait occulté un réalisme de bon aloi, compte tenu de l'absence totale de diagnostic quant aux dommages subis mais cette détermination affichée s'est confirmé dans les jours qui ont suivi par le dépôt d'un projet de loi rédigée à la hâte, pourvu d'une étude d'impact sommaire et soumis à une procédure accélérée, or ce texte opère des choix qui me paraissent aussi étonnant que dangereux outre il confie la mission de reconstruction un établissement public créé pour l'occasion, alors que le pic ou le CMN seraient des opérateurs tout à fait compétent pour ce rôle, il prévoit dans son article 9 je cite des mesures d'aménagement et de dérogations en matière d'urbanisme, d'environnement, de construction et de préservation du Patrimoine, Monsieur le Ministre, de quels aménagements et de quelle des grosses dérogation, s'agira-t-il la production de nos monuments historiques est assurée par un ensemble de lois et de règles déontologiques, issu d'une très longue tradition française, la France figure parmi les pionniers en la matière, il serait très périlleux d'initier des dérogations qui plus est par voie d'ordonnance moyen redoutable d'éviter le débat la France dispose par ailleurs des meilleurs spécialistes de la protection du Patrimoine, y compris dans votre ministère, je m'interroge donc également sur le concours international d'architecture envisagée pour reconstruire la flèche de la cathédrale, prenons garde Monsieur le Ministre, qu'après avoir connu l'outrage des flammes, l'intégrité de Notre-Dame ne soit pas mise à mal par des innovations visant à la ronde, selon l'expression même du président de la République, plus belle encore et à votre avis, que veut dire, dans ce contexte, cette expression, plus belle encore.

lundi 15 avril nous étions tous bouleversés par les images que nous avons vu de Notre-Dame de Paris en flammes et je dois dire, et vous le savez bien que sans le travail extraordinaire le courage, la compétence et le sang-froid des sapeurs-pompiers de Paris, le drame aurait pu être bien pire qu'il n'a été, lundi, et je dois dire que depuis lundi aussi le travail des équipes du ministère de la Culture a permis, en lien avec les sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi avec les sapeurs-pompiers, de tout l'Île-de-France de sécuriser de sécuriser, Notre-Dame de Paris pour éviter, pardon, excusez-moi de d'éviter que les drames, soit, plus grave encore, depuis, nous avons pris rapidement Salon de dispositions, notamment à travers la loi que nous allons vous soumettre pour faire en sorte d'avoir un dispositif notamment fiscales spécifiques pour accompagner l'engouement des Français le la générosité des Français si la question concerne la loi, la générosité des Français pour Notre-Dame de Paris et nous avons mis et nous allons pouvoir en débattre ensemble un certain nombre de dispositifs qui nous permettront d'avoir le meilleur dispositif législatif pour restaurer de la meilleure façon possible Notre-Dame de Paris, nous en discuterons ensemble mais je suis le garant des principes fondamentaux de la préservation du Patrimoine, et vous pouvez compter sur moi pour avec les équipes du ministère de la culture, les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des Bâtiments de France qui oeuvrent en ce moment même sur Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Paris, que tout, que tous les dispositifs qui vise à préserver le Patrimoine seront respectées pour Notre-Dame de Paris, mais, Monsieur le Sénateur, ne nous privons pas de dispositif qui nous permettrait effectivement de restaurer Notre-Dame de Paris, à la hauteur de ce qu'est notre dame de Paris pour toute l'humanité la créativité, ce n'est son la créativité des architectes s'exprimer et le moment venu, nous déciderons de restaurer à l'identique ou de restaurer, en tenant compte de ces gestes architecturaux. la parole est à monsieur Dominique Théophile pour le groupe, la République en mars. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, madame la Ministre, la faculté de médecine et de la de Desanti et de la Guyane, il y a sept Bastareaud existe depuis 1988 et elle doit désormais jouer pleinement son rôle dans la formation des futurs médecins de la région nous étudions partent vers l'Hexagone, à partir de la 4ème année afin de pots suivent le pas au cours, ils sont ainsi accueillis d'un des universités déjà surchargé et avec la réforme du numerus clausus, l'accueil de nos autres fusions deviendra encore plus difficile pour rappel, le numerus clausus est à ce jour à 5 de 140 pour les Antilles, et 20 pour la Guyane, de plus, le départ des étudiants en métropole ne favorise pas le retour sur nos territoires qui manque pourtant cruellement de médecins, en effet, seule la moitié d'entre eux choisi de revenir la faculté a pourtant acquis un savoir-faire, de qualité, elle Aspire légitimement à une évolution à la mesure des besoins de la région de plus, nous avons une recherche épidémiologique et clinique d'excellence madame la Ministre, l'université doit s'inscrire pleinement dans la déclinaison régionale de la stratégie de transformation du système de santé et offrir une formation complète et de qualité dans le contexte actuel, il est difficile d'attirer ou de retenir les meilleurs spécialistes dans nos territoires et de nourrir le réseau d'émettre ces 2 villes et des praticiens hospitaliers, l'accès de nos patients au sur-spécialités de recours, mais aussi à une médecine de proximité en est obérée par ailleurs l'enjeu du positionnement des pays avoisinants et cruciale du point de vue de la recherche et du bassin de population de nos hôpitaux cette demande vous a déjà été adressée par l'université des Antilles, il s'agit pour l'université du projet le plus important pour les années à venir, inscrit dans sa stratégie de développement et d'ouverture à l'international, cela permettra d'affirmer son ancrage dans la zone Caraïbes ma question sera donc la suivante : à quand la mise en place d'une faculté de médecine Antilles-Guyane de plein exercice. La parole est à madame Frédéric Widal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche de l'innovation. Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Dominique Théophile, vous l'avez rappelé l'université des Antilles à un 1er cycle des études médicales et un 3ème cycle des études médicales mais pour la formation des médecins durant le second cycle, effectivement, les étudiants sont envoyés sur l'ensemble du territoire métropolitain pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur profession, l'université des Antilles est actuellement en cours de. L'examen, en plus de la loi de 2015, est actuellement en cours d'examen par une mission parlementaire, de manière à s'assurer que la séparation entre l'université des Antilles et l'Université de Guyane, poursuit son cours et j'ai moi-même demandé à François Weil de d'avoir une mission auprès d'université des Antilles pour le gouvernement, pour la ministre des Outre-mer pour moi-même, il est effectivement extrêmement important de nous assurer du développement du système de soins et du développement de la formation en santé au sein de l'université des Antilles

à l'université des Antilles et l'important pour le gouvernement, vous le comprendrez, c'est bien de nous assurer de la présence de terrains de stage suffisant pour assurer une formation complète médical au sein de l'université des Antilles dans le cadre du projet de loi de santé, un amendement a été proposée par des députés, et a été donc inscrit dans la loi qui nous permettra de faire un rapport précis sur la pertinence de l'ouverture d'une formation complète en médecine, notamment au regard du rayonnement de l'université des Antilles dans l'arc caraïbe, je vous remercie. La parole est à monsieur Guillaume chevreuils et pour le groupe, les républicains merci madame la ministre. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, après la conférence du président de la République et après votre séminaire gouvernemental du flou toujours du flou mais pas sur le dérapage des déficits publics, au moment où la croissance faiblit, vous avez fait le choix de creuser le déficit, comme l'indiquait un ancien rapporteur général de la Cour des comptes interrogé suite à vos annonces, le déficit public se dégrade et votre politique budgétaire menace la cohérence de la zone Euro à long terme, pourtant le candidat Emmanuel Macron le disait lui-même : ne pas réduire nos dépenses courantes et notre dette serait irresponsable pour les générations à venir et il avait raison, mais 2 ans après ses belles paroles, l'État dépense encore plus que sous la présidence de François Hollande, il faut tout de même le faire, et sans faire d'économies structurelles en effet vous supprimez 23 milliards de taxes d'habitation, comment on finance et surtout qu'elles sont les compensations pour les collectivités locales, fin 2018 vous tentez d'acheter la paix sociale avec un chèque de 10 milliards et aujourd'hui, vous annoncez 5 milliards de réduction d'impôts là encore comment finance la réalité c'est que c'est la dette qui paye, c'est de l'impôt, c'est de l'impôt pour nos enfants, sur qui vous vous déresponsabilisé, vous aviez promis le réenchantement une révolution destinée à construire la prospérité du XXIe siècle, le soulèvement populaire récents le déclassement d'une partie des Français, l'inquiétude de nos concitoyens pour leur avenir, illustre l'effondrement de cette illusion, alors Monsieur le 1er ministre quelle France voulez-vous transmettre aux générations futures et quel est votre objectif de dette pour la fin du quinquennat. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des coûts qui publie. Merci à Madame la Présidente, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Chevrolet, vous dressez un tableau sombre. Une situation qui n'est pas la situation des comptes français cette situation que vous décrivez n'est pas la vraie situation et vous me permettrez de d'illustrer cette affirmation mon tour par 4 chiffres d'abord pour dire que, en 2018 l'année comptable s'est terminé avec un déficit de 2,5 pourcent au lieu des 2,7 prévues dans le PLF c'est la 2ème année consécutive que la France respecte son engagement à être en dessous de 3 pourcent ça n'était pas arrivé depuis 2006, la 2ème, chose que je voudrais souligner, c'est que, en 2018 toujours, la dépense publique, pardon en volume a diminué de 0,3 pourcent et c'est la première fois de l'histoire contemporaine, cela s'explique par la maîtrise des dépenses de l'État, cela s'explique par le fait que les collectivités ont maîtrisé leurs dépenses de fonctionnement avec N'augmentation de seulement 0,7 pourcent et de 0,3 pourcent pour celle, celle des collectivités qui ont accepté le principe de la contractualisation les comptes de la Sécurité sociale se sont améliorés de presque 4 milliards d'euros par rapport à 2000 et le taux de prélèvements obligatoires est passé de 45,2 45 pourcent du PIB, ce qui signifie que nous avons commencé à diminuer la pression fiscale sur nos compatriotes sur les contribuables, ces 4 chiffres monsieur le sénateur, illustre le fait que ce que vous avez décrit comme situation n'est pas la réalité de la situation des comptes publics, vous nous interrogez vous interroger le 1er ministre sur la France que nous voulons laisser et la France plutôt que nous voulons construire si vous me permettez cette nuance : nous voulons construire une France qui soit maîtresse de son destin qui ne soit pas à la merci des marchés qui ne soit pas à la merci d'un endettement public trop important de génération en génération nous avons transmis sur nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes : nous voulons une France où la dépense publique soit efficace, une France où la dépense publique aussi synonyme synonyme, d'attention aux plus fragiles et d'accompagnement du développement et du progrès de chacun dépend de notre société, ces objectifs, nous les poursuivrons avec de la rigueur avec la maîtrise des comptes, je le répète, les 2 exercices 2017, 2018 et l'exercice que nous vivons en 2019 avec pistes de financement des mesures que j'ai évoquais en réponse à la question de la sénatrice dernier démontre que nous pourrons s'y arriver sans renoncer à nos objectifs, ni comptable ni politique. La parole est à madame d'Isabelle ah pardon. Pardon, vous avez 16 secondes mais une réplique, je vous en prie, chers collègues. Merci la présidente, monsieur le ministre, vous serez jugés sur les résultats de votre politique à la fin du quinquennat aujourd'hui vous ne maîtrisez pas la dépense publique, alors que vous devriez la diminuer la majorité sénatoriale vous fait des écoutez-nous et de plus votre gouvernement et président de la République donne des leçons à nos partenaires européens, au lieu de montrer l'exemple sur la gestion publique. La parole est à madame, qui s'appelle Raymond pas vivront. Pour le groupe, les républicains. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues monsieur le 1er ministre l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales et vient de publier sa dernière enquête de victimisation, les chiffres sont inquiétants, la délinquance a explosé en 2018 par rapport à l'année 2017 qui marquait déjà une très forte hausse des actes délictueux, augmentation de la délinquance malaise croissant des forces de l'ordre, allant jusqu'au suicide, tirent leur source de la même cause, une incapacité à prendre en compte les besoins de ce qui nous protège le président de la République pendant sa très longue intervention la semaine dernière n'a pas fait allusion à la question de la sécurité des Français monsieur le 1er ministre la responsabilité de cet échec incombe à votre gouvernement, inutile de me répondre que cette hausse est la faute des gilets jaunes en 2017 il n'y avait pas de gilet jaune inutile la demeure répond que cela vient de loin, l'augmentation de la délinquance ne peut être considérée comme une fatalité, comptez-vous, Monsieur le 1er ministre revoir la feuille de route des ministères de l'Intérieur et de la justice afin de mettre un terme à la croissance de l'insécurité dans notre pays.

de, de, de vous répondre d'abord de m'étonner, des chiffres que vous annoncez, puisque la délinquance en 2018 n'est pas si catastrophique que ça, je crois que pour vous rappeler que les cambriolages ont baissé, les atteintes aux biens ont baissé, les vols dans les véhicules ont baissé, je pense que vous devez confondre avec le 1er trimestre 2019 qui effectivement au 1er trimestre 2019, effectivement, nous enregistrons une hausse des items de la délinquance et notamment des atteintes aux biens des cambriolages, effectivement, mais uniquement au 1er trimestre 2000 19 et pas en 2018 simplement vous dire que nous avons bien conscience du travail des policiers et des gendarmes qui est devenue bien plus compliqué, cela ne vous a pas échappé avec la menace terroriste, nous en parlions un il y a un instant, avec de nouvelles menaces comme les menaces cyber et la cybercriminalité, avec également de nouvelles missions qui leur sont dévolues, comme la gestion de leur public qui balance ou ceux qui basculent souvent en violences urbaines en émeute et donc nous devons préparer les policiers à tout cela, que faisons-nous pour répondre à cela, je crois que vous le mettez dans le panorama vous fête ses 10000 emplois en plus sur l'ensemble du quinquennat ce sont des moyens budgétaires en plus, c'est 300 millions par an que nous allons investir dans l'immobilier pour la police nationale pour la gendarmerie nationale, ce sont des policiers et des gendarmes que nous déchargeant des tâches indues, notamment des tâches procédural des tâches administratives, des gares statique pour qu'il soit présent sur le le terrain et faire ce qu'ils aiment faire, être présent auprès de nos concitoyens et lutter effectivement effectivement contre la délinquance, donc nous engageons énormément de moyens en faveur des policiers et des gendarmes nous concevons de nouvelle doctrine opérationnel qui empêche comme c'était trop le cas auparavant, il y a 10 ans, c'était encore le cas, on travaille en tuyaux d'orgue c'est fini, nous déployons des dispositifs de coopération le 1er ministre- cela dit pour la lutte antiterroriste, je pourrais longuement développé tout ce que nous faisons en matière de lutte contre les stupéfiants ou les services apprennent à travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre la délinquance et vous savez sur certains territoires, nous avons multiplié par 5, les réseaux de stupéfiants démantelé, ceux-là même qui viennent gangréner Nossiter causer tant de tracas à nos concitoyens, policiers et gendarmes sont efficaces et la politique du gouvernement, l'est tout autant en matière de sécurité intérieure. contre le malaise des forces de l'ordre et l'augmentation de la délinquance, vous le savez, par votre expérience, vous n'aurez des résultats que si le management de la police n'est pas profondément revu si la réponse pénale aux actes délictueux n'est pas certaine, et enfin, si une loi de programmation sur la sécurité intérieure ne vient pas pas aux policiers et aux gendarmes les moyens dont ils ont besoin, si tout ne peut pas être rattrapé rapidement, il est nécessaire d'ouvrir une perspective positive pour redonner le moral à nos forces de l'ordre. La parole est à Monsieur André Vallini pour le groupe socialiste et républicain. Merci madame la présidente, madame la Ministre des armées depuis 4 ans une guerre fait rage au Yémen, cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts. Plus de 70000 à ce jour, dont une grande majorité de civils, des femmes, des enfants, des vieillards et le Yémen connaît aujourd'hui la crise humanitaire et alimentaire qui est sans doute selon plusieurs ONG, la plus grave de l'histoire contemporaine. Cette guerre est conduite, chacun le sait, par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, grâce à des avions grâce à des bombes grâce à des canons grâce à des navires fabriqué en France,

les navires sont notamment utilisés pour un blocus de nourriture et de médicaments, un blocus qui peut être considéré en vertu des critères de l'ONU comme un Crime de guerre, quant au traité sur le commerce des armes dans la France est signataire, je rappelle qu'il interdit aux États d'exporter du matériel militaire s'il existe un risque que ce matériel soit utilisé pour des violations graves et répétées du droit international humanitaire. Violation dont la France pourrait donc être. Complices au Yémen, alors Madame la Ministre, ma question est simple : pouvez-vous nous garantir que ce n'est pas le cas.

la France est depuis longtemps engagée en faveur du processus de paix et le gouvernement encore récemment reçu l'envoyé spécial de l'ONU Monsieur Greenpeace et lui a réitéré son plein soutien dans sa mission ô combien difficile. Alors croire que cet horrible conflit disparaîtrait si la France mettait fin à son partenariat avec l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes unis et faux, on ne peut pas abandonner des pays qui eux-mêmes font face à des menaces telles qu'Al-Qaïda cette organisation qui est celle qui nous a frappé sur notre propre sol en 2015. Le gouvernement n'a jamais nié l'existence d'armes d'origine française au Yémen. Ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas de preuve que ces armes ont été employées contre les populations civiles et vous le savez fort bien, monsieur le sénateur, pour avoir été vous-même ministre au Quai d'Orsay, l'autorisation de vendre des armes n'4 d'être accordée qu'après un examen interministériel rigoureux auquel le Quai d'Orsay lui-même participe cet examen pardon tient compte de différents critères : la nature des matériels, l'utilisateur final, le respect des droits de l'homme, la stabilité régionale, la nécessité de lutter contre le terrorisme et aussi la sécurité des civils qui font partie des critères qui sont pris en compte pour délivrer ou pas des autorisations de licence, alors oui, nous avons un dialogue très franc avec l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sur l'urgence qu'il y a à sortir de ce conflit car la France n'a qu'un objectif, c'est la fin de cette guerre. les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique, le Canada, ont suspendu tout commerce d'armement avec l'Arabie Saoudite, pourquoi la France ne fait pas de même j'ajoute que des journalistes français qui enquêtent sur ce dossier sont actuellement inquiété par la DGS il est on ne peut que dénoncer cette atteinte à la liberté de la presse.

Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces, il a notamment essayé de rassurer les maires et les élus, mais ces élus et notamment les élus ruraux se demande quel sera leur devenir quant à leur statut, et surtout, surtout, quels moyens financiers se verront attribuer ces collectivités, peut-on aujourd'hui avoir quelques orientations sur ces 2 points, le statut de l'élu et les ressources des collectivités locales seront-elles encore une fois, par la volonté de faire des économies, d'autre part, le président souhaite mettre en oeuvre une nouvelle loi de décentralisation améliorant la loi notre qui pose problème, qu'Alain Soral le calendrier et quelles compétences seraient concernés, par ailleurs, avec la suppression de la taxe habitation, il ne reste plus que le foncier maire comme ressources financières avec les économies demandées, le peu de ressources fiscales, les maires de ces petites communes ne savent plus comment financer leurs projets cette perte d'autonomie financière, ajoute aux difficultés à se faire entendre au niveau des intercommunalités et la crise de vocation pour les prochaines municipales risquent d'être bien présente, j'espère, monsieur le 1er ministre que vous avez noté la lassitude de ses élus et la complexité de mettre en place une véritable politique de développement local alors Monsieur le 1er ministre à moins d'un an des prochaines élections municipales, il devient urgent d'exposer aux élus ruraux et au futur candidat des ressources dont pourront bénéficier ces mêmes collectivités, il en va de notre démocratie car pour présenter un projet municipal, parce que ce sera tout simplement le lien étroit avec les élections municipales, il faut savoir sur quelles ressources on peut compter, sinon ce ne seront que des promesses qui ne pourront pas être tenues, je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des Comptes publics. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, lu, vous avez évoqué dans votre question, la nature et l'intensité du lien entre l'État et les collectivités territoriales, permettez-moi de vous répondre en 3 points, 3 points qui ont été évoquées hier à l'occasion du séminaire du gouvernement par le 1er ministre et en écho bien évidemment. En application des décisions annoncées par le président de la République, nous avons 3 chantiers devant nous, qui concerne les relations entre l'État et les collectivités territoriales, un 1er chantier concerne de manière extrêmement précise le statut de l'élu, le statut des maires en particulier et la nécessité d'apporter un certain nombre de corrections d'améliorations au texte qui régissent l'organisation territoriale, vous avez notamment évoqué la loi nôtre c'est un texte que je connais bien, qui a été adopté à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat, à l'issue d'une commission mixte paritaire mais qui gagnera certainement à trouver quelques améliorations pour corriger ce qui peut apparaître parfois comme des irritants Sébastien le corps nu, mon collègue, ministre délégué aux collectivités territoriales, or en charge cette concertation dans les semaines qui viennent, pour pouvoir déboucher avant 2020 avant les élections municipales et ce de manière à donner de la visibilité aux élus, comme vous l'appelez de vos il il y a une 2ème concertation nous devons ouvrir : elle concerne la clarification de la répartition des compétences et la capacité des territoires, a bénéficié d'un principe de différenciation cela renvoie à la fois la révision constitutionnelle que le gouvernement a présenté et sur laquelle nous aurons à revenir, mais aussi à une discussion, territoire par territoire avec les collectivités, discussions qui sera menée par la ministre en charge des collectivités et la cohésion des territoires Jacqueline Gourault dans les mois qui viennent, enfin vous nous avez interrogé sur les relations financières entre l'État, les collectivités territoriales, permettez-moi de vous répondre en 2 points : d'abord pour rappeler que ce gouvernement maintient l'enveloppe globale des dotations aux collectivités et que celle-ci a même augmenté de 500 millions d'euros entre 2017 et 2019 que nous nous inscrivons dans une volonté de contractualisation de responsabilité aussi des collectivités et les chiffres de 2018, montrez nous avons fait un pari qui est réussi et enfin concernant la taxe d'habitation, nous aurons avec Sébastien le corps à rouvrir ainsi de négociations et de concertation avec les associations d'élus, de manière à ce que le projet de loi de finances pour 2020 apporte des réponses disent quel est le dispositif de compensation avec un objectif si madame la prison n'autorise tenir l'engagement du président de la République de donner des ressources stables pérenne et juste aux collectivités pour qu'elles puissent assurer leur politique et répondre aux besoins de leurs concitoyens. et seront retransmises sur Public Sénat, le site internet du Sénat et sur Facebook je vous je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 17 pour le débat sur le thème: quelle politique de lutte contre la pollution et le recyclage du plastique et plus généralement que l'utilisation du plastique en France, la séance est suspendue.

La séance s'est reprise, la parole est à monsieur Joël Bigot pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, merci Monsieur le Président, je souhaiterai procéder à de rectification de vote concernant le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité de la chasse sur les scrutins 80 et 81 Laurence Rossignol et André Vallini souhaitaient voter contre. L'acte et donner de votre mise au point, elle figurera dans l'analyse politique du scrutin, l'ordre du jour appelle la nomination des 27 membres de la mission d'information sur le thème : transport aérien et et aménagement du territoire, créé à l'initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, en application du droit de tirage prévu par l'article 6 bis du règlement en application de l'article 8 alinéa 3 11 et de l'article 110 de le règlement, la liste des candidats établie par les groupes a été publié, elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure, l'ordre du jour appelle le débat quelle politique de lutte contre la pollution et le recyclage du plastique et plus généralement que l'utilisation du plastique en France demande du groupe socialiste et républicain, nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents, je vous rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de 8 minutes, puis le gouvernement répond pour une durée équivalente, la parole et l'ont tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat madame Angèle prévisible pour le groupe socialiste et républicain et pour 8 minutes, vous avez la parole chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous remercie d'abord pour l'organisation de ce débat sur l'utilisation du plastique en France, longtemps nous avons cru que la Terre offrait un espace infini tellement nous sommes petits face à elle, longtemps nous avons cru que jeter de prêtait pas à conséquence et pourtant ce matériau fantastique et le plastique est devenue notre trouble-fête Le Chant du styrène vire au fiasco, l'air du gaspillage, a conduit à la gabegie d'un matériau qui se retrouvent aujourd'hui dans nos assiettes consommation effrénée et habitudes délétère consistant à jeter toujours plus après un usage éphémère, c'est le gobelet en plastique jeté après quelques gorgées ou la bouteille utilisée lors d'un unique repas le boomerang de notre surconsommation nous revient avec des conséquences catastrophiques, aujourd'hui nous sommes effarés de découvrir qu'un estomac de cachalot échoué peut contenir plus de 15 kilogrammes dont un filet de pêche de 13 mètres de long, scandalisé de voir le contenu d'une dépouille de cormorans à l'estomac rempli de déchets de toutes sortes, ému, enfin par cette tortue dont la carapace en forme de 8 semblait par un anneau de canettes, on recense des centaines d'espèces animales touchées par le phénomène d'enchevêtre ment et d'ingestion images terribles notre futilités face aux souffrances Ovi meurtri d'animaux innocents ou insouciance coupable aveuglement incompréhensible inconséquence condamnable, cette situation est le résultat de notre addiction à une certaine forme de faciliter le confort d'un hygiénisme exacerbé, face à cela, l'océan meurt et si nous ne faisons rien, il y aura en 2005 ans plus de plastique que de poissons dans les océans, comment en sommes-nous arrivés là, c'est après la Seconde Guerre mondiale, que le plastique se battaient Rio sous-produit du pétrole léger, peu coûteux, très stable malléable, s'impose comme le matériau idéal, il peut prendre toutes les formes car fabriqué par moulage il est robuste, coloré, il va peu à peu concurrencer les autres matériaux et finalement remplacé le verre, le métal, la porcelaine la céramique, le papier, le carton et le bois, apportant d'abord de réels progrès, créateur de richesses et d'emplois, son usage va se généraliser de nouveaux besoins vont être créés et la dérive consumériste va nous mener aux objets à usage unique au suremballage qui enfle nos poubelles dans un glissement progressif vers un comportement frisant le ridicule, s'il n'était dramatique et c'est l'indigestion, la France produit 5 millions de tonnes par an, et dans le monde, ce sont 10 tonnes par seconde qui sont produites depuis 1950 plus de 8 milliards de tonnes ont été produites, dont la moitié depuis l'an 2000 simplement au total seulement 9 pourcent ont été recyclés 12 pourcent incinérés tout le reste dans la nature sur cette quantité colossale, la moitié a fini dans les mers et les océans jusqu'au pôle, dans les îles les plus éloignées et jusqu'au fond des océanique n'a-t-on pas vu un sac plastique entier dans la fosse des Mariannes à 10000 mètres de profondeur dans le Pacifique Nord dans le même temps, les infrastructures pour recycler n'ont pas suivi la croissance de production, elle peine à se mettre en place et ne sont toujours pas dimensionné pour la quantité de plastique produites et jeté en France actuellement, à peine plus de 20 pourcent et recyclé la gestion non conduit à des déversements à ciel ouvert qui atteignent les Bastien aquifères et les plans d'eau, les courants marins ont provoqué, d'autre part, la formation de cinq GIR ou continents plastiques véritable soupe où flotte en moyenne 500000 fragments par kilomètre carré le plus important, celui du Pacifique Nord appelée 7ème continent couvre 7 millions de kilomètres carrés, l'équivalent du tiers de l'Europe ou de 6 fois la France notre mer Méditerranée n'est pas en reste et a le redoutable privilège de présenter en certains endroits, des concentrations en micro-plastiques quasi identique à celle du fameux continent plastique, notamment au large de Nice et de Cannes c'est choquant regrettable et tellement triste. Il est temps de préciser quelque chose d'important pour comprendre l'étendue du problème que nous avons à gérer le plastique n'est pas biodégradable et restera toujours du plastique dans la nature, la seule évolution qu'il va subir, c'est de se casser de se fragmenter en morceaux, de plus en plus petit, sous l'effet des rayons ultraviolets de la chaleur et des effets mécaniques et comme il y a des dizaines d'années qu'il y a des plastiques dans la nature il y en a maintenant de très petites particules microplastiques et même Nano plastique les plastiques sont des macro-molécule obtenue par polymérisation en accrochant les unes aux autres, par réaction chimique des petites molécules identiques appelé monomère dans leurs 3B création entre malheureusement aussi des additifs qui vont donner aux plastiques des propriétés particulières adaptées à leur utilisation anti-UV anti-statique retardateurs de flamme antichoc antimicrobiens et j'en passe, certains contiennent ainsi de véritables cocktails d'additifs, d'un point de vue sanitaire les problèmes viennent du relargage le relargage de ces additifs lors des fragmentations ou par la chaleur ou au contact des graisses dans la mesure où ces additifs sont des perturbateurs endocriniens qui affecte notamment la fertilité, le système nerveux le QI le QI cause des puberté précoce et sont classées cancérigènes, une étude récente sur l'eau embouteillée a révélé une contamination microplastiques dans 93 pourcent des bouteilles pour 11 marques testées les plastiques récoltés pour le recyclage sont fortement dégradés et nécessitent des opérations complexes de décontamination, ce que nous appelons Recyclage Plastique est en réalité d'abord du des cycles âge de plus une bouteille ne peut pas se recycler à l'infini, qu'en est-il des vêtements, produits à partir de matières recyclées, le tissu polaire vanté comme solution miracle de recyclage se révèle être une source de polluants lors de ses passages en machine à laver ou se détachent des fibres minuscule par abrasion et qui pollue l'eau chaque jour la station d'épuration de Nice on voit ainsi 6 milliards de fibres en mer au-delà des conséquences inévitables sur les habitats naturels sur l'économie, rappelons que les nanos plastique traverse les balles barrière tissulaire pour venir s'accumuler dans les organes, ce qui à terme perturbe leur fonctionnement c'est minuscule et invisible, fragments de plastiques contaminent de façon invasive toute la chaîne alimentaire, avec des effets sur la santé encore trop mal évalué, de plus, tous ces petits radeaux de plastiques qui flottent sont Connolly colonisé par des bactéries, des micro-organismes qui pourraient être pathogènes et, d'autre part, ces petits radeaux fixe également les polluants persistants, tels que les PCB, les fameux polychlorobiphényles, les dioxines qu'ils rencontrent sur leur chemin, puis qu'il transporte les enjeux sont immenses, la France n'est qu'au 28ème rang de l'Union européenne en matière de recyclage du plastique, et nous avons même repoussé à 2021, l'interdiction des pailles en plastique, le texte du projet de loi pour une économie circulaire et une meilleure gestion des déchets très attendu mais sa première version restent décevantes, il s'agit tout de même d'éviter une crise écologique et sanitaire sans précédent et prendre dès à présent, des mesures radicales d'interdiction de certains contenants d'emballage et de produits en plastique afin que les politiques publiques menées en faveur du recyclage ne soit pas un aveuglement collectif attention nous dès à présent à réduire de manière drastique, notre consommation plastique pour envisager le retrait du marché rendant réorientation du secteur, l'enjeu est de garder seulement les plastiques irremplaçable par exemple dans les hôpitaux et recyclés en circuit fermé, comme c'est le cas pour les bouteilles en polyéthylène Terry phtalates, le fameux P. E. T. ne tombons pas dans l'illusion du tout recyclage, nombre de pays ont plus d'une longueur d'avance sur nous comme le Costa Rica, qui a déjà interdit le plastique à usage unique, il est temps en France de mettre en place une véritable politique de lutte contre les plastique par une réduction à la source, qu'en s'attaquant donc au mal à la racine, à l'instar des avancées obtenues par la France lors de la COP 21 la France ne peut-elle pas impulser une initiative d'accord international pour lutter contre la pollution, plastique, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est en dame brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire pour 8 minutes également.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs. Alors, en guise de préambule j'envie vous propose un voyage dans le temps aux origines du classique. Il y a 1000 600 en Amérique du Sud, on a manipulé le 1er plastique. Du latex, produit à partir de la fève transformer du Chafia élastique à ou arbre à caoutchouc il servait à réaliser des balles ou des figurines, c'était en plastique qui était issu de matières premières non fossiles que les Amérindiens avaient appris à mêler Ali paumé blanche, une fleur pour produire in fine et la matière dont ils avaient besoin ces objets ont traversé les siècles sans devenir des déchets polluants. Pour une raison évidente, hé bien ils étaient issus de matières naturelles, née de la Terre, il pouvait mourir en terre. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça. Eh bien parce que chaque époque innove en fonction des avancées scientifiques, mais surtout de ses besoins ainsi les Amérindiens ont appris à produire du plastique pour répondre à la nécessité, qui était la leur à un moment précis, l'évolution des sociétés de leurs usages, l'augmentation de la population mondiale ont accompagné la montée en puissance de la production du plastique fossile est à l'origine, c'était pour le meilleur, pensons par exemple à la médecine et dont notre santé bénéficie encore aujourd'hui, à titre d'illustration, je pense, et je cite souvent l'intubation cette rupture technologique qui a était permise grâce à l'utilisation du plastique et qui a été une avancée majeure pour le monde médical, mais malheureusement. Par la force des outrances de la société de consommation, notre niveau de production de production de plastique dépasse l'entendement. En 2016, la production de plastique dans notre pays représente 120 kilos par Français et par an. Je trouve qu'il faut dire les choses clairement et je rejoins tout à fait la sénatrice près ville clairement, il ne s'agit plus uniquement de plastique utilisé pour sauver des vies, mais bien de surconsommation et de gaspillage, si nous avons aujourd'hui à merveille à extraire les hydrocarbures et nous continuons à investir massivement à l'échelle mondiale pour en extraire toujours plus, j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de m'exprimer très clairement sur cette question-là. Nous mettons nettement moins de temps et nettement moins de coeur au service de la fin de vie de ces produits transformés, résultat, c'est qu'à l'échelle mondiale, nous déversons l'équivalent d'un camion poubelle remplis de plastique chaque minute de chaque jour dans la mer. Anthony votre prolifération des plastiques est devenue insoutenable alors quel rôle pour l'État, quel rôle aussi pour la France. Quand on sait la petite taille de ce pays dans le monde, hé bien moi, je crois que nous avons un rôle très important à jouer, a commencé par être le plus exemplaire possible au niveau national et part continuer à mobiliser comme nous faisons elle fait encore plus activement au niveau européen et international. Dès le début de son mandat, le président de la République nous a fixé 2 objectifs très clairs : réduire de moitié la quantité de déchets mis en décharge et tendre vers 100 pourcent de plastique recyclé, d'ici 2025 pour nous ministres comme parlementaire, il est grand temps d'oeuvrer ensemble pour aller plus vite, plus fort contre la prolifération du plastique, c'est dans notre intérêt à tous car nos concitoyens ne cesse d'une commander d'agir le plus rapidement possible ces derniers mois, votre mobilisation, notamment sur le projet de loi pacte nous a permis de mettre en conformité le droit national et le droit européen, c'était crucial pour amplifier la première victoire que représente la directive sur la fin des produits à usage unique votée cette année appliquer d'ici janvier 2021, d'autant plus que la France a été en première ligne en première ligne pour rehausser l'ambition tout au long des négociations européennes. Cette mise en conformité, représente le 1er pilier de notre stratégie en 3 actes. lutter contre les plastiques inutile superflues, cela passe par l'interdiction de certains produits plastiques et en 1er lieu ce à usage unique, mais ça ne suffit pas, en parallèle, nous devons mener une réflexion collective et profonde sur nos usages, une question, par exemple, qui me semble centrale et sur laquelle nous pouvons, nous pourrons pardon revenir demeure quels sont nos meilleurs leviers à activer pour réduire rapidement drastiquement notre consommation, moi je pense qu'il faut transformer en profondeur le système de production et de consommation, ça pose une question d'organisation de notre système économique plus largement le débat d'aujourd'hui est l'occasion d'aller plus loin, j'attire votre attention sur un fait : comment continuer à supporter par exemple ce jour des incohérences je crois que nos concitoyens ne les supporte plus l'incohérence qui visent par exemple à commercialiser un brocoli bio en supermarché, mais totalement emballés dans du plastique, je suis convaincu que nous devrions encourager par exemple la vente en vrac pour cesser ces pratiques polluantes dévastatrices pour la planète est contraire au mode de vie, de consommation et au modèle économique que nous voulons promouvoir, nous y travaillons d'ailleurs activement, j'aurai l'occasion d'y revenir, et vous savez que nous présenterons d'ici à l'été une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui nous permettra aussi d'aller encore plus loin. Deuxièmement. 2ème, pilier de notre stratégie concernant le plastique dit utile. Ma conviction, c'est que nous devons mettre en oeuvre l'objectif qu'il soit 100 pourcent recyclé et cela dans les plus brefs délais, cet objectif est réaliste parce que nous sommes déjà sur le chemin d'une réduction de notre consommation inutile de plastique mais pour accélérer la cadence, il faut nous assurer que toutes les résines qui sont mises sur le marché soient recyclables que les filières industrielles soit mature que la collecte soit optimale et que la demande en plastique régénérer croissent, c'est donc toute une boucle, il faut mettre en place, c'est ce à quoi nous nous attachons et ce que nous faisons depuis les premiers mois de l'arrivée de mon arrivée en tout cas au gouvernement, dans le cas de l'élaboration de la feuille de route pour une économie circulaire 3ème, pilier. Nous avons besoin d'un boom de l'innovation, de la recherche et du développement dans ce secteur, nous devons stimuler le potentiel des solutions mécaniques biotechnologiques chimique car elles sont la clef de notre capacité à toujours mieux recycler, de même nous devons porter une attention toute particulière aux compétences Inès de la nature pour bio-dégrader préparé de la meilleure manière, l'air passe plastiques d'origine fossile, je suis convaincu, notre meilleur allié, il y a, c'est la nature elles-mêmes. Une stratégie victorieuse et toujours servi par une méthode pragmatique, concrète, qui vise des résultats pratiques dans les plus brefs délais, bien sûr, vous pourriez me dire que j'évoque des perspectives qui sont utopique. Pourtant, nos premiers résultats donnent de bonnes raisons, je crois, d'être optimiste pour ne prendre qu'un exemple, celui par exemple le de l'objectif de 100 pourcent de plastique recyclé, certes il n'est encore très loin d'être atteint, sur les 3,6 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année en France, nous nous recyclons que 300000. On est donc loin du compte, mais l'objectif que nous avons porté par le biais de la feuille de route de l'économie circulaire amis tous les acteurs de la chaîne de valeur sous une en tension, si je puis dire, une tension positive, résultat il y a quelques jours, les industriels du secteur se sont engagés à utiliser un 1000000 de tonnes de plastique recyclé, d'ici 2020, preuve que nous sommes aujourd'hui en capacité de déclencher un vrai changement d'échelle nous avons aussi mis en place une méthode pour aller vérifier la bonne mise en oeuvre de ses engagements, de façon à rendre les comptes et à ce que les acteurs travaillent de façon transparente. Par ailleurs, brutalisé notre appareil industriel en allant trop vite serait contre-productif. Il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale importante et là encore, une méthode qui me semble pertinent, c'est de nous donner, c'est de donner de la visibilité aux filières, c'est-à-dire un objectif de cours moyen ou long terme est très ambitieux et ensuite accompagné des acteurs dans leur adaptation, nous soutenons leurs investissements grâce à des dispositifs comme le programme des investissements d'avenir opéré par l'Adem nous action non parallèle des leviers incitatifs par exemple les bonus-malus mis en place pour l'éco- contribution des filières REP, nous mettons aussi en oeuvre de nouveaux dispositifs pour améliorer la collecte, l'appel à projets de collecte innovante et solidaire, qui a été financé par leur l'éco-organisme cité au en est un bel exemple

qu'une tonne de matières enfouies, il y a donc un enjeu aussi de développement des emplois locaux non délocalisables qui ont du sens partout sur notre territoire en stimulant les filières, grâce à des incitations et en imaginant une menace réglementaire crédible, hé bien nous transmettant un message clair aux acteurs ce qui ancre dans entrent dans la boucle de l'économie circulaire ont tout à y gagner, quant aux autres, le temps presse et la contrainte ira crescendo cette dynamique, vous le savez je l'occasion d'en parler, en introduction, hé bien elle a été engagé par la feuille de route de l'économie circulaire aux côtés du 1er ministre j'ai lancé cette feuille de route de l'économie circulaire pour installer cette méthode que je viens de tailler à laquelle nous croyons un an de consultations des parties prenantes ont mené à l'élaboration de 50 mesures, un an après l'engagement concret sur cette voie, le bilan est positif 95 pour 100 des mesures ont été enclenchées sont en train d'être mises en oeuvre, déjà j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, nous avons lancé un pacte classique, non pas sur les emballages plastiques qui réunit 13 entreprises qui sont moteur et qui veulent accélérer avant même la la loi sur l'économie circulaire qui va arriver, comme je le disais, d'ici à l'été, qui veulent accélérer la lutte contre le suremballage contre le plastique inutile et nous voulons aller et accompagner cette dynamique-là vraiment conclure, que je me réjouis aussi d'une chose pour conclure cette fois-ci, Monsieur le Président, vraiment c'est que lorsque les citoyens on participe au grand débat national, beaucoup d'entre eux ont fait beaucoup de contributions et je pense par exemple à la moitié de leurs 150000 contributions sur l'écologie qui faisait référence au mot déchets, d'autres encore ont beaucoup fait référence au mot plastique alors que ce n'était pas dans le cadrage initial du président de la République, c'est dire l'importance du sujet, c'est pour ça que je vous remercie encore mesdames et messieurs les sénateurs, d'avoir mis ce débat à l'ordre du jour, et je me réjouis d'avoir un échange de répondre à vos questions et je remercie Monsieur le Président pour sa patience. dans la suite du débat chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente 2 minutes je rappelle dans le cas où l'Otan dans la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à la condition expresse que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé et le 1er à intervenir sera Monsieur Guillaume Gontard pour le groupe CRC eux 2 minutes. Merci monsieur le Président, Madame la ministre, je ne reviendrai pas sur l'aberration écologique que représente l'usage du plastique, tant en termes de consommation de pétrole qu'en termes d'de d'émissions de gaz à effet de serre de production de déchets qui défigurent nos paysages et empoisonne nos océans ma collègue Angel prévu il a remarquablement démontrée et je la remercie, ainsi que le groupe socialiste d'avoir proposé ce débat en quelques décennies, les matières plastiques sont devenus tellement incontournable dans tous les domaines de notre existence, que son passé semble une tâche insurmontable, même quand il s'agit d'objets insignifiants à usage unique, comme les gobelets ou les pailles nous tergiverse, on est un débat récent ici est venue le rappeler et je ne parle même pas dans cette maison de la difficulté à supprimer, verres et bouteilles en plastique, le commerce national ne s'est pourtant pas effondrée avec interdiction des sacs plastiques en 2016, les industriels se sont adaptés, sans grande difficulté, heureusement que l'Union européenne nous force la main, avec une première interdiction d'objet plastique à usage unique, en 2021, il faut pourtant, elle est beaucoup plus loin, il est incompréhensible qu'en France nous recyclons qu'un qu'un qu'un petit quart des 5 millions de tonnes de plastique que nous produisons chaque année, nous sommes en deçà de la moyenne européenne, qui se situe autour de 30 pourcent très en deçà de l'Allemagne qui recycle, plus de 40 pourcent de son plastique notre société poussent l'aberration et vous l'avez d'ailleurs rappelé jusqu'à priver certains fruits de leur peau, leur emballage naturel pour les prix et les emballés dans du plastique, comble de l'absurdité, madame la ministre, vous êtes engagés pour améliorer le recyclage des bouteilles plastique et on vous invite à l'instar d'Istanbul de Sydney ou encore de Pékin, instaurer une consigne qui permet par exemple de payer des tickets de métro participe en participant au recyclage, mais cela reste largement insuffisant, la prochaine étape est une obligation à court terme de 100 pourcent d'emballages plastiques recyclés, cela passe par l'interdiction des matières plastiques non recyclables, ce qui contribuera également à simplifier les consignes de tri du plastique trop confuse, que comptez-vous mettre en place précisément pour favoriser notamment le commerce en vrac, est la seule alternative crédible du plastique et madame la ministre, votre gouvernement souscrite il à l'ensemble de ses objectifs, merci. Merci, Madame le Ministre. Merci monsieur le président, j'ai 2 minutes pour répondre. Oui, écoutez, je crois que ma question à Monsieur le président, Monsieur le Sénateur Gontard traduit combien j'aurais aimé avoir pour répondre à votre question, absolument essentiel et qui je crois est posée selon exactement les mêmes termes que le gouvernement s'est lui-même posé, si je puis dire, à lui-même pour lutter drastiquement contre la pollution, et je sais que nous avons eu l'occasion d'échanger sur cette question-là, alors, puisque je n'ai effectivement que 2 minutes 3 objectifs principaux : d'abord d'abord avant tout supprimer les plastiques inutile. Deuxièmement, et continuer et vous l'avez dit nous allons supprimer une bonne quantité de plastique à usage unique, mais continuons à regarder autour de nous ce qu'on peut supprimer, deuxièmement parce que ça finit souvent dans la nature, madame la sénatrice, ville d'ailleurs l'a bien souligné en introduction, deuxièmement quand c'est nécessaire, encouragé et pas, non pas encourager, mais faire en sorte que tous les objets plastiques au moins du quotidien, soit 100 pourcent en plastique recyclé, et pour ça, hé bien nous allons mettre en place un bonus malus par le avec des éco-modulation par le biais des éco-organismes de façon peu à peu en fait à éliminer les plastiques ne serait pas recyclables et à favoriser l'éco- conception autre mesure aussi, par exemple, nous réfléchissons, nous avons déjà lancé des appels à manifestation d'intérêt pour voir identifier comment nous pourrions et quelles seraient les meilleurs systèmes de collecte innovante et solidaire entre autres mendient pudiquement, en fait, ça veut dire des systèmes de consignes pour explorer, par exemple, des solutions comme lesquels comme celle que vous proposez, enfin ce que nous voulons aussi faire s'est considérablement développé, encouragé le réemploi.

bien, en signant avec 13 industriels du monde par exemple des supermarchés en signant avec un pacte national sur les emballages plastiques dans lequel il se fixe des objectifs très ambitieux de réduction drastique des matières plastiques, notamment pour lutter contre tous le sur-emballage et vérifier tous leurs engagements et la mise en oeuvre vérifié par des ONG telles que VVF ou encore Tara Expéditions, la Fondation Ellen MacArthur vérifier chaque année publiquement, et bien que c'est sans engagement sont bien mises en 9 concrètement parce qu'il est temps d'agir, vous l'avez souligné merci monsieur le sénateur. Merci, la parole est à monsieur Joël Bigot pour le groupe socialiste et républicain 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le débat que nous avons en ce moment, est d'une brûlante actualité alors que débute au siège de l'Unesco à Paris une semaine scientifique pour porter haut la protection de la biodiversité au niveau politique et enfin déboucher sur un protocole international dans lequel la lutte contre les déchets plastiques devra figurer en bonne place pour enrayer l'extinction massive des espèces, l'action diplomatique de la France depuis la COB 21 initiée par le précédent quinquennat est à la hauteur des enjeux, mais qu'en est-il de nos actions concrètes, notre taux de recyclage à fleurs, les 22 pourcent alors que la moyenne européenne est à 31 en outre, vous avez signé en février dernier, le pacte national sur les emballages plastiques qui invite les entreprises sur la base du volontariat à mettre en place des stratégies de gestion de déchets plastiques mais que faire pour les entreprises qui ne souhaite pas s'engager ou qui d'ores et déjà ne respectent pas l'obligation légale des 5 flux prévue par la loi pour la transition énergétique de 2015, nous attendons avec impatience la dernière mouture de votre projet de loi censée mettre en musique la feuille de route pour l'économie circulaire qui fête ce mois d'avril, sa première année, le 1er jet fut fort décevant et finalement très peu contraignant dans le domaine du plastique, enfin, un projet de consortium visant à mettre en place une consigne sur les bouteilles plastiques, ainsi que sur d'autres la emballage seraient à l'étude, sans que les collectivités locales soient consultés les collectivités représentent des acteurs incontournables de la gestion et de la prévention des déchets, il me paraît assez important de les ascensions des associés, pouvez-vous donc nous préciser la position du gouvernement sur ce projet, le consortium et sur les solutions retenues sur la question de la consigne pour les bouteilles plastiques principe sur lequel la dame n'est pas favorable, il y a un vrai risque pour les collectivités de déstabiliser toute la filière de collecte séparée sans même poser la question ô combien crucial de la réduction des déchets plastiques en amont. monsieur le sénateur merci là aussi de votre question alors plusieurs points : d'abord la feuille de route de l'économie circulaire représente un changement majeur je ne doute pas que vous avez suivi de près les discussions que vous avez participé aussi à l'élaboration de cette feuille de route que vous avez pu constater par vous-même, combien les collectivités locales étaient combien aussi les entreprises vont participer à l'élaboration de même que les associations et continuent d'ailleurs à enrichir l'élaboration ensuite du projet de loi vous savez aussi combien la France a été mobilisée au niveau européen, je suis donc étonné de votre remarque préliminaire j'ai eu l'occasion déjà de détailler dans ma réponse au au sénateur Gontard combien nous avons 3 priorités qui rythme et qui sont vraiment les 3 piliers de mise en oeuvre de la lutte contre la pollution plastique de la part du gouvernement, effectivement nous explorons de façon sérieuse et dans le détail, la possibilité de mettre une de mettre en place une consigne sur les emballages. Classique, mais aussi sur l'aluminium, comment est-ce que nous procédons, hé bien je vais vous dire les choses très simplement, au départ, quand nous avons évoqué cette idée-là, il y a eu une levée de boucliers de la part de beaucoup des parties prenantes. Les entreprises nous disaient que c'était impossible nos administrations, nous disait qu'en France, était totalement infaisable, puisqu'en France, où nous avions un système de filières REP qui était bien différent par exemple de l'Allemagne, c'était un système de consignes avec dont c'était donc infaisable et les collectivités locales. étaient très sceptiques à force de discussion, hé bien nous avons avancé sur la question de la consigne, je peux même vous dire une chose, c'est que les entreprises maintenant sont particulièrement moteurs sur cette question-là et figurez-vous que c'est l'État et en l'occurrence, moi qui, bien souvent, et qui est demandé aux entreprises de ne pas avancer trop vite de façon à garder dans la boucle, les collectivités locales parce que plus que jamais, il faut que les municipalités puissent conserver l'accès et puissent elles aussi bénéficier je dirais de la manne Man, c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas, puissent bénéficier, eux aussi, des matières plastiques qui constitue et qui doivent constituer un vrai gisement de valeurs pour les municipalités, mais donc, bien au contraire, un travail extrêmement étroits que nous menons avec les collectivités locales parce qu'il faut que chaque acteur de l'économie circulaire en ait pour son argent. Merci Monsieur Migaud 30 secondes de plus pour vous. Oui, donc j'ai bien entendu votre réponse, Madame la ministre et votre volonté de mettre en place une consigne pour le plastique, on a demandé aux collectivités locales de de faire des des structures de dimension importante de traiter, notamment à partir de 30000 des des capacités d'au minimum 30000 tonnes si on met en place des consignes plastique, on risque de déséquilibrer l'approvisionnement, et donc la ressource matière pour les collectivités locales, donc l'Adem s'est prononcé là-dessus d'ailleurs et se montre frileuse sur cette question, vous avez raison, il faut sans doute travailler ce sujet mais le rapport Vernier, faisait état d'une difficulté sur le les consignes plastique, par contre, ils sont très favorables au aux consignes Vert et puis le 2ème sujet c'est vouloir conclure oui les mais ce qui mettent sur le marché, qu'en est-il là aussi il y a une véritable responsabilité qui me semble-t-il, n'est pas prise en compte à la règle. Merci, la parole et comme je suis rigole pour le groupe RDSE pour 2 minutes, merci monsieur le président. Madame la ministre, mes chers collègues, d'après une étude publiée récemment 365 particules de microplastiques ont été retrouvés par mètre carré et par jour dans la station météorologique de Berne à 12 dans les Pyrénées cette station se situe en zone protégée Natura 2000 à 1500 mètres d'altitude et à plus de 5 kilomètres du village le plus proche, nous avons eu donc ici la preuve qu'en terme de pollution plastique aucun territoire n'est à l'abri, élu d'un département rural, le Puy-de-Dôme, connu pour ses grands espaces et son air pur, je m'inquiète naturellement des résultats de cette étude qui montrent des taux de pollution aux micro-plastiques comparables à ceux de Paris ou de Pékin favorisés par un certain nombre d'industries des micro-particules de plastique s'accumulent dans les sols et les cours d'eau et sont transportées par le vent, la pluie et la neige sur de très grandes distances dans l'océan Pacifique 94 pourcent des 2000 milliards de déchets en plastique sont des micro-particules. Même s'il ne représentent, de fait, qu'une petite partie de la masse totale de ce continent de plastique, ils sont les plus difficiles à traiter et s'intègre durablement dans notre écosystème. La question des macros déchets n'est que la partie visible du problème. Au-delà des conséquences sanitaires pour l'homme que nous connaissons mal pour l'instant, il existe des risques majeurs pour la biodiversité, alors que de nombreux scientifiques évoquent une probable sixième extinction de masse. Ces fragments ou microfilms sont utilisés à grande échelle dans l'industrie et notamment dans le secteur des cosmétiques et des fibres synthétiques, des voix s'élèvent aujourd'hui pour interdire l'utilisation des micro-particules notamment dans l'industrie cosmétique, ma question est donc la suivante quelle est la position du gouvernement sur ce sujet et comment comptez-vous inciter les industriels à préparer un changement dans leur mode de production, je vous remercie. Si 2 minutes Madame le Ministre. merci, monsieur le sénateur, mais si merci monsieur le président, excusez-moi, monsieur le sénateur Gold. Les microbes billes plastiques ajoutée intentionnellement dans certains produits, et vous l'avez cité par exemple les cosmétiques ou encore les détergents sont une source de pollution sur laquelle il est d'agir, d'autant qu'il existe des alternatives qui sont beaucoup plus réelle bien bien plus respectueuse de l'environnement avec la loi biodiversité qui date de 2016, la France a montré la voie en interdisant l'usage des micro-billes plastiques dans les cosmétiques, remplacés depuis 2018, j'ai passé cette mesure au niveau européen. Afin que celle-ci soit généralisée à tous les États-membres et ça, c'est un engagement de la feuille de route de l'économie circulaire qui, on le voit, a quand même eu un certain effet puis dont, en effet, très concret, puisque il vise et il a permis déjà d'interdire ces microbes plastiques à la suite de cette démarche, la Commission européenne a saisi les cas, l'Agence européenne des produits chimiques pour étudier la possibilité d'une restriction de mise sur le marché, sur la base de règlement Reach en janvier 2019, cette agence a préconisé une restriction de l'usage des microplastiques non seulement dans les cosmétiques, mais aussi dans les détergents, les fertilisants, les pesticides et je veillerai à ce que la commission se saisisse rapidement de cet avis et fasse une proposition législative. Enfin, j'ai demandé à la Commission en 2018, de prévoir des mesures pour récupérer les microplastiques issus du DRH des textiles en machine et toutes les options sont sur la pour déployer cette mesure, d'autre part, au niveau européen sur une base volontaire déjà nous travaillons avec différents pays, notamment les Pays-Bas à impact classique européen pour aller encore plus rapidement que la législation comme je vous ai dit que, sur laquelle la France est déjà très moteur d'autre part, nous avons fait de nos discussions sur l'environnement dans le cadre du G7, nous voulons des résultats très concrets, notamment en matière d'installation de filtres sur les machines à laver sur les stations d'épuration de façon à bloquer et empêcher que ces microplastiques qui viennent souvent de lavage de textiles synthétiques hé bien finissent dans l'environnement donc nous voyons, c'est une priorité pour le gouvernement et sur laquelle nous avons déjà commencé concrètement agir, nous avons déjà des résultats, il faut aller encore plus vite et plus loin. Si Madame la ministre, 30 secondes de plus si vous le souhaitez, Pierre collègues non alors la parole est à monsieur Claude pour le groupe Union centriste pour 2000. Oui, Monsieur le Président, Madame la ministre, le plastique offre une illustration parfaite de notre économie linéaire et aujourd'hui la France comme l'Europe accusent un retard important sur la collecte et le recyclage des plastiques, principalement parce qu'elles n'ont pas su entraîner l'ensemble des secteurs économiques dans une dynamique d'éco-conception et de recyclage si les récentes exigences en la matière, notamment européennes sont à saluer la France peine toujours à trouver son modèle et à mettre en place un dispositif cohérent, 6 mois après la publication de la feuille de route, les engagements pris sont globalement très décevant, en effet, l'ensemble des mesures actuellement en discussion en faveur du recyclage se concentre sur quelques annonces mais ces mesures ne s'attaquent pas à la question des différents plastiques qui ne sont pas recyclables née du partage de responsabilités et de coût entre l'amont et l'aval pour l'établissement de filières de recyclage pérennes afin de renforcer davantage la responsabilité d'émetteur sur le marché, il est nécessaire de créer l'environnement adéquat pour que soient gérés efficacement les flux entrants entraîner des flux sortant de qualité et contribuer ainsi à l'économie circulaire je pense urgemment à imposer un véritable plan de prévention et d'éco-conception aux entreprises avec des objectifs de réduction des déchets et de production de produits réutilisables ou recyclables l'intégration de matériaux recyclés dans tous les produits mis sur le marché en 2025, à mettre en place, nouvelles REP, tels que le sport n'est joué, le bricolage à contraindre fortement les produits non recyclables ou non valorisables énergétiquement en cohérence avec la réglementation, Madame la Ministre, comment comptez-vous aborder concrètement ces impératifs que je viens d'énumérer, car c'est bien de la mise en commun des synergies et des actions de toute la chaîne de valeur que dépend la réussite du défi de recyclage du plastique. Si Madame le ministre pour 2 minutes. Merci, merci, monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Kern vous avez raison, la France effectivement est en retard par rapport à certains voisins et je vais vous dire une chose, elle est tout simplement en retard par rapport à l'urgence et certains de vos collègues ont précédemment cités et mentionné la nature la biodiversité et je crois que les 2 sont intimement liés, je voudrais d'ailleurs. Les en remercier et souligne à quel point, donc il faut que nous accélérions et c'est ce que nous avons fait, c'est une priorité depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, les premiers résultats commencent à être palpables, avec plus 12 pourcent donc nous voyons, nous sommes sur une bonne trajectoire, c'était d'ailleurs là tout le rôle de l'État en de rassembler des acteurs qui n'aurait pas travailler ensemble et ne se serait pas échanger des matières si je puis dire, si nous n'avions pas enclencher cette dynamique, puis il faut aller encore plus loin, ça sera d'ailleurs et c'est tout l'objet de la loi qui va arriver d'ici à l'été et qui va comprendre en particulier des réformes importantes, notamment concernant le montant des éco-contributions qui est versée par les entreprises à des éco- organismes nous voulons notamment sur les classiques, elles augmentent de façon significative pour créer quelque part une incitation à mettre hors marché et à moins utiliser des emballages plastiques, c'est donc toute une économie toute une série d'incitations que nous voulons mettre en place tout au long de cette boucle parce que vous l'avez dit, il s'agit de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire c'est un effort qui est très significative, qui est donc demander à tous les acteurs, c'est un changement de méthode aussi profond et radical, mais je crois qu'il est urgent, il est urgent pour la nature pour la biodiversité, il est urgent, parce que les Français veulent des emplois sur les territoires non délocalisables qui ait du sens, il est urgent, aussi parce que c'est une façon pour les entreprises et pour beaucoup d'entre elles, elles ont partagé avec moi de regagner un Avantage compétitivité quand compétitifs et il est urgent, enfin, parce que nous devons avoir, et vivent dans une économie qui a du sens. Merci 30 secondes supplémentaires. Oui, Madame la Ministre, cette approche globale amont aval que nous avons abordé est capital en témoignent malheureusement le tristement célèbre 7ème continent plastique et les images choc qui y sont associés, toute notre énergie doit désormais être déployés pour lutter contre les plastiques à usage unique et je vous le dit sans ambages, Madame la Ministre, nous sommes particulièrement amer du vote de l'Assemblée nationale contre ce qu'avait décidé le Sénat sur les plastiques à usage unique, le jour même de la mobilisation mondiale en faveur du climat. Si la parole est à notre collègue Jérôme Bignon, pour le groupe des indépendants pour 2 minutes. Madame la ministre, le plastique prolifèrent à défaut d'être récupérées après usage recyclé, il est jeté dans la nature, il ne disparaît pas, se désagréger en petits morceaux, puis en fines particules, le vent et l'eau, le disperse et il affecte la planète dans toutes ses composantes, la biodiversité, sur laquelle se penche en ce moment, PBS en France est concernée, l'homme qui en étude des composantes est au 1er chef on ne dira jamais assez que le meilleur plastique et celui que l'on produit plus. Certains de ses usages ont récemment, et d'ailleurs, été interdit au niveau français et européen, c'est une bonne chose mais il faut continuer de recycler les plastiques utilisés, nos concitoyens sont plutôt efficace en France 75 pourcent dès son emballage plastique sont collectés collectés mais seulement malheureusement 26 pourcent sont recyclés, cela ne suffit pas, on voit néanmoins apparaître de nouvelles technologies la société française car bio vient ainsi à recycler la quasi totalité du plastique P. E. T. grâce à des enzymes bactériennes, certains pays ont développé l'usage et le tri du plastique bio-sourcées et compostable pour améliorer la valorisation de leurs déchets plastiques un problème fondamental demeure le plastique vierge coûte souvent moins cher que le plastique recyclé, madame la Ministre, premières questions, comptez-vous faire en sorte que le prix du plastique vierge reflète l'externalités négatives que comporte sa production et son utilisation pour notre planète, afin de favoriser l'usage du plastique recyclé 2ème question : le gouvernement envisage-t-il donc courage et la mise en place d'une filière de valorisation biodéchets consolidé par des évolutions réglementaires et fiscales rapide 3ème question : quelles mesures concrètes vont être prises par le gouvernement pour diminuer la pollution due au plastique dans les filières de traitements biodéchets je vous remercie. Merci, 3 questions en 2 minutes, Madame la Ministre, ou plutôt 3 réponses. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Bignon et mesdames, messieurs les sénateurs. Vous m'interrogez sur les mesures à mettre en 9 pour favoriser l'usage du plastique recyclé et sur les risques de pollution due au plastique dans les biodéchets alors j'ai parlé de la feuille de route de l'économie circulaire, j'ai parlé des différentes mesures que nous avions pris et mis en oeuvre, en plus de cette feuille de route et de la loi à venir. plusieurs points d'abord des engagements volontaires avec les filières industrielles et un pacte avec une partie des distributeurs qui vise l'incorporation de 1 1000000 de tonnes de plastique recyclé, contre 300000 aujourd'hui, pour le moment c'est volontaire, nous espérons et ça deviendra. Obligatoire de des bonus malus plus incitatif, qui vont être progressivement déployés sur les produits Plastiques en s'appuyant sur les éco-organismes pour responsabiliser financièrement les fabricants. Et on sait que ça fonctionne, il y a un bonus comme celui-ci qui a été mis et qui a été fixé en janvier dernier sur les films d'emballage en polyéthylène recyclé et ce n'est que le début, troisièmement, un taux minimum de plastique recyclé, qui pourrait être fixé sur certains produits, comme par exemple les bouteilles en plastique, quatrièmement, d'autres leviers nouveaux qui peuvent être mobilisés et à titre d'illustration, je veux parler du Label bas carbone qui récompense les externalités offerte par les activités réduisant l'impact de CO2 notamment les filières agricoles et forestières, il pourrait être étendue au secteur du recyclage concernant aussi le risque de pollution classique dans les biodéchets pour ceux qui restent, jeter la loi a prévu qu'il respecte une nombre de compostage domestique plus exigeante que celle appliquée par certains de nos voisins, si celles-ci s'avèrent insuffisantes ces exigences seront renforcés, enfin j'ai missionné monsieur Alain Marois pour élaborer un pacte de confiance visant à renforcer les exigences de qualité des matière fertilisante issus des biodéchets notamment sur les Indiens désirable comme par exemple le le plastique fort merci. 30 secondes supplémentaires chers collègues. locales afin qu'elles puissent s'équiper au plus vite dans leur centre de tri d'équipements innovants permettant de mieux répondre aux questions de pollution par les plastiques, je pense que là aussi ça passe évidemment par une mobilisation citoyenne, ça passe par de la science, mais ça passe aussi par un appui aux collectivités qui ont besoin de de ne pas avoir une charge supplémentaire dans leur dans l'exploitation de leur de de leur territoire, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Jean-Marc Boyer pour le groupe, les républicains 2000. Président, madame la ministre, l'impact émotionnel est fort quand nous voyons les images des bouteilles en plastique flottant sur les mers mais ne cédons pas au plastique bashing, radical, sans savoir pourquoi et comment afin de savoir pourquoi il est nécessaire de recueillir l'ensemble des données qui conduisent à la pollution du plastique, des éléments sur sa production et son recyclage en France et dans le monde afin de savoir comment il est fondamental de dresser un état des lieux des dangers avérés ou non du plastique sur la santé, il est aussi essentiel de faire le point sur la recherche fondamentale et les solutions innovantes afin de permettre une alternative de remplacement adaptées aux réalités bien sûr nous sommes parfaitement conscients de l'urgence à trouver des solutions de substitution en plastique mais ne cédons pas à une application précipitée du principe de précaution, car les enjeux sont d'ampleur autour de la production du plastique, c'est un secteur économique et des milliers d'emplois qui sont ici concernés, notamment dans le domaine de l'embouteillage concernant les solutions innovantes du recyclage, une première mondiale, une première mondiale, issu d'une société Puy-de-Dôme car Biosse mon collègue a cité tout à l'heure, produit des premières bouteilles en plastique 100 pourcent bio recyclé, fabriqué à 100 pourcent à partir de déchets plastiques cette innovation est porteuse avec les 6,3 milliards de tonnes de déchets plastiques que l'on retrouve dans les décharges et les océans ou Dandenault unités de recyclage française aussi, Madame la ministre, ma question est la suivante : quels moyens techniques et surtout financiers, l'État compte-t-il engager afin de soutenir les solutions innovantes pour permettre une transition écologique efficiente en tenant compte des réalités de production des contenants plastiques et des réalités économiques. Merci madame la ministre, il ne s'agit pas là. Quelque part, de jeter le bébé avec l'eau du bain mon ministère s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire, et nous savons donc des changements brutaux radicaux, je crois que nous en avons fait l'expérience hé bien nuisent à l'acceptabilité sociale des politiques publiques environnementales, or nous visons l'efficacité, il faut donc trouver cet équilibre entre avancer le plus vite possible et ne laisser personne. Au bord de la route, hé bien c'est tout l'objectif des politiques publiques que nous menons au sein de ce gouvernement là, elle concerne aussi le plastique, vous avez vu, je l'ai dit réaffirmé partager avec certains de vos collègues ici, notre objectif c'était entrer tablent sur la pollution plastique d'enclencher aussi une vraie révolution avec un changement de modèle économique vers une économie qui soit circulaire mais pour ça, hé bien il faut s'assurer que nous ne laissons personne sur le bord du chemin et donc à l'heure où je vous parle, hé bien je mène des discussions avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail pour développer accélérer l'apprentissage, la formation, de façon permettre aux employées qui travailleraient pour des usines qui viendraient seraient peut-être amenés sinon à fermer en tout cas à se transformer, il faut les accompagner, il y a aussi d'autres agences de l'État, le fait que, par exemple, la dame qui travaille, qui déploie le pays à ce programme d'investissements d'avenir pour travailler aux côtés des collectivités avec les entreprises à l'émergence de solutions alternatives, encore une fois, ne nous voilons pas la face, c'est bien dans le recyclage que se situent les employes, je l'ai dit : pour une tonne qui n'est pas enfoui, hé bien ces 10 enfants 10 emplois supplémentaires en plus, c'est donc ensemble que nous vous devons travailler aux solutions, c'est tout l'objectif de cette feuille de route de l'économie circulaire c'est tout l'objectif et toute la méthode du gouvernement auquel j'appartiens. Merci, merci, 30 secondes de plus non, alors la parole est à monsieur Frédéric Marchand pour le groupe, la République en marche pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, nous savons qu'ils sont très difficile, voire illusoire de pouvoir se passer complètement du plastique est une matière face à peu coûteuses inerte biologiquement et résistante sur le plan mécanique, en effet, le plastique est utilisé dans les transports, dans le bâtiment, dans l'électronique dans la santé, dans quasiment bon nombre de domaines de la vie quotidienne : le plastique, ça a été dit, c'est fantastique, mais c'est surtout catastrophique quand il n'est pas recyclé or s'il est bien trier bien collecter, il peut être recyclé et peut ainsi connaître une 2ème voire une 3ème vie pour parvenir à l'objectif de 100 pourcent de déchets plastiques recyclés, une des mesures proposée dans la feuille de route visant à inciter les industriels à entrer dans la boucle en incorporant davantage de matières premières issues du recyclage dans les produits, tout en assurant leur qualité et leur traçabilité une réelle sécurité pour nos concitoyens ainsi d'ici 7 ans, il y aura 2 fois plus de matières premières issues du recyclage dans nos produits du quotidien, mais cela reste largement insuffisant, au-delà, l'engagement des industriels pour augmenter le taux de recyclage du plastique, il semble qu'il faille améliorer sa collecte en modernisant les infrastructures et mieux informer le consommateur des gestes correct à adopter afin qu'ils puissent mieux différencier les plastiques, le papier, les métaux puisque chaque effort de tri est bénéfique pour toutes les filières et initie un cercle vertueux, une solution déjà existantes et facilement exportable dans le monde pour lutter contre la pollution due au plastique et d'inciter au développement des bio-plastiques biodégradables et compostables on en produit en France actuellement, 2 millions de tonnes par an, soit 1 pourcent du marché des emballages plastiques, l'émergence de ces bio-plastiques dits de nouvelle génération permet la valorisation des biodéchets qui peuvent contenir et qui créent aujourd'hui des émissions de CO2 ces biodéchets qui sont actuellement enfouis ou incinérés pourrait être valorisé, notamment par compostage les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduel des Français c'est un gisement non négligeable qu'il faut maintenant dite tournée de l'élimination en vue d'une économie circulaire de la matière organique pourra train de l'objectif de 100 pourcent des plastiques collecté, recyclé avant 2007, pouvez nous donc nous indiquer quelles mesures seront mises en oeuvre pour rendre la collecte plus efficace et pour moderniser nos centres de tri en France et ainsi améliorer la valorisation de nos déchets, merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, merci, monsieur le président, Monsieur le mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le CDH, le sénateur. Frédéric Marchand d'abord permettez-moi tout d'abord en introduction de vous remercier encore pour votre aide, soutien contribution sans faille et sans aucune d'ailleurs concession à nos travaux sur la feuille de route de l'économie circulaire et je sais que vous serez encore à nos côtés pour nous stimuler et encourager les innovations

je voudrais dire, et préciser une chose, c'est que le terme biodégradable génère des confusions dans l'esprit des Français, il laisse penser que ces places, il se dégraderont dans la nature, ils peuvent être abandonnés dans l'environnement, or c'est tout le contraire, en réalité, ces plastiques dits biodégradables ne se dégradent que dans un environnement contrôlé l'oxygène par exemple ou à bonne température soit un site industriel spécialisé soit dans un composteur domestique bien gérée pour quelques produits très fins, telles que les sacs en plastique et donc nous voulons faire en sorte que le remède ne soit pas pire que le mal, et c'est pourquoi, hé bien plusieurs informations seront indiqués sur certains produits en plastique, comme par exemple l'éviter que certains fabricants trompe les Français ou encore les amener à mieux indiqué le geste de tri associés à chaque produit grâce à un message clair et spécifique, c'est l'objet d'une des mesures du projet de loi anti-gaspillage que nous préparons et vous avez aussi évoqué la question absolument essentielle de l'accompagnement des collectivités locales, Très régulièrement vous partager les préoccupations des collectivités locales sur votre territoire et, plus largement, je l'ai dit, il va y avoir et nous allons continuer la mobilisation dans le cadre du pays a avec différentes agences de l'État, nous voulons aussi mettre à contribution si je puis dire de façon plus efficace les éco-organismes avec des objectifs de performance Claire mesurables et qui doivent être relayées de façon transparente, ça fait partie des quelques pistes, il y en a d'autres, nous aurons à nouveau l'occasion d'échanger je vous remercions. Merci madame la ministre, pas de temps supplémentaire, la parole est à monsieur Bernard Jomier pour le groupe socialiste et républicain. Merci monsieur le Président, Madame la ministre, à ce stade du débat, je voudrais faire une remarque préliminaire, c'est ce que j'ai, j'ai le sentiment comme souvent malheureusement en matière d'écologie que dans notre pays, on est très fort pour poser des objectifs à 2030 2040 2050, puis on les pose de plus en plus fort, mais quand il s'agit de 1000 19 août 2020 on avance très lentement en fait, on fait des sauts de puce, et c'est pas, c'est pas des sauts de puce, enfin, on peut faire 10 autres puce ça voudra jamais à un bond de kangourou, or vous avez employé vous-même l'expression d'urgence en la matière, il y a urgence, d'autres pays ont des ont pris des mesures très fortes, et voilà et ce ce, ce grand écart écologique il me préoccupe mais je revenir à ma question, elle porte sur la santé, conserves contiennent un certain nombre de de substances, notamment les plus connus sont les phtalates, le bisphénol ou le très Occident Team One, qui est présent dans le poète qui sont, qui ont des conséquences graves pour la santé humaine, ils peuvent être cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, or l'évaluation et la recherche ont considérablement fait progresser la connaissance en matière mais les décisions derrière suivent difficilement clairement, c'est la question de notre gouvernance de notre tous mode de décision en santé environnementale qui est interrogé, même quand une substance est identifié comme étant toxiques, nous avons beaucoup de mal à avoir un process partager et clairement identifié de retrait de la substance, pour des raisons sanitaires, y compris en en émettant des priorités en la matière parce qu'on ne peut pas tourtereaux retire du jour au lendemain, j'en suis bien d'accord, donc cette question-là, c'est la gouvernance en santé environnementale est essentielle, elle est mal organisée dans notre pays, comptez-vous travailler sur cette question et faire des propositions en la matière pour modifier notre gouvernance en santé environnementale chômeurs. Merci madame la ministre. Merci, merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénat. Thor Jomier alors plusieurs choses dans votre question, d'abord, vous parlez de sauts de puces et de sauts de kangourou, moi j'ai l'honneur de vous dire que peut-être, je me suis transformant en kangourou, depuis, j'ai été nommé au gouvernement, mais en tout cas, j'estime que j'ai fait quelques sauts de kangourou, alors ils seront jamais suffisants les sauts de kangourou, ça je vous l'accorde, étant donné l'urgence. Je le regrette et tous les jours, j'essaie d'y remédier, avec tous mes collègues au sein du gouvernement et on y remédie aussi parfois à bas bruit, c'est-à-dire au niveau européen, au niveau international, on est d'ailleurs parfois critiqué pour faire beaucoup de bruit, soi-disant au niveau international, or c'est là aussi beaucoup que se trouvent les solutions et en matière, santé, environnement, c'est le cas, c'est le cas. C'est pour ça que la France se bat et nous avons adressé plusieurs courriers en ce sens à la Commission européenne, par exemple, puisque vous parlez de substances sur la question des perturbateurs endocriniens, nous avons lancé la une 2ème stratégie en France mais nous devons poursuivre ce combat au niveau européen, notamment pour avoir une stratégie qui soit transversales qui sont aussi prises en question en en comptant les questions sur l'dans les cosmétiques, dans les jouets, par exemple, ça, ça fait partie de nos objectifs, premièrement, deuxièmement mais ça c'est un un énorme travail de conviction nos autres pays ce pays européens et, deuxièmement, vous avez parlé de gouvernance et pour prendre des mesures, souvent, il nous faut des preuves et les preuves qui soit efficace qui soit scientifique pour cela nous avons réformé et nous avons mené un combat là encore à bas bruit, mais je me suis rendu avec la ministre de l'Europe de l'école Nathalie Loiseau dans les différentes agences cas élève ça que vous devez bien connaître si vous interrogez d'intéresser à ces questions-là, monsieur le sénateur, de façon à rendre à transformer de façon profonde, leur système d'évaluation des substances chimiques et qu'elles soient beaucoup plus indépendant des industriels pour que nous ayons une vraie science à portée de main, indépendante indépendante des entreprises qui guident nos décisions, nous voulons aller là aussi encore plus loin et c'est un combat qui se situe et qui se portent en grande partie au niveau européen mais nous menons aussi au niveau français, preuve en est, vu ce que vous parlez substance du glyphosate. Nous allons sortir d'ici 3 ans en Europe ces 5 sans la France aurait été encore 15 ans d'autorisation au niveau européen et là je crois qu'il faut le rappeler, aussi, d'autre part, d'autre part, il me reste un peu, moi je vais, je vais le prend, si vous m'autorisez pas, Monsieur le Président, mais simplement pour vous dire aussi que nous faisons quand même un certain nombre de, de, de sauts de kangourou notamment plus 12 pourcent d'utilisation de plastique recyclé,

30 secondes de plus Monsieur Jomier. Je remercie Monsieur apprenez donc moi je souscris à votre analyse sur les instances européennes sur la situation, mais il y a notre propre responsabilité en France, le ministère de la santé, c'est le ministère du soin et ça reste le ministère du soin, il n'y a pas d'Direction de santé environnementale, il y a une part qui auront une direction générale de soins Lens vous parliez de la présence des industriels qui posait problème, regardez la composition du conseil d'administration de Lens, regardez comment sont répartis les responsabilités actuellement entre les différentes agences relativement chaotique explique et vous allez pas me dire que cet adulte actifs et et déplacé, on sait relativement chaotique et donc il faut revoir cette gouvernance. Merci, la parole est terminée, Françoise Férat pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, beaucoup de constats et de positions que je partage, ont déjà été évoqués ce soir ce débat fait écho à la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la lutte contre les déchets en plastique déposé le 8 octobre dernier par ma collègue Nathalie Goulet que j'avais d'ailleurs cosigné mais je vais aborder 2 points importants qui doivent être pris en compte dans ce débat primordial pour l'environnement le 1er est l'acceptabilité par les consommateurs, il est demandé aux industriels de diminuer le volume des emballages plastiques de réduire leur poids et de stopper les objets à usage unique, mais le consommateur a un pouvoir des industriels ont testé auprès des consommateurs, la réduction du poids de la bouteille de soda et d'eau, certains ont renoncé car le client trouver le produit trop cheap, c'est-à-dire pas Guillaume comme pour beaucoup de mesures environnementales, il pointe aussi les dégâts écologiques en Asie par exemple ou des vidéos de rivières de déchets plastiques et des maires de bouteilles de sachets circule sur Internet, on ne retrouve heureusement pas désastre en Europe, il faut ainsi que le consommateur change ses habitudes d'achats et se tournent vers des objets réutilisables accepte de voir ces produits favoris évoluer dans la conception de leurs contenant se détournent du plastique pour les objets à usage unique, des solutions existent déjà, mais comment les inciter à faire plus, le second point à développer et à soutenir et la substitution du pétrole par des biomatériaux algues plante amidon, l'utilisation des déchets végétaux est un formidable levier de transition énergétique et de développement économique, rappelons aussi que la plante dans son processus de photos ça c'est synthèse captent du carbone, couplée à une réduction des volumes de production du plastique, les agriculteurs et la bioéconomie sont des acteurs importants pour sortir du plastique issu du pétrole par le remplacement des biomatériaux, certains estiment que près de 70 pourcent des familles de polymères sont susceptibles d'être bio-sourcées, qu'en est-il, madame la ministre, je vous remercie. Merci madame la ministre, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, fait rare. Alors vous parlez du rôle clé des consommateurs qui pourrait, qui sont parfois appelés consom'acteur sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, alors je suis d'accord avec vous sur le fait que les consommateurs ont beaucoup de pouvoir, maintenant, je pense, ils ont beaucoup de pouvoir, par leur choix maintenant, je pense, et pour avoir échangé par exemple avec des jeunes, des étudiants, beaucoup m'ont dit souvent : nous n'avons pas envie d'attente que les entreprises nous propose de meilleurs produits, nous pouvons et nous voulons nous-mêmes agir mais ils doivent nous donner les moyens d'agir, et moi je considère aussi que cette eau, c'est à l'État de donner aux citoyens les moyens d'agir et pas uniquement d'essayer de faire sans cesse reposées les changements sur l'innovation, la créativité, la volonté de changer du consommateur, je crois qu'il faut un mouvement qui aille dans tous les sens, il faut autant de dynamique du consommateur que de moyens qui sont donnés par l'État par les entreprises aux consommateurs sur cette suite à cette introduction un peu longue, je voulais vous dire que nous avions déjà commencé à agir concrètement, là aussi, c'est et, et que certains consommateurs ne veulent pas de produits qui soient mieux et et souvent mieux éco-conçu, parce qu'il n'en n'aime pas la qualité, moi je dois vous dire aussi que souvent quand j'échange avec beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'elle me dise au départ et en réalité finalement quand elles testent les nouveaux produits, elles s'aperçoivent qu'il y a beaucoup plus d'acceptabilité de la part des consommateurs que ce qu'elle croyait elles-mêmes. Et c'est ça aussi sur la lutte contre les invendus et le gaspillage beaucoup beaucoup plus. Et donc je crois qu'elles peuvent donc faire plus et d'ailleurs, elles savent qu'elles peuvent faire plus, puisque il y 13 entreprises ont signé ce pacte national sur les emballages plastiques, il y a quelques semaines au ministère de la transition écologique et solidaire avec des objectifs très ambitieux et surtout qui sont mises en oeuvre dès dès aujourd'hui avec des changements parfois drastiques des habitudes et des rues, des repères même des consommateurs par exemple changer la couleur d'un plastique l'épaisseur d'un plastique et finalement les consommateurs et bien ça leur convient et ils font ils franchissent le pas et notamment enfin en ce qui concerne les plastiques bio-sourcées, hé bien c'est une il faut les encourager, moi je voudrais simplement dire une chose : il ne faut pas que le dépasse le le développement de plastique bio-sourcées et de l'autre côté des conséquences négatives pour la biodiversité et pour la nature. Merci, la parole est à monsieur Patrick chaise pour le groupe, les républicains pour 2 minutes. C'est le président Madame la ministre, mes chers collègues, derrière le mot plastique, il y a différentes réalités car différentes résines plastiques et certaines sont plus recyclables que d'autres. Au-delà de la recycle étiez il y a de la réalité que sont les filières de recyclage existe-t-elle des différents plastiques le P. E. T. polyéthylène Terry phtalates 100 pourcent recyclable et puis recommandés pour les usages alimentaires et les boissons, il permet un usage vertueux du plastique lorsqu'il s'inscrit dans une économie circulaire. C'est le deuxième emballage le plus recyclé en France après le Vert, des progrès ont en effet été fait depuis 10 ans et des engagements ont été pris par les embouteilleurs de boissons pour réintégrer une partie croissante de ce plastique recyclé dans les bouteilles, ce qui nous permet d'être optimiste pour être en phase avec les objectifs d'incorporation de la directive européenne à venir imposant 25 pourcent de plastique recyclé dans les bouteilles P. E. T. de boissons d'ici 2025 afin d'assurer. La disponibilité de plastique recyclé compétitifs sur le territoire français, en quantité et qualité souhaité, il est nécessaire de progresser sur la collecte des plastiques post-consommation pour recyclage, les citoyens ont pour une grande partie d'entre eux, la chance de profiter d'un système de collecte sélective à domicile un véritable service au profit du recyclage pour parler de pérenniser ce système français il faut doper nos performances de collecte en s'inspirant de certains pays voisins, comme la Suisse ou la Belgique, plus performant que nous, en ce domaine par la mise à disposition obligatoire de poubelles de tri multi-flux sur la base de ces éléments, pouvez-vous nous éclairer sur la politique que votre gouvernement entend mener afin de limiter le plastique bashing qui est à la fois et réaliste est insupportable.

là aussi absolument essentielle puisqu'il s'agit de mettre en place une vraie filière industrielle 10. Politique industrielle en faveur du recyclage et c'est exactement ce que nous avons Mail, nous voulons mettre en oeuvre, je travaille notamment là-dessus avec le ministère de l'Économie et des Finances, parce qu'il s'agit là et nous devons développer avec les moyens nécessaires, une véritable politique industrielle je partage beaucoup de votre constat, je crois que pour que cette économie circulaire autour du place puisse se développer, il faudrait déjà que nous ayons réussi à collecter en nombre suffisant, la matière initiale, c'est-à-dire le plastique à recycler et c'est pour ça que nous n'avons pas attendu la loi, nous avons des récemment mis en place et nous sommes en train d'explorer différentes solutions d'afin d'identifier la meilleure pour développer et considérablement augmenter l'efficacité d'un système de collecte qui en France a été conçu pour être relativement efficace il y a quelques dizaines d'années aujourd'hui, maintenant il faut passer un cran supérieur et c'est tout l'enjeu, c'est donc une vraie révolution qui est et qui va s'avérer probablement compliqué néanmoins nécessaire, je parlais tout à l'heure par exemple de la consigne pour plastique et aluminium, hé bien c'est ce que nous cherchons à mettre en place actuellement, il y a 20 projets qui vont être déployés sur le territoire de projets innovants développés avec l'Adem et avait cité au pour voir quelles seraient les meilleurs moyens de collecter c'est plastique là. De façon à créer une vraie filière de recyclage, il y a aussi la question de la compétitivité entre pris entre la matière brute et la matière recyclée, on sait qu'il y y a trop de fluctuations, ce qui fait que bien souvent les industriels continuent à utiliser du plastique vierge, c'est-à-dire directement fossiles, hé bien nous voulons utiliser les éco-modulation pour lisser ces variations du baril et du coût du pétrole qui ont des conséquences négatives sur l'utilisation de matières et la commercialisation de matières plastiques plastiques recyclés, de façon à ce qu'elle reste toujours au moins on sait compétitif, si ce n'est plus que le plastique vierge, voilà donc les différentes solutions, je sais aussi, monsieur le sénateur que hé bien il y a une vraie tradition une vraie expertise des vrais champions de l'économie Placid, j'ai eu l'occasion de m'y rendre dernièrement avec le ministre de l'éducation monsieur Jean Michel Blanc. Car pour observer et voir tous les projets qui avaient au coeur de ces territoires très riche, j'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous de me rendent là-bas pour qu'ensemble nous développions des solutions pour garder cet Avantage, tout en faisant en sorte qu'il soit le plus adapté possible à l'économie du XXIe siècle. Je vous remercie, monsieur je sais, Madame la Ministre, juste pour vous dire que bien sûr la invitation, vous l'avez. ça sera avec grand plaisir et que je crois effectivement qu'il faut arrêter d'avoir une vision globale sur le plastique et de généraliser le plastique, le plastique a aussi apporté service à sa vertu et je crois qu'il faut aussi pouvoir le dire. La parole est à monsieur Roland Courteau pour le groupe socialiste. Merci monsieur le président, oui j'ai noté Madame la ministre d'ici même, alors que j'évoquais l'État de la Méditerranée, face aux pollutions, madame la secrétaire d'État Madame Hoarau a bien précisé que sur la base de mon rapport Opecst et de l'alerte que j'ai lancé le 1er ministre avait demandé, comme plein de réduction de l'apport de macro-déchets microplastiques à la mer serait mise en place d'ici 2020, je suis donc preneur de toute précision, le mal est mondiale, tout le monde l'a, l'a dit et répété chaque seconde de plus de 200 kilos de plastique aboutissent dans les océans, résultat les résidus plastiques sont partout dans les organismes, les espèces marines et jusque dans la chaîne alimentaire, comme on l'a précisé d'ailleurs un gel prévisible a Méditerranée par exemple le nombre de micro-déchets plastiques varie de 5000 à 900000 par kilomètre carré et d'certaines ozone on compte autant de micro-déchets que de plaintes ont ils sont partout, et pas que dans les mers jusqu'à nous sommes maîtres d'altitude dans les Pyrénées ariégeoises, quel est le coût des dommages environnementaux et quel va être le coût sanitaire saluons donc la la volonté de la France et de l'Union européenne, de sortir de notre culture, du tout jetable avec l'interdiction d'une dizaine de produits plastiques à usage unique, mais l'essentiel étant de réduire la production et la consommation à la source tout en favorisant le déploiement des alternatives au plastique, mais l'important, c'est aussi la collecte et c'est aussi le recyclage et l'incinération et là nos marges d'erreur non moi je de progrès sont énormes, toutefois attention, on ne peut pas recycler indéfiniment les plastique donc comment entendez-vous promouvoir le déploiement des alternatives au plastique, où en est-on de l'application du principe pollueur c'est-à-dire de la prise en charge des frais de nettoyage de collecte de ces déchets plastique par les fabricants et enfin comme il faut une régulation mondiale, sous quels délais un traité mondial sur la réduction de la production. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Courteau tout d'abord, permettez-moi de vous me joindre à à à mes collègues du gouvernement mise état et et la secrétaire d'État pour vous remercier pour votre travail et pour votre implication sur ces sujets-là, en particulier sur la pollution de la mer Méditerranée, je sais que ça vous tient beaucoup à coeur que vous nous avez proposé des solutions pragmatiques et concrètes, alors la France a fait de la lutte contre la pollution plastique dans les océans, dans la mer, une vraie priorité une priorité, puisque vous l'avez souligné, c'est une question éminemment internationales, européennes et internationales, et bien nous avons donc décidé d'en faire. La lutte contre la pollution classique un point et un axe important du G7 à Biarritz et nous en voulons construire une coalition autour de la lutte contre la pollution plastique en réunissant au moins 20 à 25 pourcent des acteurs et des des parties prenantes à l'échelle mondiale en matière de lutte contre le plastique de façon à faire 2 choses, c'est à faire en sorte que à envoyer un signal aux 75 pourcent, qu'ils n'auront pas joints cette coalition-là, de lutte contre la pollution, plastique et bien que s'ils ne le font pas, et nous pouvons les points. C'est du doigt et de façon envoyer aussi un message aux États qu'il est temps de réguler et d'aller plus loin et vous parlez par exemple de traiter différentes solutions peuvent être explorés, d'autre part, la France tient à prendre ses responsabilités et à être en fer de lance, sur la question, c'est pourquoi nous allons accueillir le congrès mondial de l'hiver. à Marseille le congrès de la nature qui va faire là encore de la lutte contre la pollution classique, un objet central des discussions et qui vise à préparer la COP 15 de la biodiversité qui va avoir lieu en Chine et qui est aussi importante que ce que la COB 21 a pu être et nous voulons et nous tenons à ce que la lutte on des plastiques, ils tiennent une place importante, enfin en France, il y a eu le pacte national contre les emballages plastiques qui vise encore une fois, à lutter contre la pollution plastique sur le sur le, Parce qu'une fois que les plastiques sont dans les océans, dans les mers, c'est trop tard, c'est donc notre système de production et de consommation que nous avons changé en amont. Nous ne pourrons pas nettoyé tous les océans, malheureusement, il est donc conclu leur de faire un changement radical important, je vous remercie de votre. C'est-à-dire sur la

pour cette mère une véritable bombe à retardement pour la faune, la flore et la santé humaine, mais je m'interroge gravement sur les risques de polymérisation de cette mère qui est toute petite équipe quasi fermés et qui est fragile et la réponse à ces études dans la mobilisation des 21 États riverains autour de la Méditerranée, et là il faut un leader qui aime plus de nouvelles actions et je compte je la France madame la Ministre. Monsieur Pierre Cuypers, quand le groupe les républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le Président, Madame la ministre : notre maison brûle et nous regardons ailleurs : nous sommes tous responsables, ces mots prononcés par le président Jacques Chirac en 2002 au sommet de Johannesburg gardent toute leur acuité et reste brûlant d'actualité la lutte contre les déchets plastiques doit devenir impérativement une priorité pour l'Europe, la pollution par les plastiques sur terre ou dans les mers doit être réduite, le plus tôt possible, chacun d'entre nous, en convient or madame la ministre, à ce jour, vous le savez bien, seuls 26 pourcent des emballages plastique sont recyclés. De nombreux plastiques recyclables ne sont dans les faits, pas en raison de contraintes techniques ou économiques, c'est par exemple le cas de plastique qui sont souillées par des restes de déchets alimentaires ces applications pourraient être réalisée en plastique bio-sourcées est compostable dans ce cas, elle pourrait être valorisé industriellement avec les biodéchets et donc contribuer à l'augmentation du pourcentage global de plastique recyclé en son temps des flux de recyclage mécanique, la loi impose le tri à la source et la valorisation des biodéchets à l'horizon 2023 je salue ce dispositif, qui malheureusement ne se suffira pas lui-même cette valorisation passera en note entre autres par le compostage sur site qui permet d'obtenir un compost propres permettant un apport au sol de qualité et favorisant ainsi son acceptabilité par les agriculteurs, je reconnais que le développement de cette filière industrielle est amorcée mais il reste très insuffisant en France aujourd'hui pour atteindre les objectifs réglementaires de valorisation des biodéchets qui sont fixés, alors que le gouvernement français a reconnu la pertinence de plastique bio-sourcées compostable dès le vote de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 et plus récemment dans le pacte emballage que fait-il alors pour en favoriser le développement à l'évidence, peu de choses, madame la ministre vous passer par pertes et profits les milliards investis en R&D et les emplois créés par la filière française et européenne qui jouit pourtant d'une avance technologique considérable sur ses innovations, véritable fer de lance de la bio-économique, croyez-vous que notre pays puisse supporter une telle erreur d'appréciation, une telle erreur dans le choix économiques du gouvernement, madame la ministre, que comptez-vous faire pour développer la filière de compostage et celle des plastiques bio-sourcées est compostable qui contribueront à une amélioration significative des taux de valorisation des plastiques elles lutteront contre une pollution galopante que nous pourrions stoppée, il s'agit de courage politique alors oser et nous vous suivrons. Alors vous l'avez dit, en 2002, Jacques Chirac a dit la maison brûlée et nous regardons ailleurs, c'était l'époque où, où les mots suffisaient où maintenant, hé bien, il nous faut nous salir les mains et rentrer dans le dur et c'est là que les choses deviennent compliquées et que parfois, nous sommes dans des situations relativement paradoxal, hé bien c'est le cas des plastiques compostables. Force est constater, et nous avons là une évaluation, notamment de la LTE CV qui avait préconisé une évaluation de l'utilisation notamment des plastiques compostables et fort cette cassette et qu'elle pourrait être plus positive cette évaluation, c'est-à-dire pour le dire très simplement, ça fait partie des effets un peu indésirables de ce type de méthode, c'est pour ça, c'est Très concrètement, beaucoup des plastiques dits biodégradables en réalité ne le sont pas, et c'est pour cette raison-là que bien souvent, je parle et je préfère dire que je préfère supprimer dans la mesure du possible, les classiques du quotidien, de façon à lutter contre la pollution plastique est-il changer et transformer nos modes de production et de consommation, en amont, il faut cesser de considérer que nous pouvons systématiquement trouver une alternative sans jamais changer nos modes de vie, de production, de consommation, c'est bien ça, un des objectifs, cela dit, je ne nie pas qu'il existe des plastiques bio-sourcées qui soient, eux, utile, efficace, là encore, il nous faudra veiller à une chose, c'est que le développement de ces pratiques bio-sourcées ne se fasse pas au détriment de la nature. C'est pour ça que je préfère privilégier en 1er, les changements de comportement et l'autre changement économique d'autre part, vous avez à très grande remet raison les biodéchets, là aussi, on en retrouve encore beaucoup trop dans nos poubelles, ce qui revient finalement dans le meilleur des cas à incinérer de l'eau, c'est bien paradoxal et c'est totalement intolérable, c'est une question qui est très difficile qui est épineuse, là aussi, parce que elles, elles demandent des changements de comportement profond et des consommateurs et de tout le système, c'est pour ça que nous avons et j'ai demandé à Alain Maroua de travailler sur ce qu'on appelle un pacte de confiance, pardon, avec l'ensemble des acteurs de cette filière des biodéchets pour trouver des solutions et si on parle de pacte de confiance, c'est bien parce que la confiance, c'est la monnaie la plus utile dans ce système-là, pour développer un système de collecte des biodéchets qui soit réellement efficace, encore longue, les changements sont profonds et nous aurons besoin de l'ensemble des sénateurs pour nous aider à travailler main dans la main avec les collectivités locales avec nos concitoyens, pour trouver des solutions pérennes et efficaces. La parole est à monsieur Guillaume Chevrolet pour le groupe, les républicains. Merci monsieur le président de la la ministre la question du recyclage des plastiques hors emballage, soit 60 pourcent des volumes utilisés dans des produits de consommation courante est très complexe du fait de la variété des plastiques. De la variété de leur utilisation et de celle des additifs ou substances dangereuses ajouter car il n'y a pas un mais des plastiques et c'est là où mon avis, le point de vigilance au risque de tuer l'économie circulaire en effet si on réutilise ses plastiques pour l'utilisation qu'ils ont à l'origine, il n'y a pas de problème, mais si on les mélange avec d'autres, en vue de diluer les éléments dangereux qu'ils contiennent, il y a une perte de traçabilité et ça peut présenter un risque pour la grande majorité des déchets plastiques qui sont issus des jeux, des équipements sportifs, des véhicules, par exemple, sur toutes ces filières, il est nécessaire de tourner en boucle fermée si on veut éviter un risque sanitaire majeur la question de la traçabilité est fondamental : il faut absolument empêcher tout risque de dilution, le vrai enjeu, c'est de ne pas remettre dans des produits manufacturés des substances dangereuses qui risque de détruire la confiance des consommateurs dans les produits issus du recyclage, il vaut mieux, me semble-t-il, se priver d'un peu de valorisation pour conserver celle qui est pertinente, efficace et assurer la pérennité, voici le point de vigilance que je souhaitais vous présenter le recyclage de tous les plastiques peut être dangereux, qu'une telle ambition n'est pas encore possible étant donné qu'il n'existe pas encore de modèle économique viable en effet jusqu'à présent, le plastique étaient exportés en Chine qui a récemment fermé ses frontières, on n'a pas encore développé en Europe les unités qui permettent de bien trier et de recycler et de valoriser il faut donc boosté les filières de recyclage, quelles sont les ambitions et leviers d'action du gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénat. Peur Chevrolet alors tout d'abord, première chose avant tout quand on parle et quand il s'agit de la santé

il est fondamental que ce c'est, c'est une véritable priorité et c'est d'un niveau d'exigence que nous assumons totalement et sur lequel nous ne reviendrons jamais maintenant vous parlez et vous mentionnez la question et je crois comprendre, dans votre question est aussi celle de la possibilité de recycler quand il y a plusieurs matériaux classiques, par exemple, ou plusieurs matériaux différents dans un dans un un emballage ou dans un produit, hé bien sachez que ce que nous voulons faire par toute une série de mesures je cite par exemple le bonus-malus sur les plastiques en fonction de leur quantité de d'incorporation de classique recyclé, je pense, par exemple aussi à à l'utilisation de différentes modulations d'éco-conception, bref, toute une série de mesures que je pourrais détailler, on pourra en parler si vous voulez, monsieur le sénateur, mais j'ai malheureusement que 2 minutes. Pour répondre, qui vise en fait peu à peu et le plus rapidement possible à créer des incitations pour faire en sorte que les plastiques qui ne soit pas recyclables souhaite éliminer peu à peu du système et encore une fois le plus rapidement possible afin de développer, de permettre l'éco-conception l'éco-conception des produits et donc un recyclage qui soit plus facile, recyclage, certes, mais niveau de qualité niveau sanitaire égal et si ce n'est toujours supérieure puisque c'est notre priorité, mais puisque vous parlez de traçabilité et de santé aussi des Français bien très imprécise que beaucoup de micro-classique se retrouve. Partout dans la nature, il songe ou s'agit donc d'une priorité, celle de changer notre modèle économique, nos façons de consommer et de produire et de développer toute une palette de solutions technologiques pour éviter que ces microplastiques se trouve dans l'environnement et in fine et malheureusement dans nos assiettes. Merci 30 secondes supplémentaires chers collègues. davantage de recettes l'habilité et puis aussi agir sur des produits qui soient démontables et pour faciliter le recyclage et lutter contre l'obsolescence programmée merci. La parole était à madame Anne-Marie Bertrand pour le groupe, les républicain pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il est indéniable que l'utilisation croissante du plastique depuis les années 60 contribuent au changement climatique et implique ainsi la biodiversité quand celui-ci restait nécessaire, nous devons alors développer de nouveaux types d'emballages, c'est notamment le cas dans les Bouches-du-Rhône, où une entreprise comme si rap développe une gamme d'emballages biodégradables et compostables ceci afin de répondre aux exigences aussi forte que légitime des consommateurs. Vous le savez, ces avancées exige d'importants investissements, ces investissements peuvent néanmoins être porté par nos entreprises, si nous prenons le soin de ne pas les fragiliser et c'est sur ce point que je souhaitais vous alerter le pacte national sur les emballages plastiques et susceptible, me semble-t-il, de fragiliser des entreprises volontaires, notamment celle qui aujourd'hui produisent des emballages en polystyrène expansé alors même que celles produisant des emballages avec d'autres, polystyrène, nous ne sommes pas concernés par cette interdiction, et que ce polystyrène expansé et tout aussi recyclables ne vous semblerait-il pas judicieux d'exalter pour une période donnée, les entreprises proposant une gamme d'emballages écologiques afin d'encourager toujours plus ces de 6 humain et ainsi préserver des emplois mieux d'en créer sur notre territoire, hein, je vous remercie. Madame le Ministre. Si monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bertrand. Je vais vous répondre directement enfin cash comme on dit parfois vulgairement alors que je ne tiens pas allez être bien sûr mais le polystyrène expansé ne se recycle pas, ne se recycle pas, en tout cas pas à des coûts qui serait acceptable pour les industriels ou les consommateurs ou même l'environnement en France il y a tout simplement pas de filière de recyclage en France, alors après c'est une question de choix, nous pensons, nous avons fait des études et nous vous affirmons très clairement que ce n'est pas une filière qui pour le moment est dans l'État de se développer en France et il y a des priorités fondamentalement importante aussi sur d'autres résines et toute une palette de mesures que j'ai l'occasion détaillé à plusieurs reprises à vos collègues sénateurs toute une palette de mesures qui permettront d'accélérer le développement de hein l'utilisation plus importante des résines plastiques qui elle se recycle auraient plus facilement et, deuxièmement, de concevoir aussi des emballages qui soient recyclables beaucoup plus facilement et donc constitué de résineux unique par exemple le bref c'est aux industriels d'être créatif, nous leur fixons des objectifs ambitieux. Nous au sont aussi des objectifs ambitieux aux éco-organisme aux collectivités, aux citoyens, bref l'écosystème se développe et mise en place de façon à ce que nous puissions accélérer l'éco-conception le recyclage, la transformation d'un système de production et de consommation, et pour cela, il faut prendre des priorités. Les décidé les assumer certains de vos collègues, parlait de courage en politique, hé bien je crois que c'est le cas et je peux vous dire que il n'y a pas de filière de police de recyclage de polystyrène expansé en France, je vous remercie. Comprenez bien que les salariés de ces entreprises ont pleinement conscience de la nécessité de changer de modèle de consommation consommateurs salariés citoyens sur les mêmes personnes nous devons tous pouvoir à défaut d'un être signataire adhérer à ce pacte, bref cette transition écologique et l'affaire de tous et doit le rester. Merci la dernière question sera posée par votre collègue Cyril va pour le groupe, les républicains pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, d'après la Banque mondiale, 2 milliards de tonnes de déchets sont produits par an dans le monde dont 33 pourcent ne seraient pas traités correctement le plastique est l'une des matières qui pose le plus de problème étant difficiles à recycler et ça a été rappelé, vous avez évoqué les chiffres en France pour 2016, au niveau mondial, ce sont 242 millions de tonnes de déchets plastiques qui ont été produits or seuls 9 pourcent sont recycler le plastique hein mettant en moyenne 4 siècles à se dégrader et des exemples récents montrent que même le plastique dégradable, ne le sont pas vraiment la majorité du plastique fabriqué par l'homme, se trouve dans la nature dans les décharges sauvages dans les océans, causant de gros dommages pour la biodiversité marine, ça a également été rappelé si certains emballages plastiques ne se recycle pas, c'est essentiellement en raison du coût, soit parce que les produits sont jugés trop léger ne contenant pas assez de matière pour qu'le respecte le recyclage soit rentable, exemple des pot d'yaourt en soi parce que le recyclage est jugé trop complexe, c'est le cas des jouets, par exemple, nous devons réussir à recycler tous les emballages, y compris les pot d'yaourt les barquettes ou les sacs plastique et je rejoins vos propos sur les solutions innovantes, élu de Haute-Savoie, vous êtes venue madame la ministre, ce département est très touristique et je suis fortement sensibilisé à cette problématique de la lutte contre la pollution plastique que nous pouvons voir dans nos montagnes et le lac, mais il n'y a pas que le recyclage en amont du recyclage, il reste beaucoup à faire, la lutte conte le sur-emballage ne semble ainsi très importante le suremballage tous 9 produits sur 10 Éric les consommateurs, nous devons aussi lutter contre le jetable, tous ces produits à usage unique, qui ne sont pas indispensables et sur lequel il y a des alternatives, enfin j'aimerais soulever l'importance de la sensibilisation des enfants à l'école, l'éducation à l'environnement est primordial pour favoriser la prévention des déchets : les bons gestes de recyclage peuvent être appris dès le plus jeune âge, des supports pédagogiques ou équipements pour sensibiliser enfants recyclage existe, j'en avais acheté quand j'étais maire, il pourrait être développé davantage l'État pourrait-il un s'engager, éduqué à l'environnement dans tous les établissements scolaires sensibiliser la jeunesse au développement durable et notamment au recyclage me semble être une voie intéressante et le pont éduqué à leur tour leur entourage, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, elle va. Alors, plusieurs réponses à votre question et je vous remercie de votre souci sans pour la lutte contre la pollution, plastique et, plus globalement, celle qui finit bien trop souvent, comme vous l'avez souligné dans la nature alors l'objectif du gouvernement, il est triple : il est d'abord et avant tout de supprimer toute classique qui est inutile vous avez parlé de sur-emballages, vous avez parlé aussi de plastique jetable, hé bien c'est dans ce sens-là, exactement, que nous allons nous avons supprimé déjà toute une série de place de plastique à usage unique et dès l'année prochaine, ce seront les gobelets par exemple en plastique et les couverts en plastique qui seront. Interdit, nous voulons aussi d'autre part favoriser et développer le recyclage et cela de façon massive en permettant notamment et en donnant et en mettant en place toute une série d'incitative d'incitation pardon pour favoriser l'éco-conception, mais aussi pour permettre de mieux collecter ces plastiques afin qu'ils soient recyclés qu'ils rentrent dans cette boucle. Vertueux, j'ai parlé d'appel à manifestation d'un d'intérêt qui ont été lancés de façon à développer et à identifier de nouveaux systèmes de collecte innovants, comme par exemple des systèmes de consignes enfin troisièmement, ce que nous voulons faire c'est encourager très massivement le réemploi le réemploi d'objets en plastique qui pourrait l'être nous n'avons pas va la loi qui va arriver d'ici à l'été pour commencer à agir, nous avons lancé un pacte sur les emballages plastiques qui réunit 13 entreprises qui ont pris des engagements très significatives pour réduire drastiquement le suremballage et commercialiser des produits qui des produits qui soient entièrement fait à partir de matières premières recyclées d'ici 2025, ça c'est l'objectif de ce pacte national avec des zoos ONG qui verront vérifierai vérifier l'avancée de ce pacte de la mise en oeuvre de ce pacte. Enfin, la sensibilisation des enfants dans les écoles, c'est absolument fondamental, j'ai rencontré moi aussi des mères qui ont mené des actions tout à fait remarquables aux côtés des écoles dans leur municipalité, je crois que c'est à encourager le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le fait est activement, est en train de réfléchir à des mesures à mettre en oeuvre, j'ai été moi-même en visite pendant 2 jours dans l'Ain, sur le terrain près et à côté de ce pôle de compétitivité sur le plastique pour voir très concrètement ce que nous pourrions faire et nous sommes en train d'y travailler, nous aurons l'occasion d'en reparler, je serais ravi d'apprendre aussi et de d'apprendre de vous et de savoir ce que vous avez fait

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il nous revient donc au nom de mon groupe de conclure ce débat fort utile qui fut riche d'enseignements, celui-ci aura permis de souligner, s'il en était encore besoin, l'urgence de la situation et donc la nécessité d'agir pour éviter une catastrophe écologique et sanitaire, comme nous l'a rappelé avec beaucoup d'émotion, notre collègue Angel près ville rappelons les chiffres selon un rapport de WTF de mars 2019 il a été produit dans le monde, autant de plastique entre 2000 et 2016 qu'entre 1950 et 2000 plus de 310 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générés en 2016, dont un tiers se sont retrouvés dans la nature 150 millions de tonnes de plastique se trouve dans les océans, et si rien n'est fait, la production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de plus de 40 pourcent d'ici 2030 et la quantité dans l'océan pourrait ainsi doubler en 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer, rappelons également que la France a encore de gros progrès à faire en matière de recyclage, puisque seulement 22 pourcent des plastiques sont recyclés, contre 31 pourcent au niveau européen, une prise de conscience semble cependant avoir lieu dans l'opinion, les discours se multiplient pour bannir les plastiques superflue et réduire l'usage unique, une sorte de plastique bashing se développe de plus en plus avec lequel, comme l'a indiqué notre collègue Patrick Chesnais, il faut néanmoins prendre ses distances, des mesures ont certes été prises par le gouvernement, et vous venez de le rappeler, Madame la Ministre, le pacte national sur les emplettes Balaj plastique que vous avez signé le 21 février dernier va dans le bon sens, les entreprises et les grands groupes signataires s'engagent en effet à arrêter l'utilisation du PVC dans les emballages ménagers commerciaux et industriels d'ici 2 1000 22 et à éliminer les emballages plastiques problématique ou inutiles d'ici 2025, à commencer par le polystyrène expansé le pacte vise également à atteindre 60 pourcent d'emballages plastique effectivement recyclés d'ici 2000 22 et incorporé en moyenne 30 pourcent de matière plastique recyclée dans les emballages, mais ces mesures semblent insuffisantes, eu égard aux enjeux l'approche volontariste sur laquelle repose le pacte et l'absence de contraintes risquent d'en limiter les effets une il ne donne pas non plus d'objectifs chiffrés quant à la réduction de la quantité d'emballages à la source par ailleurs, le recyclage ne peut pas être la seule solution apportée au problème, d'abord parce que le recyclage du plastique n'est pas infinie, contrairement aux Verts, au papier ou métal et plastique ne se biodégradable pas et parce que le meilleur déchet, c'est avant tout et ça a été rappelé, celui qu'on ne produira pas, il faut intervenir à la source, le plus possible en produisant le moins de plaintes l'aspect international du problème doit également être pris en compte, s'il est vrai que les principales sources de plastique des océans sont les pays en voie développement de nombreux pays dont la France exporte eux aussi une partie de leurs déchets plastiques vers ces régions et c'est aussi en raison du caractère transnational du phénomène que de nombreuses organisations demandent la mise en place d'un traité international juridiquement contraignant pour enrayer cette pollution, je pense qu'il y a sur ces bancs, un large consensus et que Madame la ministre nous souscrivons aux 3 piliers que vous avez énoncé la suppression des plastiques inutile le recyclage de 100 pourcent des plastiques utile et la préparation par l'innovation de l'après-plastique alors oui, nous souhaitons que ce débat est et permis d'enrichir la feuille de route sur l'économie circulaire et vous pouvez compter sur notre application sur celle des collectivités locales pour sa mise en oeuvre, c'est sans doute toute une diversité de mesures cohérentes et ambitieuses qu'il faut mettre en oeuvre des mesures certes à la fois colère si TIW mais aussi des mesures incitatives, mais au-delà, et vous avez parlé, Madame la ministre de la force de l'outrance de notre société de consommation, c'est donc un autre modèle de consommation et de développement que nous devons promouvoir et sachez que nous prendrons toutes nos responsabilités dans ce domaine, je vous remercie. Merci. Nous voici au terme de ce débat, mes chers collègues, je vais lever la séance, ordre du jour du jeudi 2 mai 2019 de 14 heures 30 à 18 heures 30, proposition de loi résiliation des contrats de complémentaire santé ensuite propositions de lois et de loi organique sur la clarification du col électorale, puis de 18 heures 30 à 20 heures et de 21 heures 30 à minuit, proposition de loi affectation des avoirs issus de la corruption transnationale, proposition de loi reconnaissance du Crime d'la séance est levé.